La séance est ouverte, en application de l'article 28 de la Constitution, la session ordinaire 2022 2023 est ouverte le compte-rendu intégral de la séance du jeudi 4 août a été publié sur le site internet du Sénat : y a-t-il des observations non le procès verbal est adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Louis Grillot, qui fut sénateur de la Côte-d Or, de 1998 à 2008 Michel doublé qui fut sénateur de la Charente-Maritime de 1989 à 2014 Jacques Mahéas, qui fut sénateur de la Seine-Saint-Denis de 1995 à 2011. J'informe le Sénat que conformément à l'article 8 de notre règlement le 11 septembre dernier Monsieur Jean-Marie Janssens est devenue membre de la commission des affaires sociales, madame daphné Ract-Madoux est devenue membre de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, la conférence des présidents a inscrit le prochain débat d'actualité à l'ordre du jour du mercredi 5 octobre à 16 heures 30 après concertation avec les groupes politiques ce débat porterait sur proposition de monsieur le président du Sénat sur le thème suivant atteinte aux droits des femmes et aux droits de l'homme en Iran sous forme de discussion générale. Y a-t-il des observations, il en est ainsi décidé. La parole est à monsieur Jean-Pierre Sueur pour un rappel au règlement. Merci madame la présidente, madame la présidente en 2017 Monsieur Emmanuel Macron, président de la République a déclaré que lorsqu'un ministre était mis en examen et lui paraissait qu'il devait quitter le gouvernement d'ailleurs un président, un précédent garde des Sceaux a été amenée à quitter le gouvernement, je constate par ailleurs que les avocats du présent, garde des Sceaux, tiennent des propos mettant lourdement en cause les plus hautes autorités de la magistrature. S'il vous plaît. Et notamment monsieur le procureur général près la Cour de cassation, dans ces conditions, on peut se demander comment le garde des Sceaux peut être garant de l'indépendance de la justice, enfin, je constate, mes chers collègues, qu'il est tout à fait possible dans l'état actuel des choses, que monsieur le garde des Sceaux soit conduit à contribuer à la désignation du prochain procureur général près la Cour de cassation qui sera ou qui serait son accusateur, dans ces conditions j'en viens au rappel au règlement, monsieur J'ai l'honneur, madame la présidente, de vous demander, au nom du groupe socialiste de vous demander de bien vouloir saisir de ces questions, monsieur le président du Sénat et de lui demander de demander à Madame la première ministre de venir devant le Sénat pour s'exprimer sur la position du gouvernement sur les faits que je viens de citer et sur les conditions dans lesquelles dans ces dans cette situation-là sera garantit l'indépendance de la justice, je vous remercie, Ces données de votre rappel au règlement. Et votre demande sera bien entendu transmise à monsieur le président du Sénat. L'ordre du jour appelle le débat sur les états généraux de la justice, la parole et tout d'abord à l'orateur du groupe, qui a demandé ce débat Monsieur François Noël Buffet pour le groupe. Les républicains et pour huit minutes chers collègues.

Madame la présidente. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je suis heureux que de ce débat au Sénat inscrit à l'initiative du groupe Les Républicains sur les suites du rapport du comité des états généraux de la justice qui a été remis au président de la République le 8 juillet dernier je vous dans quelques instants pour quitter l'estrade sur laquelle je suis. Parce que. Une impression de hauteur un peu étonnante voilà c'est mieux comme ça, merci de votre patience, il est le fruit d'un travail approfondi auquel d'ailleurs, j'ai eu l'honneur de participer, entre le mois d'octobre 2021 et le mois d'avril dernier, il faut rappeler que ces états généraux de la justice ont été initiées par le président de la République, suite au cri d'alarme, je crois que l'on peut employer ces mots assez forts, d'une part de madame Chantal Arens à leur première présidente de la Cour de cassation et de Monsieur, François Molins ce procureur général près de cette même cour sur la situation critique de la justice française. Plus de 7000 magistrats ont ensuite signé une tribune dans la presse, en réaction aux suicides dramatiques de l'une des l'heure qu'une de leurs collègues, dénonçant leurs conditions de travail et la perte de sens de leur métier, ce qui est naturellement sans précédent, le malaise dans la justice, c'est une réalité, on ne peut pas le contester la perte de confiance des citoyens dans son action, aussi, comme l'a montré l'Agora de la justice, organisé par le Sénat le 27 septembre 2021.

cette réalité, le Sénat, la mise en lumière depuis plusieurs années, tout en faisant des propositions qui n'ont pas toujours d'ailleurs reçu un accueil favorable des chancelleries, je dirais, car ce n'est pas récent, je citerai les 3 principaux : rapport de la commission des lois sur le sujet, d'abord en 2017 5 ans pour sauver la justice au terme d'une mission d'information conduite par notre collègue Philippe Bas avec plusieurs co-rapporteur je me plais à citer Jacques Bigot François Zocchetto Madame Herman ici présente notre collègue, et Madame, Esther Benbassa, en 2019 la justice prud'homale au milieu du gué conduite en commun avec la commission des affaires sociales et dont Agnès Canayer Nathalie Delattre et Pascale Gruny, madame la présidente, fuir les rapporteurs et en 2021, le droit des entreprises en difficulté à l'épreuve de la crise non François Bonhomme et Thani Mohamed Soilihi fut rapporteur nos rapports budgétaires également suivent attentivement chaque année la situation de la justice et ont souvent alerté sur ces difficultés concrètes, il est donc heureux de retrouver de nombreux points de convergence parmi les constats et propositions du rapport des états généraux, avec les travaux du Sénat, je pense par exemple à la mise en place d'un tribunal des affaires économiques, ou à l'orientation à Benicio des affaires devant le conseil des prud'hommes, la commission des lois, entendu le 21 novembre dernier Jean-Marc Sauvé, président du comité des états généraux, ainsi que Madame Arras Monsieur menacé Monsieur Gavaudan, président du Conseil national des barreaux, je retiens parmi les points évoqués, outre l'augmentation des effectifs, la nécessité de mettre en place une véritable politique civile avec un renforcement de la première instance, là encore, le Sénat avait déjà pointé ce besoin véritable justice du quotidien, qui représentent 60 % du contentieux judiciaire, alors que les projecteurs sont principalement braqués sur la justice pénale en 2019 la justice civile, représentée en effet plus de 2000 Lyon 200000 décision 2 1000000 200000 décisions pour la seule justice civile tandis que la justice pénale n'en représentait que 800000 ces chiffres sont ceux de 2019 alors qu'en 2020, évidemment, la crise du Covid ne nous a pas permis d'avoir un reflet réel de la situation. Pour réformer, il importe que le ministère Monsieur le ministre accepte de changer la méthode en agissant de manière systémique au service du justiciable du d'un meilleur fonctionnement en évoluant en amont les conditions pratiques nécessaires à la réussite de ces réformes et finalement que l'on sorte d'une approche strictement normative à cet égard le niveau d'exigence des études d'impact doit être revu pour vraiment prendre en compte la réalité du terrain trop souvent la réforme présentée par le gouvernement ont volontairement ignoré les effets réels induit sur l'organisation des juridictions, le travail des juges et, au final, les justiciables eux-mêmes ce type d'approche doit impérativement être abandonnée, d'ailleurs, malgré les efforts financiers accomplis ces dernières années, Monsieur le Ministre. La politique numérique tarde à produire des effets concrets sur le terrain où les équipes se plaignent encore de dysfonctionnements, notamment du à l'impréparation de nos réformes législatives il faudrait en outre nous discipliner collectivement pour modifier les textes que lorsque cela est strictement nécessaire est-ce un voeu pieux, je ne le crois pas, les juridictions sont épuisés par les modifications incessantes des règles, et cela vaut tant pour la loi que pour les textes réglementaires, les 12 sénateurs de la commission des lois ont pu le constater lors de nos stages jeu Dixie lors de leur stage en juridiction cette année au sein des tribunaux judiciaires de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Lille de Rouen ou encore de Marseille, il faut donc désormais s'attacher à la mise en oeuvre des propositions qu'il s'agisse des moyens de l'organisation et du fonctionnement de la justice ou des réformes législatives je crois pouvoir dire à cette tribune que le Sénat dans son entier, il veillera au final, le rapport des états généraux de la justice, c'est un rapport plutôt pragmatique et opérationnelle, il donne les clefs pour mieux faire fonctionner, je le crois l'existant plutôt que d'inventer de nouveaux systèmes souvent de caractère illusoire la mobilisation des magistrats, mais aussi celle des greffiers qui sont moins dans la lumière, évidemment nous oblige, ils sont pour la très très grande majorité et tous sans doute dévoué au quotidien et à la continuité de l'institution judiciaire, il suffit de regarder ce qui s'est passé pendant la 2ème. Crise du Covid ou ce qui se passe aujourd'hui, compte tenu, certaines situations et de travaux supplémentaires qu'ils doivent assumer sans forcément avoir des moyens supplémentaires malgré difficultés nous serions d'ailleurs, je le crois, collectivement, coupable de ne pas leur apporter les moyens de leur travail, bien sûr, le débat ne se résume pas simplement à ceux-là, il y a un moment. Des choix politiques à faire sur des stratégies de justice, il y a un continuum entre la police, la justice et bien sûr la pénitentiaire pour la partie pénale mais en toute hypothèse, la justice est en crise, la justice civile l'de façon très caractéristique, la justice pénale peine surtout je le crois, par la problématique liée à l'exécution des peines à la rapidité de celle-ci et à l'efficacité de celle-ci mais je ne crois pas sincèrement que nous devions à ce stade, revoir encore et encore notre législation certes sur un certain nombre de points particuliers, sans doute, mais je crois qu'il vaut mieux se concentrer sur les moyens que nous mettons à disposition de nos magistrats et de nos greffier, qu'ils soient numériques, qu'il soit humain ou qu'il soit dans une organisation plus systémique de façon à privilégier la réussite de cette mission, et chacun est bien conscient ici que ce lieu de de Rennes essaye de résoudre les conflits entre la société les délinquants ventre des particuliers est un lieu absolument essentielle au fonctionnement de notre vie tout court et de la vie sociale en particulier, c'est un lieu d'apaisement, la justice, contrairement à ce que l'on imagine, c'est un lieu dans lequel les conflits privés doivent trouver des solutions qui apaise les partis qui finissent par accepter les décisions rendues, c'est absolument fondamental aujourd'hui tous les magistrats que nous rencontrons tous les greffiers se rendent compte ou s'inquiète se pose même la question de leur propre utilité voire de leur reconnaissance au sein de nos institutions, c'est un bien précieux que notre justice, mes chers collègues, et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, nous attendons cet après-midi dans. Ce débat qui s'organise un certain nombre de questions, notamment peut-être sur le calendrier de mise en oeuvre des conclusions des états généraux et et des concertations qui sont prévues quand même, vous avez déjà engagé mais aussi quel type de mesures réglementaires ou législatives souhaitez vous engager et enfin, on nous parle ou on entend parler d'un projet de loi de programmation. Sinon, pour la justice à Caen ce projet sur. Le pupitre du Sénat merci.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs. Je suis tout particulièrement heureux de revenir. Devant vous, alors que s'ouvre la première session ordinaire de cette nouvelle législature. Je souhaite poursuivre avec chacun d'entre vous, le travail de coconstruction qui a guidé mes relations avec le Sénat depuis mon arrivée à la chancellerie. C'est pourquoi, dans le cadre des états généraux qui nous réunissent aujourd'hui. Je veux faire en sorte que les réformes aux indispensable se fasse dans le plus large consensus, c'est le principe même de ces états généraux, impulsée par le président de la République à la demande des 2 plus hauts magistrats. De notre pays qui constitue par ailleurs un exercice démocratique absolument inédit avec près d'un 1000000 de contributions citoyennes. Alors que le rapport de très grande qualité issus de ces états généraux de la justice, a été remis au président de la République par le président en juillet dernier, je conclus actuellement la dernière phase de concertation de tous les acteurs du monde judiciaire et je veux ici un instant saluer le Sénat dans son ensemble. Et, en particulier, votre président Gérard Larché, ainsi que votre président de la commission des Lois François-Noël Buffet qui était d'ailleurs membre du comité des états généraux pour l'engagement qui est le leur, en matière de justice mais c'est sincère, monsieur Karoutchi. Pour l'engagement qui est le leur, en matière de justice. Que ce soit dans le vote des Budgets. Qui sont bons. Il faut bien l'admettre, ou bien dans les propositions formulées je, je pense par exemple. Aux Zagora de la justice, en passant par l'indispensable travail législatif menée de concert, je ne compte plus les fois où le gouvernement et le sénat ont joint leurs forces avec l'Assemblée pour faire progresser notre justice mais vous le savez, ce travail n'est pas fini, loin s'en faut, c'est pourquoi, comme je l'ai annoncé je présenterai dans les semaines qui viennent. à nos concitoyens. Ainsi qu'au Parlement, bien sur un plan d'action détaillé pour réformer et améliorer le service public de la justice avec un impératif, la rendre plus plus protectrice, plus rapide, plus efficace, plus proche de nos concitoyens, ce plan qui, je vous rassure, reprendra un certain nombre de propositions sénatoriales. Comme celle concernant les recrutements à venir ou encore la réflexion autour d'un tribunal des affaires économiques se déclinera à travers tous les leviers dont nous disposons, l'objectif sera pour moi d'aller vite, c'est pourquoi tout ce qui pourra être fait par voie réglementaire, le sera et ce dans les plus brefs délais, je pense par exemple à la matière civile ou encore à l'organisation propre du ministère. Je vais néanmoins vous répondre en quelques points concernant les premières priorités qui font déjà consensus premièrement. Nous allons poursuivre le renforcement inédit : la justice en termes humains et financiers, car on ne résout pas 20 ou 30 ans d'abandon politique humains, financiers en un claquement de doigts, vous le savez, le budget de la justice pour 2023 ce rare si vous l'acceptez, pour la 3ème fois consécutive en hausse de 8 %. C'est ça nous laisse peu à peu entrevoir l'horizon d'une justice de qualité que tous les acteurs du monde judiciaire, mais surtout les justiciables appellent de leurs je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'une première recommandation et non des moindres, du rapport Sauvé sera suivie nous embaucherons au moins 1000 500 magistrats et 1000 500 greffier sur le quinquennat. Il s'agit là du plus grand plan d'embauche de toute l'histoire des services judiciaires après le volet réglementaire budgétaire organisationnel, les arbitrages issue des concertations en cours prendront corps à travers une ambitieuse loi de programmation pour la justice, sur la période 2022 2027. Fidèle à la démarche de coconstruction qui est la mienne, le Parlement sera très étroitement et j'insiste consultés en amont des débats et aura toute la place qui lui revient au moment de l'examen de ce texte, ces discussions viseront à nous accorder sur l'ampleur des réformes législatives de la justice que nous aurons apporté qu'elle soit pragmatique programmatique ordinaire organique ou même constitutionnels. Si la loi de programmation permettra d'inscrire dans le marbre les recrues les recrutements massifs de magistrats, de greffiers, mais aussi. 2 contractuel de personnels pénitentiaires, elle aura également vocation à transposer dans la loi et de façon concise les principales propositions. Qui auront fait, pour la plupart déjà consensus en matière pénale. Mes priorités. à savoir une réponse ferme et systématiques ont été fixées par la circulaire du 20 septembre dernier je pense par exemple à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et aux mineurs, lutte contre la délinquance du quotidien et la criminalité organisée, lutte contre le terrorisme, lutte contre les atteintes à l'environnement, mais aucune politique pénale ne pourra efficacement prospérer sans la simplification de la procédure, réclamée par l'ensemble des acteurs du monde judiciaire, le président de la République s'y est engagé et j'aurai donc vocation vous proposer une méthode consensuelle et une feuille de route claire pour qu'ensemble, si vous en êtes d'accord, nous puissions mener ce chantier législatif colossal, la nécessité de cette réforme fait l'objet. D'un consensus des forces de l'ordre aux magistrat en passant par les avocats. Politique pénale ne peut exister sans politique pénitentiaire volontariste et c'est pourquoi nous poursuivons le grand plan immobilier immobilier pénitentiaire, avec la création de 15000 places d'ici 2027 afin d'assurer la réponse pénale d'améliorer les conditions de travail des agents pénitentiaires, ainsi que les conditions de détention qui nous indigne trop souvent. Sur le volet réinsertion. Qui, je le répète, est absolument indissociable du volet répressif, nous poursuivons la hausse des moyens alloués, ainsi que la mise en oeuvre du contrat du détenu, travailleurs et les remises de peine conditionnée à l'effort. En matière civile, nos objectifs sont les suivants. Poursuivre sans relâche nos efforts de résorption des stocks. Les stocks. Mesdames et messieurs les sénateurs, en matière civile, ont diminué de plus de 28 % au niveau national, c'est absolument considérable, il faut lancer à l'échelle nationale, une politique ambitieuse de l'amiable, une décision de justice oh construite est une décision mieux acceptée. Il faut simplifier le parcours juridictionnel du justiciable qui ressemble, il faut le dire bien souvent un parcours du combattant. Le temps imparti ne me permet pas un exposé complet, mais les questions qui viennent me permettront d'approfondir d'expliciter mon projet qui tient difficilement vous me le concéderaient en 8 minutes. Je pense notamment, parmi d'autres sujets cruciaux questions absolument essentielles que sont la transformation numérique du ministère. Absolument essentiel est cher à votre collègue. Madame la sénatrice veut rien ou encore la justice économique et commercial si importante face à la crise, c'est Sans aucune polémique à l'attention de monsieur le sénateur sueur. Pour lui dire que mes avocats expriment ce qu'ils estiment nécessaires à ma défense. Deuxièmement. Madame Élisabeth Guigou pour qui j'ai le plus profond respect. A été chargé d'un travail très important sur la présomption d'innocence.

Et le gouvernement, monsieur le garde des Sceaux dispose pour répondre d'une durée équivalente, c'est-à-dire deux minutes le gouvernement s'ils le souhaitent, aura la faculté de répondent à une réplique pendant une minute et l'auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répondre pendant une minute. Je serai le gardien du temps, la parole est à monsieur Guy Bénard Roche pour le groupe écologiste solidarité et territoires donc pour 2 minutes maximum. Madame la présidente, monsieur le Ministre, les travaux de ces états généraux s'inscrivent dans le Costa partagé du de justice malade si vous marteler que jamais de gouvernement n'a autant fait pour la justice, les faits sont têtus et les chiffres d'augmentation de budget, peine à convaincre les acteurs du quotidien, magistrats, greffiers, ainsi que les citoyens qui, malgré des projets pour la confiance dans la justice, alors du mal à appréhender un système judiciaire souvent maltraitant le groupe a eu plusieurs fois l'occasion de regretter de trop nombreuses réformes n'étant dans l'adéquation, ni avec les attentes des citoyens ni avec des demandes de magistrats ou du personnel pénitentiaire, voir des réformes d'affichage dans les moyens nécessaires à leur bonne exécution au mieux ne suivent pas, au pire, ne sont même pas prévu, par exemple, les nouvelles prérogatives du juge de la liberté de la détention sans augmentation de leur nombre ou la généralisation des cours criminelles départementales avant de prévoir l'arrivée de nouveaux magistrats ces états généraux, eu le mérite de remettre sur la table de nombreuses discussions, y compris celle de redonner du sens à la peine pour favoriser la réinsertion, la peine doit favoriser la réinsertion de l'auteur et réduire les risques de récidive, à ce titre en dehors des effets positifs que cela pourrait avoir sur la population carcérale, l'idée de recentrer le juge d'application des peines sur ses missions premières pourrait s'accompagner d'une plus grande présence des services pénitentiaires de l'insertion et de l'approbation dans des juridictions, comme cela est proposé dans les états généraux de la justice, ma question est la suivante : l'activité en milieu ouvert des SPIP supérieur au nombre de personnes concernées qu'en milieu fermé, est encore trop méconnus que comptez-vous faire pour valoriser soutenir cette activité essentielle de la pénitentiaire dans les compétences ne cesse de croître. madame la présidente, mesdames, messieurs, monsieur le sénateur Ménard. Punir mais réinsérer. Punir et réinsérer, vous m'interrogez sur la situation des ces pipe alors d'abord en terme de de personnel c'est 1500 recrutements depuis 2018, ce qui a permis de diminuer le nombre de dossiers suivis par sacs chaque c'est pipe, on est passé de 80 dossiers 71

plusieurs avancées importantes passage en catégorie A revalorisation indemnitaire de 220 euros par mois en 2022 les des pipes ont bénéficié d'une revalorisation indemnitaire 3 millions en 2021 et 2022 je souhaite aller plus loin en 2023 la poursuite de la hausse des primes à hauteur d'un 1000000 d'euros, réforme du statut pour faciliter la promotion professionnelle revalorisation de leur rémunération indiciaire à hauteur de 1 virgule je le sénateur, vous évoquiez également le travail en milieu ouvert, s'il faut punir le délinquant et de protéger nos concitoyens avec la prison, l'émission réalisée par le pipe en milieu ouvert sont essentiels, politique volontariste en faveur des amateurs, je monte peines et des mesures alternatives à l'incarcération et menée par le ministère de la justice en 2023 la dotation correspondance élevé à 53 4 millions d'euros, soit une progression de plus 34 % par rapport à 2022 28 millions d'euros seront consacrés au placement sous surveillance électronique, le placement extérieur bénéficiera d'une dotation de 11 3 millions d'euros, soit un complément de de 5 millions d'euros destinés au relèvement du prix de la journée pour favoriser l'octroi de ces mesures, enfin la dotation allouée à la politique de réinsertion et de lutte contre la récidive se rapporter en 2023 à 122,5 millions d'euros.

Oui 28 secondes juste pour demander la précision suivante, hein, Monsieur le Ministre, les moyens que vous avez mis à disposition dans le budget 2023 permettra-t-il enfin la convergence du régime de rémunération des directeurs et directrices de service pénitentiaire d'insertion et de probation qui sont, qui n'ont pas bénéficié de mesures depuis de nombreuses années, avec ceux de la pénitentiaire aujourd'hui la revalorisation des ces pipes, fait que les des PIB, c'est-à-dire que les directeurs de ces services ont des carrières et des avancements de carrière qui les mettent au-dessous, au niveau salarial

c'est que il faudrait également veiller à augmenter la dotation budgétaire des spis pourquoi, parce que ceux-ci doivent pouvoir disposer de Budgets propres leur permettant de financer ou de participer au financement croisé de prise en charge par le milieu associatif de suivi intensif intensif et individualisé, vous savez qu'on ne peut pas y arriver sans ces accords croisés, il faudrait également augmenter les effectifs des ces pics je je comprends bien que vous avez dit qu'ils ont augmenté, mais vous savez qu'a ratio qui a été fixé le ratio, il a été fixé d'un agent pour 60 personnes suivies, vous avez vous-même dit qu'actuellement

Merci madame la présidente, constat sévère au bord de la rupture, état de délabrement avancé crise majeure, perte de sens, on ne compte plus les qualificatifs moribond pour décrire la justice au fonctionnement dans notre pays, le rapport du comité des états généraux, remis au président de la République le 8 juillet dernier a formulé une série de recommandations pour redresser le service public de la justice, il souligne que, renforcement des moyens financiers, humains et en matériel, les réformes resteront déconnectés de leur capacité d'application aussi et pour la 3ème année, le budget consacré à la justice et en hausse dans le projet de loi de finances pour 2023 en 5 ans, il a augmenté de plus de 40 % avec près de 700 magistrats, 850 greffiers et plus de 2000 juristes, recrutés, ce qui est historique, cette nouvelle augmentation de 8 pour permettra la création de 2253 emplois un équivalent temps plein dans son rapport, le comité relève à juste titre, que l'ensemble des constats sur la justice sont aggravées, un autre et que la défiance envers l'institution, il est plus accrue, c'est le cas du déficit et de la mauvaise gestion des moyens humains à Mayotte et en Guyane par exemple, les acteurs de la justice se plaignent d'une désorganisation permanente des juridictions liée à un fort absentéisme des magistrats et des greffiers, épuisés par leurs charges et conditions de travail, la dépendance financière des juridictions de Guyane ou de Mayotte empêche de répondre directement et efficacement aux besoins de ces territoires, c'est le cas également du manque de réponse pénale en dehors de la prison elle- même en crise sévère, c'est enfin le cas de la fracture numérique démultiplier un autre maire, monsieur le garde des Sceaux je vous sais concerné par les problèmes que rencontrent à l'outre-mer, nos citoyens dans l'accès à la justice et les acteurs du monde judiciaire dans leur travail, vous présenterez prochainement un plan d'action et une loi de programmation pour la justice, comment un putain des vous ventiler les crédits et moyens dans ces territoires reculés afin d'y relever les défis constaté. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, ce sénateur Dani, comment vous dire je, je suis très préoccupé, évidemment, par la situation guyanaise et et je rentre de Guyane, je m'y suis rendu avec Gérald Darmanin Gabriel Attal, nous avons renforcé considérablement les moyens douaniers, forces de sécurité et magistrats et greffiers le problème principal est un problème d'attractivité et nous avons créé à la chancellerie, une brigade de soutien. Qui consiste à demander à des magistrats métropolitains de partir six mois et un jour le un jour pour des raisons fiscales que que vous avez évidemment et pour aider les magistrats sur place, nous allons dupliquer cela nous le mettons en place, en Guyane, nous le mettrons en place à Mayotte, bien évidemment et nous enverrons des personnels supplémentaires, j'ai par ailleurs lorsque je me suis déplacé à Mayotte, indiquait que pour un magistrat pour un greffier, se rendre à Mayotte, ça devait être un tremplin et nous faisons en sorte que, au sortir de Mayotte, les greffiers, les magistrats sache exactement où ils seront nommés ou plus exactement renommé, alors il y a évidemment des opérations immobilières importantes qui sont prévues, cité du ministère de la justice à Saint-Laurent du Maroni cité judiciaire à Cayenne cité judiciaire et centres éducatifs fermés à Mayotte et bientôt un 2ème établissement pénitentiaire les outre-mer ont besoin évidemment de davantage de moyens, nous le savons, je souligne ici l'engagement total qui est le vôtre, à la fois pour votre territoire mais également pour la justice, vous êtes toujours Monsieur le sénateur au rendez-vous et vous nous rappelez ce que nous devons faire et ce que vous dites nous oblige. Merci, la parole est à Madame Laurence arrivé pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci madame la présidente, monsieur le le ministre, le rapport des états généraux préconise l'augmentation des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation mais pas seulement, il préconise aussi la généralisation de la présence de psychologues dans tous les services, c'est une nécessité que nous avons largement mesuré lors de notre mission d'évaluation sur les SPIP avec ma collègue Marie Mercier qu'on tait constater que le le faible nombre des assistants sociaux, un par département seulement pourtant fondamentaux puisque les ces pipes évolue vers un métier qui est plus de mesurer le risque de récidive, plutôt que la seule réinsertion donc la question est simple : quelle suite allez-vous donner à ce volet sur l'Inde, l'interdisciplinarité Alain à l'intérieur des SPIP, d'autre part, nous avons aussi remarqué un problème d'attractivité et un manque d'accompagnement face à l'évolution même des métiers nécessité d'un écosystème des acteurs en la matière, quelles suites voulez-vous donner au rapport. Si monsieur le garde des Sceaux, vous avez la parole. Merci madame la sénatrice, vous posez là une question très importante que celle de l'interdisciplinarité, je voudrais vous dire que c'est la boussole qui est la nôtre pour les recrutements qui sont à venir, j'ai déjà répondu tout à l'heure monsieur le sénateur ben arrange sur l'intérêt, évidemment, que nous Portions c'est pipe qui sont absolument indispensables, je rappelle pour mémoire, 1500 ces pipes engagé depuis 2018 j'ai rappelé tout à l'heure, les revalorisations, ce qui témoigne évidemment de l'intérêt que nous portons à cette profession que nous considérons comme absolument essentielles dans la politique de réinsertion et de lutte contre la récidive des personnes placées sous main de justice. La priorité, c'est évidemment de valoriser le travail des ces pipes d'en embaucher davantage, j'ai souhaité que la dotation allouée en 2023 soit porté à 122,5 millions, soit plus 12 9 millions d'euros, qui représente, ce qui représente une hausse de 13 % par rapport à 2022 politique active de préparation à la sortie à la réinsertion, en lien étroit avec les services de l'État, les collectivités territoriales, bien sûr, et les partenaires privés mais également les dispositifs de formation professionnelle des personnes détenues et le développement du travail en détention, auquel je suis, vous le savez, particulièrement attaché l'interdisciplinarité, pour revenir à la question, c'est une réponse bien sûr que nous envisageons, il n'est pas possible d'ailleurs de faire autrement, il est logique que cette interdisciplinarité trouve écho dans les recrutements à venir. je vous interroger plus que sur les c'est pipe sur les assistants sociaux puisque vous aviez déjà répondu en partie sur les c'est en fait, on est bien à la croisée des chemins, dans ce domaine-là, avec de nouveaux métiers et une approche beaucoup plus d'transdisciplinaire, nous sommes passés en gros d'une culture d'assistance sociale et d'accompagnement à l'insertion, à une culture plutôt du de la mesure du risque de récidive pour laisser d'où la nécessité d'autre métier à côté et d'une, et pour plaider une autre ingénierie de la sanction et ceci nous ramène aussi à des éléments que nous avons vu dans la mission d'information relative à la à la lutte de la délinquance des mineurs et qui est du même type, il est clair que l'augmentation du nombre de de places dans les prisons n'est pas la solution et c'est ce que dit très clairement le rapport Sauvé. Merci. La parole est à Madame Cécile Cukierman pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Merci madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le rapport du groupe de travail sur la simplification de la procédure pénale prévoit l'intronisation de l'Intelligence artificielle comme outil d'aide à la décision pénale certes le droit pénal, la procédure pénale sont devenus très complexe, certes, je ne fais pas partie de ceux qui rejettent la science et la technologie quand elles apportent à l'émancipation humaine pour autant, le recours à l'Intelligence artificielle lors du jugement n'est-ce pas avoir recours à un juge robot déshumanisé à une justice qui entrent dans une logique d'automaticité, perdant ainsi tout son sens, son sens 1er à savoir rendre justice au nom de tous en prenant en compte la situation de chacun. Vous n'avez pas prononcé ces mots, madame la sénatrice mais je pense que nous préférons une justice humaine. Merveilleusement humaine parfois terriblement humaine à n'importe quel robot s'il suffisait d'introduire je ne s'écarte quelle carte informatisée dans une machine pour avoir les solutions, je crois que d'abord nous n'aurions plus de raison d'être, il y aurait plus de difficultés plus de problématique, moi je suis très attaché comme vous à l'indépendance de la justice, l'indépendance a pour corollaire que parfois certaines décisions qui sont vendus peuvent nous faire un peu tiqué oui mais dans les états totalitaires, la justice est à la botte, alors moi je préfère une justice indépendante et d'ailleurs on on ne parle que des choses qui vont mal, jamais de celles qui vont bien, ils sont quand même extrêmement majoritaire, donc oui, je préfère une justice humaine qui peuvent se tromper à une justice informatisé, voilà ma réponse et et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, la personnalisation de la peine, par exemple, je sais pas trop comment l'Intelligence artificielle pourrait se débrouiller avec ça, oui, je me pose franchement la question et j'ai pas trouvé la réponse. Merci madame Cukierman, vous avez une minute 12. Oui merci madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, puisque vous m'y invitez, je pourrais vous dire dans un meeting politique bien évidemment l'humain d'abord, mais je ne l'ai pas fait pensant que cela était tellement évident venant des propos de notre groupe que j'ai évité cette répétition inutile ici dans l'hémicycle Plus sincèrement et, plus sérieusement, effectivement, nous nous pensons et nous l'avons toujours défendue, que la justice ne peut se passer de l'humain de cette émotion et qui, comme toute émotion parfois être aussi con contestable mais qui en tout cas, permet de rendre une justice la plus juste possible je reprendrai d'ici et sans aucun parallèle avec avec quelques actualité, que ce soit les propos du président buffet dans son intervention liminaire liminaire, la justice est effectivement un lieu qui apaise pour pouvoir apaiser ah la, besoin de ces moyens humains qui écoutent, qui entendent qui parfois répare qui parfois réinsère qui parfois juge qui parfois contrôle les lieux, y compris de privation de privation de liberté, de de la liberté, mais en tout cas cette justice qui apaise est indispensable à notre société, à la différence d'un jugement sur la place publique qui au contraire hystérise cristallise et oppose les gens entre eux. Si la parole est à Madame Dominique, j'ai rien pour le groupe Union centriste. Merci madame la présidente. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc en cette rentrée parlementaire, je crois qu'il est important de toute de suite reprendre nos bonnes habitudes et ainsi, Monsieur le Ministre, vous avez raison, sans surprise, je vais vous parler d'informatique, en effet je vous alertent depuis longtemps sur cet aspect, en particulier sur les logiciels Cassiopée en tête, c'est une question plus central, qu'il n'y paraît, tant le personnel de justice peut se retrouver découragés face à des applicatifs obsolescence qui accumule les lourdeurs les incompatibilités et les bug votre ministère parle même de goût amer laissé aux agents, comme le note le rapport des états généraux de la justice ainsi le comité en appel, ni plus ni moins à une refondation complète de la maîtrise d'ouvrage informatique ainsi qu'à la fondation d'un véritable socle informatique commun à la fois au sein de la justice, mais aussi avec les ministères partenaires l'intérieur par exemple et pour mémoire, procédure pénale numérique qui se met en place, souffrent elles aussi des bogues de Cassiopée, en particulier dans le cadre des transferts entre gendarmerie et justice, comme j'ai pu constater moi-même dans une gendarmerie a Toussi ma question est donc simple, Monsieur le Ministre quel plan d'action entendez-vous mettre en oeuvre, à ce titre, hein, le ministère de l'intérieur par la loi Lopmi entend créer une agence numérique une seule agence pour les 2 ministères serait-elle envisageable. Merci monsieur le garde des Madame la sénatrice Verts rien on travaille en concertation avec Bercy pour répondre à la préoccupation légitime qui est la vôtre, j'ai nommé il y a peu de temps un secrétaire général adjoint du ministère qui est dédié au numérique, nous avons été, vous le savez, ça n'a échappé à personne, critiqué par la Cour des comptes, mais la Cour des comptes a cependant indiqué que nous avions fait beaucoup d'efforts et je compte évidemment les poursuivre. Le rapprochement des maîtrises d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre, projet par projet est une priorité clairement identifiés et ça permettra au projet de gagner en cohérence et en efficacité, mais je vais vous dire 2 choses : d'une part, je ne crois pas qu'il y ait en la matière un modèle unique qui serait le plus efficace pour tous les ministères, et d'autre part j'entends vraiment que le ministère au au-delà de sa spécificité ne soit plus perçu comme le ministère des vieilles pierres, mais comme un ministère moderne, efficace, exemplaire dans sa gouvernance son exécution budgétaire ces indicateurs que nous venons d'imposer, je serai donc très attentifs à ce que, par exemple, la gouvernance numérique, souhaite organiser de la meilleure manière possible et je ne doute pas que je serais interrogé dans un avenir proche, sur ce que nous avons fait pour mettre en ordre dans notre ministère, le numérique, je suis d'accord avec vous, enfin le sujet de la transformation est majeur pour l'avenir de ce ministère, bien sûr, et nous aurons, je suis sûr de cela, l'occasion d'en débattre, ne fût-ce qu'à l'occasion du débat sur le budget, voilà madame la rapporteure, j'espère vous avoir rassuré un peu. Merci madame veut rien vous avez 30 secondes. Merci beaucoup, madame la présidente, alors vous parliez de Bercy, effectivement, vous avez une interface pour le paiement des amendes qui semble être fait par Bercy qui fonctionne bien, parce que pour le coup, ils ont très bien su se mettre en ordre de marche au niveau informatique pour prendre nos sous, ce serait bien qu'on puisse nous aussi avancé pour pouvoir rendre la justice et par ailleurs on ne peut pas ne pas travailler avec le ministère de l'Intérieur, parce que la procédure pénale numérique concerne l'ensemble des 2 ministères et il faut que les gens puissent se parler. Merci Madame Esther Benbassa. Madame la la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, les conclusions des états généraux de la justice confirme l'état déplorable de notre institution judiciaire, une des premières décisions du garde des Sceaux, fut d'augmenter les magistrats judiciaires de 1000 euros je salue cette initiative mais les magistrats et greffiers souffle surtout du manque de moyens humains et matériels dans quelques semaines, nous nous a été durant le projet de loi des finances pour l'année 2023 il nous appartiendra d'être particulièrement exigeant sur la répartition des crédits, le texte Samir annoncé prévoit une nouvelle hausse de 8 % cela représente 710 millions supplémentaires sur l'année dernière, dont 41 % reviendrait à l'administration pénitentiaire, je me réjouis qu'un tel budget soient alloués aux établissements pénitentiaires, toutefois j'émets quelques réserves sur ces dépenses qui concernerait en partie le parc immobilier pénitentiaire, monsieur le Ministre, je comprends votre volonté de mettre fin à la surpopulation carcérale, mais la construction des prisons, comme vous le savez, n'est pas la seule solution, plus on construit, plus on remplit la réponse à ce problème structurel se trouve du côté de la prévention de la récidive de la réinsertion et des peines de substitution sous certaines conditions, je pose donc la question : la loi des finances pour 2022 accordées aux alternatives à l'incarcération, un budget stagnant de à 39 8 millions d'euros compte près d'un milliard d'euros d'investissement immobilier pénitentiaire pour 2023 comment comptez-vous répartir l'enveloppe budgétaire entre insertion et alternatives à la prison, je vous remercie. Si, mais si monsieur le garde des Sceaux. Madame la présidente, madame la sénatrice puisque vous m'y invitez, je vais vous répondre sur le registre budgétaire alors vous l'avez indiqué la programmation immobilière de 15000 places absolument essentiel pour mettre fin à la surpopulation pénale, ça n'est pas évidemment la seule solution je pense évidemment aux conditions indignes, bien sûr j'y attache comme vous d'ailleurs une attention toute particulière, l'émission réalisée par le SPIP, notamment en milieu ouvert, tout aussi essentiel et doivent continuer à se développer le ministère poursuit une politique volontariste en faveur des mesures alternatives à l'incarcération des aménagements de peine, et en 2023 pour répondre précisément. à votre question, la dotation correspondant s'élèvera à 53,4 millions d'euros, soit une progression de plus 34 % par rapport à 2022 28 millions seront consacrés au placement sous surveillance électronique, le placement extérieur bénéficiera d'une dotation de 11,3 millions d'euros, soit un complément de de 5 millions d'euros destinés au relèvement du prix de la journée pour favoriser l'octroi de ces mesures 6 millions sont prévus pour accompagner le déploiement du contrôle judiciaire sous placement probatoire enfin la dotation allouée à la politique de réinsertion des personnes placées sous main de justice sera elle aussi portée en 2023 122,5 millions c'est une hausse de 13 % par rapport à 2022, vous savez d'ailleurs madame la sénatrice tout l'attachement que je porte au sens du travail l'effort des publics qui exécute une peine qu'elle soient accomplis en milieu ouvert ou en détention et je vais naturellement favoriser le travail et la venue massive de ce qui peuvent t'offrir ce travail, ce qui permet bien sûr une meilleure réinsertion. Merci amène bah ça vous n'avez que 8 secondes pour remercier monsieur le garde des Sceaux, merci. Si Monsieur le Ministre, mais je voudrais vous demander qui liait prochainement un état des lieux des lieux privation de liberté et qu'on aborde spécifiquement ce sujet même si là, il est dans les échanges commerciaux de la justice maire. Merci, la parole est à Madame Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, merci, madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 13 septembre 2021 Je déposé une proposition de loi pour développer le recours à la médiation, le groupement européen des magistrats pour la médiation et plusieurs autres acteurs du monde judiciaire relevé le caractère essentiel de cette proposition, si du chemin reste à faire pour promouvoir le recours à la médiation dans notre pays, je tiens à vous remercier monsieur le Ministre pour l'engagement personnel qui est le vôtre dans le développement de ce dispositif, notamment en réaction au dépôt du rapport des états généraux de la justice, de nos jours le recours à la médiation est encore trop peu développée en France, même si des expériences ponctuelles comme au référé du tribunal judiciaire de Paris donne d'excellents résultats, d'autant que l'usage de ce dispositif est fortement encouragée par nos concitoyens, en effet, dans un sondage du CSA réalisée pour le Sénat en 2021 90 % des Français interrogés plébiscité le recours à la médiation et à la conciliation, la médiation est un outil précieux pour notre système juridique permettant aux justiciables de se réapproprier le procès en en devenant des acteurs-responsables, il permet de résoudre des situations qui semblait bloqué en renouant le dialogue avec l'aide d'un tiers compétent neutre et impartial en 2021, la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a marqué une étape en facilitant le recours à la médiation et en actant la création du Conseil national pour la médiation mais il est nécessaire d'aller plus loin et d'engager une véritable politique nationale de l'amiable judiciaire dans notre pays, monsieur le garde des sceaux, pouvez-vous m'assurer que vous développerait le recours à la médiation en faisant évoluer la loi ma PPL est à votre disposition en attendant envisageriez-vous de prendre rapidement des mesures concrètes en valorisant la médiation dans l'organisation des juridictions en développant la formation des acteurs judiciaires et en adoptant des mesures incitatives, je vous remercie.

une décision à laquelle on a participé, est une décision qu'on accepte mieux, par ailleurs, ça nous économise si j'ose dire, du temps judiciaire que l'on peut consacrer par exemple au déstockage, vous verrez que dans ces états généraux de la justice, la médiation ressort de façon très consensuel, et même une procédure dont je j'aurais évidemment l'honneur et le plaisir de vous reparler, qui est une procédure de césure, nous nous sommes inspirés de l'étranger, on a uniformisé, vous, vous l'avez rappelé la liste des médiateurs actualiser les formulaires de candidature on a triplé la rétribution aide juridictionnelle pour les avocats qui participent à la médiation, tout ça, vous l'avez rappelé, je sais que vous portez un texte et je serais vraiment ravi, je le dis que vous veniez à la chancellerie, qu'on puisse ensemble évoquer l'ensemble de ces questions, le civil est extrêmement important, Monsieur le président, il fait la rappeler, et nous n'avons pas encore arbitré, madame la sénatrice nous discutons encore, j'ai souhaité vraiment que tout le monde soit associé à ces états généraux venait à la chancellerie, c'est une invitation naturellement et pas un impératif et nous évoquerons ces questions parce qu'il faut faire progresser la médiation, je pense que c'est la justice de demain, à l'évidence, voilà je je je je vous attends. Merci, la parole est à Madame Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains Si madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, donc la confiance dans dans nos institutions et le coeur de notre pacte républicain et aux côtés du pouvoir législatif et exécutif la justice participe grandement à cet enjeu fondamental, je me félicite du travail qui a été menée par les états généraux de la justice de manière systémique globale et associant l'ensemble des acteurs pour mettre en place des pistes de réflexion, d'ampleur mais on voit aujourd'hui que le travail est abyssal, et que il va nécessiter effectivement beaucoup d'investissement mais aussi une priorisation donc j'entends que vous avez une méthode et que vous allez pouvoir définir de manière concertée, ces axes de priorisation, mais comme l'a justement rappelé le président de la commission des lois la priorisation et pour redonner confiance, il faut d'abord la proximité, la justice du quotidien, celle qui correspond aux besoins de chaque jour, c'est avant tout la justice civile et au sein de cette justice civile il y a un sujet qui nous tient à coeur, alors que le collègue, la vice-présidente Delattre, la vice-présidente Gruny et Corinne Corinne frère et nous avons remis un rapport sur la justice prud'homale qu'il y a déjà 3 ans faisait de nombreuses propositions pour justement restaurer cette confiance sur cette justice du travail cette justice du quotidien alors que, aujourd'hui, bien que le nombre d'affaires et largement diminué, moins 55 % les délais de jugement reste très long autour de 16 mois, on le voit bien qu'il qu'il y a un besoin de réforme systémique, donc cette réforme de la justice prud'homale, monsieur le garde des Sceaux est-elle dans vos priorités. Si monsieur le garde des Sceaux. C'est dément vouloir madame la sénatrice et dire que je me répète mais la réponse est oui, bien sûr, alors je je je connais évidemment votre rapport, c'est une question de temporalité puisque évidemment on ne peut moi il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, je vais pas les rappeler ici, je pense pas que nous ayons chômé que nous ayons perdu notre temps, mais voilà venu le moment effectivement de réfléchir à nouveau sur la justice prud'homale, parce que ce que nous souhaitons, c'est une justice plus proche, c'est une justice plus rapide, c'est une justice plus efficace, et donc les propositions qui ont été faites seront intégrés, évidemment dans ces états généraux et de la même façon que je l'ai fait tout à l'heure, je vous invite évidemment à venir partager avec moi un certain nombre de solutions que vous souhaitez voir reprises les arbitrages, une fois encore, ne sont pas terminées, je suis tout à fait ouvert à ça j'ai j'ai si, si, si, il me reste, oui, il me reste un peu de temps, je voudrais vous dire un peu quelle est la méthode que nous avons mis en place, moi je ne suis pas intervenu ni dans le comité des états généraux qui a été mis en place, ni dans les différents ateliers de travail : je ne voulais pas que l'on dise que c'était ce que souhaitait le ministre au fond et puis quand tu le rapport Sauvé a été rendu, ainsi que les annexes, j'ai réuni tout le monde et ce que je souhaite garder, c'est ce qui est consensuel. Voilà ce qui m'importe, je suis un peu une autre méthodologie à une autre gouvernance, ça n'est pas caporaliste vient pas du haut pour irriguer vers le bas, c'est une discussion avec tout le monde, les conférences, les syndicats qui ont valu vous vous venir à tous venus, mais peu importe, c'est leur problème, une porte que l'on ne franchit pas n'est pas une porte fermée, donc voilà un peu la méthode et donc il se dégage des choses très consensuel, je l'ai dit à plusieurs reprises, pardon de me répéter, mais c'est comme ça qu'on va progresser sur ces états généraux, parce que c'est l'affaire de tous et je pense que tout le monde a compris que c'était un moment historique et important pour notre justice, donc bienvenue madame la sénatrice. Merci alors même Canayer, vous avez 21 secondes. Merci monsieur le garde des Sceaux, bien évidemment, nous participerons pour pouvoir étoffer la réflexion j'entends cette demande de consensus, néanmoins, il est important aussi que certaines réformes s'imposent à un moment donné, et que si le consensus peut être nécessaire, je pense que ceux des réformes, elles doivent être aussi d'ampleur et systématique la justice prud'homale pour revenir sur le sujet est quand même au milieu du gué et celle demande d'aller vraiment beaucoup de plus loin. Merci, la parole est à monsieur Dany Wattebled pour le groupe, les indépendants. Merci madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, dans notre pays, la justice, en crise depuis trop longtemps, alors que le gouvernement s'apprête à consentir pas 3ème amené consécutive un effort budgétaire sans précédent. Les difficultés d'institutions n'ont toujours pas été surmontée à l'occasion des états généraux de la justice, plusieurs dizaines de milliers de contribution de nos concitoyens tant professionnel de droit que 5 justiciables ont été recueillis. Elles ont souligné la place fondamentale du récit de la justice au sein de notre société démocratique et notre état de droit, il est crucial qu'elles fonctionnent correctement et efficacement non seulement, non seulement pour les partis, mais également pour l'ensemble de notre société. Le rapport du comité d'usagères ou la justice rappelle qu'entre 2009 et 2020, le code pénal a été modifié par 11 loi chaque année en moyenne et le code de procédure pénale par 17 lois. Cette évolution complexifie à n'en pas douter, le quotidien des policiers, des gendarmes et procédure. Au-delà de l'inflation normative, le rapport estime que la refonte de la procédure pénale est nécessaire, il se prononce en faveur du maintien du juge d'instruction, mais surtout envisage d'unifier les cadres, l'enquête de flagrance l'enquête préliminaire. Il propose pour ce faire, de conduire une étude d'impact sur les différents scénarios de livres une unification des régimes d'enquête. Monsieur le garde des Sceaux, comptez-vous mener cette étude d'impact et que pensez-vous de l'autre moitié de la le 7 telle d'une telle fusion. Si monsieur le garde des Sceaux.

multiplication de textes qui sont venus complexifier la procédure pénale, au point que les professionnels disent eux-mêmes que on a aujourd'hui beaucoup de mal à s'y retrouver, donc on envisage une simplification. Les policiers, les gendarmes, les magistrats, les greffiers, les, les, les avocats, la demande il y a une unification des délais, par exemple, il y a la question de l'enquête préliminaire et de l'enquête de flagrance. On ne peut pas cependant supprimé la notion de flagrance qui figure je le rappelle, à l'article 26 de la Constitution et qui permet d'ailleurs d'arrêter sans autorisation du bureau de l'Assemblée ou du Sénat, un parlementaire en quatre Crime flagrant, ce petit clin d'oeil, mise à part, oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être simplifié en étant évidemment respectueux des droits de la défense des libertés individuelles, des libertés publiques et c'est vers cela que nous irons ce travail, on estime qu'il va durer 2 ans et je dis parce que c'est une réalité que bien sûr les parlementaires seront associés de près à l'élaboration de ce travail et que les études d'impact seront conduites bien sûr parce que on ne peut pas en la matière, avancer à l'aveugle non soyez parfaitement rassuré, nous avons commencé bien sûr à travailler sur ces sujets, ils sont colossaux, c'est extrêmement ambitieux, mais le Parlement sera associé à ce travail qui êtes aujourd'hui un travail demandé et un travail absolument indispensable. Merci monsieur. Vous avez 25 secondes. On va gagner un peu de temps, merci votre réponse, monsieur le garde des Sceaux. Merci. Si la parole est à monsieur Jean Yves Le compte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous nous vous savons monsieur le garde des shows attaché au renforcement de l'indépendance du parquet et nous partageons nombre ici sur ces bancs, le souhait de voir enfin aboutir une réforme du Conseil supérieur de la magistrature permettant d'y parvenir. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme refuse d'assimiler le ministère public français à une véritable autorité judiciaire au sens au sens de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté, le Sénat avait adopté en juillet 2013, un projet de loi constitutionnelle qui avait pour objectif de renforcer l'autorité du CSM et de mieux garantir l'indépendance et l'impartialité des magistrats, malheureusement, il aurait fallu attendre avril 2016 pour que ce texte soit voté en termes identiques par l'Assemblée nationale et puis plus rien, près de 2 ans plus tard, lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, en janvier 2018, le président de la République avait lui aussi affirmé ce soit de renforcer l'indépendance du ministère public et indiqué que la réforme se préparerait que préparer votre à leurs voeux prédécesseurs Madame Nicole Belloubet devait intégrer ces éléments, il y a une quinzaine de jours au sujet du statut du parquet lors de son audition par la commission des lois du Sénat à l'occasion du rapport remis sur les états généraux de la justice monsieur Jean-Marc Sauvé a d'ailleurs indiqué qu'il avait eu à soumettre au président de la République, un décret de convocation du Congrès sur cette réforme, puis je cite, de démontage du Congrès, ajoutant que c'était la seule fois dans l'histoire de la République, un tel acte avait été pris. Aujourd'hui, je souhaitais monsieur le garde des Sceaux, savoir si vous pouviez nous éclairer sur le calendrier relatif à cette nécessaire réforme pour qu'enfin puisse être effectif le renforcement de l'indépendance du parquet. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, le compte, je n'ai pas de réponse calendaire à vous fournir, on va redire les choses, vous les avez d'ailleurs pour partir appeler réforme du statut du parquet, il ne peut se faire que par une modification de l'article 65 de la Constitution bien le rapport Sauvé l'évoque dans des termes que vous avez rappelé Dijon pour être tout à fait précis que cette proposition ne fait pas consensus qu'être aujourd'hui discuter et moi je vous propose de mettre ce sujet à l'ordre du jour de la commission transpartisane voilà sur les précisions calendaire, vous comprendrez bien sûr que je suis incapable de vous en dire davantage. Merci monsieur le comte ah vous avez 23 secondes. secondes. Présidente nous avons absolument besoin d'avancer sur un sujet essentiel pour notre État de droit, surtout si l'on parle aujourd'hui de des des états généraux de la justice, le développement des missions des procureurs de la République exige cette réforme

merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, le rapport sur les états généraux de la justice, insiste sur le fait que la justice connaît une crise dite systémique ce mot a d'ailleurs été employé dans la bouche de mais d'une de mes collègues tout à l'heure, lorsque l'on regarde les réponses qui vous sont fournis ou qui sont fournis au président de la République, dans le cas du rapport forcé de constater que les mesures elles-mêmes sont sectoriels, on voit immédiatement que face à une crise systémique, la question est de savoir par quel bout prendre ce sujet en vous écoutant tout à l'heure monsieur le président, Monsieur le Ministre, j'ai entendu la référence à un plan d'action détaillé a des voulez réglementaires à une loi de programmation 2022 2027 ah, une feuille de route sur la réforme de la procédure pénale, a une nouvelle politique pénitentiaire à une politique ambitieuse de l'amiable, on voit bien que les priorités sont multiples et vous savez, monsieur le garde des Sceaux que quand tout est prioritaire, il n'y a plus de priorité et donc j'ai finalement de questions à vous poser : la première, quelle serait votre priorité et la 2ème, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une autre approche de ce sujet qui consisterait à tirer les conséquences et les avantages de l'effort budgétaire massif que vous avez obtenus, vous en feront, il faut vous en faire crédit de laisser les recrutements sortir leurs effets dans le monde de la justice, les nouveaux moyens financiers finalement stabiliser la structure et passer ensuite dans un 2ème temps à une série de réformes plus sectorielles, même si on sent bien que vous bouillait d'impatience sur ces sujets, donc finalement quelle temporalité dans la gestion de ce sujet, mais

Rien n'est possible ensuite renforcement bien sûr grâce à ce budget, des moyens humains, très attendu par tout le monde. Tout à l'heure, l'un d'entre vous, a rappelé ce que nous avions fait en terme d'embauche, j'ai pas le rappeler ici, nous avons dit 10000 personnels supplémentaires 1500 magistrats, 1500 greffiers des contractuels, ensuite le civil et le civil de façon réglementaire, on ne pourra pas me reprocher, comment dirais-je, une loi, une loi nouvelle une, une inflation législative mais naturellement, vous serez associés au au réglementaire et et de près ce réglementaire civil, il a pour objet, on l'a évoqué, d'aller vers davantage de de médiation de de simplifier cela ensuite, bien sûr, il y aura du législatif, une loi de programmation : bien sûr, la réforme de la procédure pénale est très vraisemblablement une loi organique, puisque les états généraux de la justice évoque un certain nombre de modifications et qui nous conduisent à passer par la loi organique, tout ça va se conduire, si j'ose dire, en même temps, en tous les cas, rapidement, moi je veux aller vite le réglementaire, très bien, loi de programmation pour janvier 2023 début d'année pour que l'on ait un étalement jusque la fin du quinquennat et puis le reste naturellement suivra son cours, j'allais dire ordinaire mais le consensus me permettra, je le crois. D'obtenir l'adhésion des parlementaires parce que je me dis, et c'est d'ailleurs ce qui a guidé ma réflexion, si tout le monde est d'accord, forces de sécurité intérieure, magistrats, greffiers, avocats mais je pense que les parlementaires constateront cet accord et qu'ils n'ont qu'une envie, aussi, c'est d'améliorer la justice du quotidien voilà monsieur le sénateur, ce que je peux vous répondre à ce stade. Merci. La parole est à monsieur Antoine Lefèvre pour le groupe Les Républicains. Merci madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les états généraux de la justice ont été convoqué à point nommé alors que l'institution judiciaire semblait condamnée à s'enfoncer toujours plus dans la détresse, soulignée par les conclusions du rapport, il est impératif aujourd'hui de ne pas se laisser de ne pas laisser s'éteindre la dynamique qui est né de cette large concertation, cela a été dit maintes et maintes fois je le redirai une fois de plus ici la toute première urgence de nos tribunaux et celle du renforcement des moyens humains proportionnellement au volume du contentieux en attente de jugement, c'est pourquoi, s'il est important de saluer la revalorisation salariale des magistrats que vous avez appelé de vos voeux, le 12 septembre dernier, celle-ci ne doit pas faire oublier la véritable priorité financière de l'institution judiciaire qui est celle de sortir ces tribunaux de la déshérence et ses outils informatiques de l'archaïsme je solliciterai Monsieur le Ministre, vos précisions sur le point suivant : les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation vous ont récemment fait part de leur souhait de voir engager une réforme de revalorisation de leur statut et de leurs indemnités cette revendication intervient après qu'une amélioration apportée en 2017 au statut des conseillers d'insertion et de probation à effacer les différences de traitement et de statut entre les 2 corps pourtant hiérarchiquement distincts, la responsabilité exercée par les directeurs sur les conseillers d'insertion souffre ainsi d'une perte de légitimité préjudiciable aux brumes l'exercice de leur mission, à cela s'ajoute l'importante perte d'attractivité du métier, qui a déjà conduit, cet été, à ce que seuls 6 postes sur les 22 proposés aux concours internes soient pourvus les demandes de détachement à l'extérieur, quant à elles, ont triplé en 4 ans, ma question, monsieur le ministre est donc la suivante : quelle place souhaitez-vous accorder aux revendications des directeurs d'insertion et de probation dans les chantiers que vous souhaiterez entreprendre à la lumière des conclusions de ces états généraux, je vous remercie. Merci monsieur le garde des Sceaux. Ici. Madame la présidente, monsieur le sénateur Lefèvre vous m'interrogez sur ce que le ministère compte faire pour rendre le métier de des pipes plus attractif, bon il est vrai que les réformes interministériel qui ont été engagés depuis 2017 ont abouti à revaloriser les salaires des conseiller pénitentiaire mais pas des directeurs il en est de même d'ailleurs pour les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse alors concernant les les des pics les des pipes c'est le sujet de votre question, le ministère s'engage en 2022 c'est en cours à revaloriser les primes des des PIB d'environ 700000 euros, qui viennent s'ajouter aux 600000 euros, qui ont été octroyés à ce corps, en 2021 et en 2023 je porterai la poursuite de la hausse des primes à hauteur d'un 1000000 d'euros, une réforme du statut pour faciliter la promotion professionnelle et les parcours de carrière plus attractif et une revalorisation de leur rémunération indiciaire à hauteur d'1 virgule 3 millions d'euros, ces évolutions sont évidemment légitime, nous avons reçu il y a quelques jours de cela, les représentants des dés je pense que, ils savent bien sûr ce que nous comptons faire et ce que nous comptons faire, vous l'avez vous-même souligné, c'est mettre, en avant bien sûr le le service qu'ils rendent à la justice et notamment avec les revalorisations adéquate. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre, vous avez 17 secondes. Bien moi je voulais remercier monsieur le Ministre, pour ces précisions et rappelé qu'un service public judiciaire clair organisé performant et la garantie de la cela dit de la solidité de notre État de droit. Merci, la parole est à monsieur Hussein Bourgi pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, monsieur le Ministre. Mes chers collègues, lors des audiences solennelle des tribunaux judiciaires comme lors des conseils de juridiction des cours d'appel de sujets reviennent de manière récurrente, le 1er concerne les moyens humains et de nombreux chefs de cour regrette que les postes de magistrats qui leur a été allouée depuis la dernière loi de finances ne soit toujours pas arrivé. Cette situation est d'autant plus difficile à comprendre que dans d'autres juridictions, des postes de juges sont en surnombre, comment et dans quel délai la chancellerie entend-elle remédier à cette réalité. Second point qui est soulevée lors de ces réunions, c'est celui qui concerne les dysfonctionnements du logiciel Cassiopée, cela a été évoqué tout à l'heure par une de nos collègue déployé depuis une dizaine d'années, à l'époque du ministre Michel Mercier, nous en sommes à une cinquantaine de version. Et il ne donne toujours pas satisfaction, Monsieur le Ministre, ce constat d'autant plus regrettable que nous ne disposons pas de référentiel d'activité pour évaluer les besoins de chaque juridiction avec des indicateurs et des éléments objectifs, dès lors, l'attribution des moyens par la chancellerie ne se fait pas dans des conditions tout à fait équitable, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, où en sont les travaux de la chancellerie pour nous doter d'outils informatiques efficient et d'un référentiel d'activité opérationnelle, je vous remercie. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, Bourgi le référentiel, nous devrions en disposer en décembre. Il faut longtemps pour créer un tel référentiel. J'ai demandé, moi il y a longtemps, trop longtemps sans doute que ce référentiel soit mises en place, il permet, effectivement, c'est un très bel outil pour le DJ décembre on nous l'aurons, il sera à disposition bien sûr et et vous serez informés de cela, alors je vais, je vais essayer de vous répondre complètement Cassiopée, d'abord, monsieur le sénateur, il est exact que des difficultés techniques ont été soulevés à Paris à Versailles, quant à l'utilisation de Cassiopée, cour d'appel, elles sont en cours d'analyse de résolution et les solutions seront probablement apporté 1er semestre 2023 Cassiopée tribunal être généralisé sur tout le territoire, s'agissant des effectifs de magistrats au sein de la cour d'appel de Montpellier en juin dernier, j'ai décidé d'augmenter les effectifs de magistrats dans cette cour de manière substantielle, c'est pas moins de 4 postes qui ont été créés de juges du siège de magistrat au parquet et ces postes sont à sept heures encore vacants, on poursuit les efforts de recrutement de magistrats 2023 verra la plus grande promotion d'auditeurs de justice, de de l'histoire de l'École nationale de la magistrature, avec 380 auditeurs ainsi et, dès 2023, nous réduirons évidemment la vacance de poste voilà je le dis et c'est une réalité, la justice et plus de 20 ans d'abandon budgétaire humain peu politique, on ne peut pas tout régler en un claquement de doigts, on s'y attache et les différents Budgets qui ont été obtenus, plus de 40 en ce qui me concerne 26 % puisque vous savez qu'en matière budgétaire trois fois huit ça fait pas 24 mai 26 c'est un effort considérable qui montre l'intérêt que nous portons à la justice de ce pays. Merci Monsieur Bourgi, vous avez 44 secondes. Monsieur le Ministre, effectivement je je reconnais volontiers les efforts budgétaires que vous évoquez, nous nous sommes en tous féliciter à la commission des lois, et par contre, la difficulté vient du fait qu'elles ont du mal à à se traduire rapidement sur le terrain et dans les juridictions et dans la cour d'appel de Montpellier que vous avez cité tout à l'heure qui est celle du ressort où je suis élu je voulais vous dire qu'effectivement des magistrats qui n'arrive pas à des postes de directeurs de grève qui ne sont pas pourvus, comme c'est le cas actuellement au tribunal judiciaire de Béziers ne facilitent pas la réduction des délais et de l'efficacité de la justice et ce qui nous anime, vous et nous tous ici et sénatrices et sénateurs si vous pouviez nous aider à remédier à ces problèmes-là, nous vous en serions engrais je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, la parole est à madame Nadine Nobel Lourau pour le groupe Les Républicains merci madame la présidente. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le constat dressé par le comité des états généraux, cela a été dit est particulièrement sévère sur l'état de fonctionnement d'une institution qui ne remplit plus ou très mal les missions de service public que les Français sont sont en droit d'attendre la tonalité de ce rapport se rapproche beaucoup d'ailleurs de celui de 2017 de Philippe Bas 5 ans pour sauver la justice mais 5 ans plus tard, nous en sommes toujours au même point, rares étant les préconisations à avoir été mis en oeuvre au cours de la précédente législature, 2 constats du rapport bah, d'ailleurs, se retrouvent dans celui du comité en 1er lieu l'augmentation continue des ressources allouées à la justice, vous vous en êtes récemment félicitée, mais cette augmentation n'a toutefois pas permis d'améliorer significativement son fonctionnement et le service public rendu aux en second lieu, l'institution judiciaire est au risque de rater la révolution numérique, les innovations technologiques les plus récentes font émerger de nouveaux acteurs privés qui peuvent concurrencer l'institution judiciaire, appelant à une nécessaire régulation, il existe 2 voies de réforme comme cela a été dit, la première concerne les procédures en matière civile, pénale, commercial, social, nous en connaissons la nécessité tout comme vous, comme nous connaissons également les contraintes internes et conventionnelle, la seconde concerne le management de la justice, quelle organisation, Monsieur le Ministre du ministère envisagez-vous pour assurer la bonne exécution des Budgets votés la fluidité de la gestion des ressources humaines, la maîtrise des frais de justice, la mise à niveau, comme cela vient d'être dit, d'une informatique judiciaire dont à chaque visite que nous faisons dans les juridictions, nous sommes obligés de constater l'incroyable inefficace. Et si merci, cher collègue, merci monsieur le garde des Sceaux. Madame la sénatrice, je ne suis pas d'accord avec vous et ça ne vous étonnera pas, nous avons embauché 700 magistrats, 850 greffiers 2000 personnels contractuels quand j'ai embauché ces contractuels, certains disaient : ce sont des rustines, mais pourquoi n'embauchez-vous pas des magistrats, je répondais benoîtement qu'il faut 31 mois pour les former, ils ont été envoyés dans toutes les juridictions auprès des parquets mille ils ont permis une réduction des stocks de 28 % et vous trouvez que ça n'est rien, pardon, mais c'est la moyenne nationale il y a des juridictions où c'est bien plus encore 28 % de ah mais je tiens les chiffres à votre disposition 28 pour 100 en matière civile, donc c'est une justice naturellement qui des stocks et c'est donc une justice qui va plus vite, vous dites que cela n'est rien, c'est votre analyse et je ne partage pas votre votre sentiment maintenant maintenant s'agissant de l'absence non mais maintenant sur la la question de la sous, exécution budgétaire au niveau du ministère alors sur les 15 dernières années c'est en moyenne moins de 1 % des crédits votés en loi de finances initiale qui n'ont pas été consommée, soit environ 100 millions sur un budget de 9 6 milliards

8 % en 2021, alors je vous concède effectivement une hausse en 2020, 2 6 % on est plus en 2020, aujourd'hui on est en 2022 ça est imputable bien sûr à la crise sanitaire, je ne doute pas que vous le savez, avec un pays à l'arrêt pendant des moins et des mois, ce qui n'a pas permis au ministère de dépenser leur crédit normalement pas plus que cela a permis au ministère de faire pousser les prisons parce que je pense que, dans un instant, j'entends dresse là, j'ai déjà entendu, vous dites oui, monsieur le sénateur, bah je je je je ne lis pas dans vos pensées mais je vous anticipe c'est bien dire. Et. Et je vais dire, et je vous ai à peu près répondu madame la sénatrice pardon. Merci monsieur le garde des Sceaux, la parole est à Madame Catherine Rithy pour le groupe Les Républicains. Merci madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, les constats issus du rapport Sauvé associe une crise de l'autorité judiciaire et une crise du service public de la justice, je voudrais insister sur le lien étroit qui les unit en vous interrogeant sur une cause commune, qui ne devrait pourtant pas être un problème les variations démographiques en tant qu'élu de Moselle je suis bien sûr sensible aux disparités de peuplement dans les zones rurales, mais je le suis plus encore à leur évolution lorsque nous soutenons les politiques urbaines et la croissance démographique de certaines zones, or j'ai pu le vérifier dans ma région, mais aussi lors d'un stage d'immersion au tribunal de Bordeaux, l'accroissement de la population urbaine, particulièrement dans les métropoles s'accompagne naturellement d'une augmentation des affaires pénales et civiles, c'est le cas récemment des atteintes aux personnes, mais aussi des affaires familiales, face à cette dynamique démographique l'accroissement d'une déjudiciarisation de certains contentieux ou l'invention d'une énième réforme, réforme, pardon de la carte judiciaire n'auront qu'un effet limité adapter la justice nécessite davantage, outre une augmentation généralisée des moyens, une meilleure anticipation et une meilleure gestion dans l'emploi des ressources humaines et matérielles de la justice, il pourrait s'agir de gestion de carrière de mobilité géographique ou d'instruments de suivi des des masses contentieuse, entre autres exemples, quelle stratégie le Ministre de la Justice entend-il adopté afin de réussir cette anticipation des évolutions démographiques et améliorer la réponse de la justice dans ce contexte. Comme vous voulez monsieur le garde des Sceaux. Pardon, pas même madame la sénatrice les moyens humains, des juridictions, il s'agisse des magistrats ou des greffiers sont ajustés chaque année après examen des données d'activité des juridictions et l'outil dont je parlais tout à l'heure qui sera à notre disposition dès le mois de décembre nous permettra évidemment permettra la DJ d'affiner les besoins des différentes juridictions les évolutions démographiques honte évidemment un impact déterminant sur l'activité des juridictions puisqu'une augmentation de la population d'un ressort entraîne inéluctablement nécessairement une augmentation de l'activité des dites juridiction et de même, nous sommes évidemment particulièrement attentifs au profil socio-économique de la population d'un ressort donné on aura tendance à favoriser la localisation de poste de juge des enfants dans les départements à la population particulièrement jeunes, je pense par exemple à Mayotte, nous avons localisé en 2022 hein postes supplémentaires de juge des enfants, j'ajoute bien sûr que les évolutions démographiques et l'activité des juridictions ont également une incidence sur l'évaluation de la charge des magistrats, il s'agit d'un chantier qui est un chantier important qui sera finalisé, je l'ai dit, dans quelques jours et on pourra ainsi localiser les postes de magistrats au plus près des évolutions d'activité des juridictions et donc au plus près des évolutions démographiques des territoires, voilà la direction des services judiciaires suit donc avec attention ces évolutions démographiques pour y répondre, judiciairement au mieux.

dans les rapports sénatoriaux, le 2017, dont celui du sénateur Philippe Bas, dont on a parlé tout à l'heure, éloquemment intitulée 5 ans pour sauver la justice, espérons qu'il puisse enfin être suivie aujourd'hui. Merci, merci. La parole est à monsieur Gilbert Favreau pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, le rapport du comité des états généraux de la justice, présidé par monsieur Sauvé souligne la crise profonde de la justice, résultat de décennies de politique défaillante, ajoutant que seule une augmentation substantielle des moyens qui lui sont alloués, permettra de résoudre cette crise, le projet de loi de finances 2020 23 prévoit effectivement une augmentation de 8 % du budget de la justice qui serait porté à 9 heures 57 milliards d'euros, c'est un effort notable. Mais il sans doute insuffisant, surtout quand le rapport Sauvé. Se montre également particulièrement sévère avec les acteurs eux-mêmes de la justice, il considère qu'il faudra clarifier leur rôle dans la société et envisager une organisation globale de l'institution, mettent en garde les magistrats contre l'illusion de croire que la justice seule peut préserver son office et garantir son indépendance. Il faut, selon lui, maintenir les rôles respectifs du gouvernement et du Parlement dans les grandes orientations de la justice tout en associant plus étroitement le Conseil supérieur de la magistrature, mais à condition de questionner en même temps, le rôle et la composition de ce même Conseil supérieur de la magistrature, dans le souci de renforcer l'indépendance de la justice, au-delà des critiques faites au système judiciaire le rapport Sauvé souligne mais nous le savons tous la complexification et la multiplication du droit et des procédures, les délais de jugement excessif, l'augmentation des missions assignées à la justice, et surtout l'incompréhension des justiciables, alors que ce rapport affirme la nécessité du rêve d'une réforme, je vous pose la question, monsieur le garde des Sceaux a quand une grande réforme de la justice en France. Monsieur le garde des Sceaux. Elle arrive, monsieur le sénateur, elle arrive d'abord on a, on a, on a, on a pris connaissance des uns et les autres du rapport Sauvé puis des annexes tout ça été transmis le jour où le président sauvez a transmis son rapport au président de la République, ce jour-là les annexes de l'Europe ont été adressées à tout le monde, bon, j'ai reçu depuis les conférences des chefs de juridiction des chefs de cour, le Conseil supérieur de la magistrature, les forces de sécurité intérieure, j'ai reçu des citoyens qui veulent d'ailleurs que la justice, vous avez raison, aille plus vite et qu'elle soit mieux connu, d'où un passeport et du droit, que je mets en place avec Pape NDiaye, j'ai reçu les huissiers, les notaires, les syndicats qui ont voulu venir, enfin tout le monde, donc maintenant on est dans une phase d'arbitrage tout à l'heure, madame la sénatrice, il m'a dit que il fallait de temps en temps, si j'ose dire, être un peu directif concertation ne signifie pas mollesse les arbitrages seront pris naturellement vous y sera associé, loi de programmation début d'année prochaine, et puis le réglementaire va se mettre en place dans les meilleurs délais, parce que nous sommes dans une forme d'urgence. Il fallait réparer d'urgence avec les moyens Il Faut embauchée, ça c'est encore les moyens et en l'occurrence les moyens humains et il faut prendre des textes qui permettent une simplification une fluidité plus grande et donc une rapidité, une proximité et une protection meilleur pour nos compatriotes, donc tout ça étant est en autre et nous aurons très prochainement l'occasion de discuter de tout ça, vous donner le calendrier, je suis incapable, précisément, de le faire mais la feuille de route, c'est que le plan d'action sera prêt pour l'Automne que naturellement il sera communiqué discuter et que nous mettrons en oeuvre ce que

la parole est à Madame Christine Bonfanti Dossat pour le groupe Les Républicains. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, j'ai lu, non sans une certaine stupeur les préconisations définitive du rapport Sauvé relatives au cours d'appel, le groupe de travail scène a réfléchi, adapter les ressorts des cours d'appel aux populations en veillant à éviter qu'une cour d'appel ne dépendent de de de régions judiciaires distinctes, pourtant, il semble difficile de comprendre en quoi le fonctionnement de la justice serait améliorée en calquant la carte des ressorts des cours d'appel sur la carte des régions administratives, sinon tout au plus, de façon extrêmement marginale pour les parquets généraux, le groupe de travail raisonne en termes de limites administratives et non pas par rapport au bassin de population, ce même rapport reconnaît qu'une telle réforme souffrirait de plusieurs difficultés sérieuses et pour l'inciter que quelques-unes, l'activité de 15 juridictions seraient impactés 8 juridiction d'appel verraient leur activité réduite du fait de la réduction de leur ressort, soit plus de 25 qu'il s'agisse du rapport on pour les raisons que j'ai évoqué ou du rapport Sauvé, qui n'exclut pas la fusion des cours d'appel, l'avenir de nombreux au cours d'appel comme celle d'Agen semble menacée et condamné in fine et à disparaître, avez-vous pour projet de retirer au cours d'appel ne siégeant pas dans les grandes métropoles leurs prérogatives de gestion allez-vous retirer ses prérogatives à la cour d'appel d'Agen au profit de celle de Bordeaux. merci madame la présidente, mais madame la sénatrice, merci de me poser la question, ça va me permettre, je l'espère, une fois pour toutes, de répondre à ces préoccupations sur la suppression de telle ou telle cour d'appel alors je vois fleurir des initiatives assez singulière et récemment dans un théâtre des avocats se sont réunis pour dénoncer une suppression d'une cour d'appel, qui n'avait jamais été annoncé, j'ai appelé le bâtonnier, j'ai dit mais va c'est curieux, vous criez aïe, avant de recevoir un coup que personne ne veut vous portez donc je vais vous rassurer : il n'y a aucune suppression de cour d'appel, c'est clair et d'ailleurs. Et d'ailleurs, je veux rappeler que j'ai créé des tribunaux des audiences foraines et j'irai ouvert des tribunaux qui était fermé, parce que je pensais que la proximité ça doit et je pense toujours que la proximité ça doit résonner dans les territoires et que, à Agen, par exemple, bah il y a un certain nombre de nos compatriotes qui doivent prendre la route pour se rendre à la cour d'appel, c'est compliqué et il préférait par exemple l'audience foraine de Villeneuve-sur-Lot et les exemples, je peux les multiplier, voilà donc il est pas question de supprimer des cours d'appel, il n'en a jamais été question, merci, vraiment merci madame la sénatrice de me poser cette question, mais je suis pas convaincu que ce soit la dernière question de cette nature

mais simplement vous ne m'empêcherait pas de craindre que, si la cour d'appel d'un gêne deviennent secondaires, elle ne soit pas condamné à fermer, alors Monsieur le Ministre, je l'avoue, je plaide coupable, coupable peut être d'avoir raison trop tôt. Merci. Alors pour conclure le débat, la parole est à monsieur le questeur Philippe Bas pour le groupe Les Républicains et pour cinq minutes chers collègues. des Sceaux, vous n'aurez pas de droit de réponse. Madame la présidente, monsieur le garde mes chers collègues. Monsieur le garde des Sceaux. Ce débat n'a pas été organisée pour discuter de votre bilan, il a été organisée pour examiner ensemble les perspectives ouvertes par les états généraux de la justice, c'est un débat très intéressant je trouve, et vous avez eu à coeur de répondre généralement avec précision à l'ensemble des questions qui vous auriez été posées bien entendu je ne prétends pas en prenant la parole à cette tribune clore le débat, il va continuer entre nous parce que nous avons beaucoup de travail à faire ensemble et j'admets la manière dont vous avez présenté les choses, gouvernement et Parlement sur la justice, comme ils le font

dans la situation actuelle et puis se le garde, je sais à quel point vous êtes sensible à ce qu'on reconnaisse les efforts que vous faites et je veux bien le faire, mais si vous voulez que nous puissions travailler ensemble et que vous puissiez obtenir de concours du Sénat, il faut mettre les problèmes sur la table, c'est-à-dire pas seulement montrer les efforts qui sont faits mais aussi montrer les difficultés qui résiste au redressement de la justice, je vais essayer de le faire, très brièvement, parce que j'ai peu de temps ah transparence le réalisme sont les gages d'un dialogue équilibré entre nous, il y a que la question des moyens, monsieur le garde des Sceaux, il est absolument exact que depuis le gouvernement Castex et. Sous votre impulsion, les moyens de la justice ont fortement augmenté, il était également exact qu'il y a eu beaucoup de recrutements de magistrats, de greffiers, même si, s'agissant des greffiers, il y a encore des vacances de postes assez nombreuses, tout ceci n'est pas discuter entre nous, mais il faut aussi prendre la mesure, y compris sur le plan budgétaire et sur le plan des effectifs de difficultés qui subsistent sur le plan budgétaire, n'oublions pas tout de même que cette année est une année à plus de 6 % d'inflation quand vous augmenter le budget de 8 % ça ne fait pas 8 % de pouvoir d'achat supplémentaire je ne veux pas ainsi relativiser à l'excès l'effort qui est fait, mais il faut bien voir que si c'était 8 % de progression du pouvoir d'achat de la justice, évidemment, l'effet de souffle serait tout différent, et en réalité à peu près un quart du chiffre nominal de 8 % ça va être la même chose pour le budget de l'année prochaine et puis on voit bien qu'avec les problèmes de la défense nationale, en pleine crise ukrainienne, les problèmes de l'éducation nationale, l'épreuve de la santé, la bagarre et pour les Budgets de chaque grand service public est quand même très difficile, sachez que vous aurez notre soutien pour le redressement de la justice, parce que pour le Sénat, c'est un engagement de longue haleine, je dois dire aussi que, s'agissant de l'effort financier, vous répondez. Exactement sur la consommation des crédits de la justice mais, ce faisant, vous oubliez de préciser que vous avez un problème et que ce problème, nous voulons bien le faire nôtre c'est que vous n'arrivez pas dépenser vos crédits d'investissement et en 3 ans, c'est l'équivalent d'une année de crédits d'investissement que vous n'avez pas pu dépenser, nous n'ignorons pas qu'il y a eu le Covid, mais c'est pas la seule difficulté parce que cette avant le Covid qu'on avait déjà cette difficulté-là, ça se traduit ensuite par la difficulté que vous avez à réaliser le programme des prisons, alors là il y a quand même, je ne veux pas vous vous vous associez à ce tour de passe-passe mais enfin, le président de la République en 2017 annonce 15000 places de prison et disent : finalement, c'est sur deux mandats, heureusement qu'il en fait un deuxième et il dit on en aura fait sept mille et puis finalement, vous faites le compte, vous n'en avez pas fait 7000 le nombre de places nette ouverte et de 2080 donc quel travail mais je mesure aussi mettait les difficultés sur la table, je ne dis pas que c'était réaliste de dire d'un quatre monde doit, je vais faire 15000 places mais il se trouve que c'est un engagement présidentiel et par conséquent il faut réaliser que nous nous ne sommes pas donné les moyens d'atteindre ces résultats et que nous avons un énorme problème parce que nos prisons sont saturés et nous ne sommes pas d'accord avec la conclusion des états généraux qui consiste à dire pour incarcérer des condamnés, on va désormais libérer des détenus, ça ça ne va pas et donc nous avons besoin absolument de travailler ensemble et de faire en sorte que ces problèmes ne soit pas escamoté mais mise sur la table pour que nous puissions prendre des mesures plus fortes que celles qui ont été prises jusqu'à présent, voilà ce que je voulais vous dire je suis attaché aussi à la stabilité des règles, notamment en matière pénale et pour autant il faut simplifier le code de procédure pénale, nous avons de gros problèmes en ce moment parce que la police judiciaire est exsangue, elle a besoin d'être encadré par le parquet mais les règles sont tellement compliqués que nos malheureux policiers ont du mal à mettre en état des affaires qui permet ensuite aux magistrats de condamner comme il le voudrait, voilà ce que je voulais vous dire Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, cher collègue, merci.

La séance est reprise, l'ordre du jour hein peine le débat sur les urgences hospitalières et les soins non non programmés. La parole et tout d'abord à l'orateur du groupe, qui a demandé ce débat monsieur René-Paul Savary pour le groupe Les Républicains et pour huit minutes chers collègues.

le président, madame le président, mes chers collègues, notre groupe a souhaité inscrire ce débat afin de permettre au Sénat, de connaître les intentions du gouvernement en matière de politique de santé et plus particulièrement celles concernant les urgences maillon clé de notre système de soins. Un chiffre peu connu mais que je voulais souligner la saturation des urgences et concentrée sur un nombre relativement faible de patients qui vont en moyenne 5 fois par an aux urgences avec un délai médian entre 2 passages de 40 jours c'est énorme, c'est quelque 3 millions de patients réguliers des urgences sont surtout des personnes âgées polypathologiques des usagers qui n'ont pas d'autres recours médicaux à proximité, ainsi que des personnes exclues socialement et bien d'autres cas également, par ailleurs, n'oublions pas qu'en 2019 une grève massive des urgences a alerté les pouvoirs publics sur l'état dégradé des services alors comment sommes-nous arrivés là au fil du temps, des décisions ont été prises qui peuvent être lourd de conséquences, faut le reconnaître, pour certains, c'est la mise en oeuvre des 35 heures, il est vrai qu'on a demandé aux gens de compter leur temps, ce qui a entraîné une désorganisation au niveau de l'hôpital pour d'autres c'est la T2A, il faut reconnaître également que la T2A s'est traduit par une course à l'acte et cette tarification initialement instaurée pour compenser les difficultés de la dotation globale a eu un effet inflationniste parfois. Et du côté de l'hôpital, la difficulté. Tu es majeure, c'est la question de l'aval des urgences alors ça regroupe un certain nombre de dispositions et tenant compte des, des, manque de lits dans les services spécialisés, la pénurie de places dans des structures extra-hospitalières et lors des auditions en 2017 par notre commission un chef de service a bien résumé la question il disait que le principal problème n'était pas d'empêcher les patients de venir aux urgences, mais de réussir à les en faire sortir l'enjeu de la prise en charge en aval des urgences est double : il s'agit non seulement d'assurer le désengorgement de ces dix d'urgence, mais également de garantir le bon aiguillage des patients vers la sur une structure spécialisée de manière à éviter le retour aux urgences ou les hospitalisations multiples, les établissements de santé privés, les médecins de ville ne participe à tous également à la prise en charge de ces soins non programmés et là où le chirurgien Bernard Cros, auteur des blouses blanches colère noire les contraintes liées à une tarification insuffisantes les en ont détourné avec une tarification en moyenne 4 fois inférieur pour les actes non programmés par rapport à l'hôpital. Le défaut de formations participent également à cette crise, nous aurons, je pense, l'occasion d'en reparler et et les médicaux par les reste. Peu ouvert le soir pour accueillir les urgences à cause là aussi d'une rémunération peut-être pas suffisant, d'une adaptation de la vie professionnelle avec la vie familiale et maintenant il faut en tenir compte, bien sûr, de notre réflexion des point positif cependant, on peut souligner que certaines communes en plus en place des Sami, service d'accueil médical initial service médical de garde ouvert en soirée le week-end ou des médecins généralistes se relayent volontairement il traite les urgences en dehors des heures d'ouverture des cabinets médicaux, à côté de cela j'aurais échoué souhaité évoquer la situation post-Covid, qui est révélait du malaise de l'hôpital, mais pas uniquement, en mars 2020 la pandémie de Covid 19 a provoqué une vague importante de recours aux soins qui a mis le secteur hospitalier sous tension des hôpitaux ont dû s'adapter pour gérer l'afflux de patients, notamment dans les services d'urgence avec des transferts vers d'autres établissements et la mobilisation de la réserve sanitaire et ça a tenu le coup après plus de 2 ans de crise sanitaire là, rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la situation de l'hôpital a pointé cette aggravation du mal du malaise hospitalier et malgré une autorisation des ça des salaires pour les personnels soignants, selon l'accord de Ségur, la dégradation des conditions de travail, de l'ensemble des personnels a généré une désaffection qui est préoccupante à l'égard de l'hôpital, les à injecter n'ont pas produit les résultats se compter l'hôpital ce n'est pas qu'une question d'argent. La médecine libérale, également très engagé dans la crise sanitaire est elle-même en crise, les Français ont de plus en plus de mal à trouver des médecins traitants, on le sait, dans l'immédiat, ce n'est pas l'annonce de la fin du numerus clausus, qui va y remédier, ni celle de la 4ème année d'internat de médecine envisagée pour 2026 en ce qui concerne le bilan des mesures prises avant l'été, nous noterons que les propositions de la mission flash sur les urgences sont principalement axée sur la régulation, elle ne traite pas bien sûr des racines du mal mais nous l'avions déjà souligné ce problème de régulation et l'importance de redonner du corps au métier d'assistants de régulation médicale, madame la ministre, il y a des rendez vous à ne pas manquer, comme la convention médicale pour permettre aux médecins de ville, de prendre en charge plus de patients en libérant du temps médical en revalorisant l'activité libérale, mais également une conférence des parties prenantes, celle-ci doit associer l'ensemble des corps intermédiaires, les syndicats de professionnels de santé, association des usagers patients, représentants des collectivités qui n'ont pas souvent été entendus ni considérer ces dernières années, elle reposera, paraît-il, sur une approche globale de la santé et de la restauration de l'éthique, dixit le ministre de la Santé, derrière ces termes bien générique, il est difficile de cerner l'ambition réformatrice du gouvernement de sujets restent majeur pour l'avenir de notre système de santé à savoir bien sûr son financement, mais également sa gouvernance en conclusion, tous ces constats nous amène à penser qu'il est nécessaire de réformer structurellement et profondément notre système de santé la situation tendue aux urgences n'est qu'une facette d'un mal profond, aujourd'hui nous ne sommes plus dans une problématique d'accès aux soins à plusieurs vitesses, mais dans celle de l'accès aux soins tout court. Les manifestations s'enchaînent pour composer ou trouver des solutions à l'accès aux soins urgents de la population persuadés que c'est au niveau des territoires avec les acteurs du soin et de la prévention avec les patients, avec les élus que doivent être élaborés des réponses concrètes et pérennes, voici quelques éléments que je souhaitais, au nom de mon groupe, formulées en préambule, madame la ministre, vous qui vous déplacer sur les territoires, nous avons eu l'honneur de vous recevoir, vous qui êtes spécifiquement chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé, entendez notre message et n'hésitez pas à nous, on a nous exposer vos ambitions pour cette mandature, je vous en remercie. La parole est à Madame Agnès. Firmin Le Bodo Ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé et pour une durée de 8 minutes maximum. Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis honoré de m'exprimer devant le Sénat, sur un sujet qui nous tient tout particulièrement à coeur et qui est au centre des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens pour ce débat sur les urgences hospitalières et soins non programmés. Les difficultés que cristallise nos urgences sont le symptôme aigu d'une crise plus large qui touche l'ensemble de notre système de santé, celle de l'accès aux soins nos urgences sont ainsi le point de convergence des fragilités structurelles qui parcourent notre système de santé, démographie médicale inadapté, difficultés d'articulation entre la ville et l'hôpital, perte d'attractivité et de sens de certains métiers, désertification médicale, un système de santé qui doit pourtant à bien des égards, faire notre fierté, en effet, nous pouvons être fiers de notre système de santé fier des valeurs d'égalité et d'universalité, sur laquelle il est fondé, nous pouvons être fiers de notre système de santé qu'il a fait preuve d'une remarquable résilience pendant les vagues successives de Covid qui ont ébranlé notre pays à ce titre, je pense qu'il n'est pas excessif de saluer une fois encore la mobilisation exemplaire de nos soignants. La crise des soins non programmés et les difficultés d'accès mettent en péril l'essence même de ce système de santé qui est notre héritage commun, nous nous devons d'entreprendre les réformes nécessaires pour le préserver, autant pour faire face aux défis du présent que pour les générations à venir dans cette perspective, la première urgence consiste assurément à repenser l'organisation de la prise en charge des soins non programmés, les attentes des professionnels de santé, comme de nos concitoyens sont fortes et légitimes en la matière, le gouvernement a répondu présent dès son installation, les 41 mesures opérationnelles de la mission flash menée par le ministre est médecin urgentiste François Braun avant sa nomination, ont permis de mobiliser des leviers nouveaux pour répondre au défi immédiat des urgences durant la période cruciale de l'été. Je le dis sans triomphalisme et avec la gravité qui sied à ce sujet la catastrophe annoncée, ne s'est pas produite. Et notre système de santé a globalement tenu certes cela ne fut pas sans effort et nous devons avant tout saluer la mobilisation des professionnels et de nos administrations impliquées dans la mise en oeuvre de ces mesures transitoires dont certaines pourraient être rapidement pérenniser en effet l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS vient de remettre un rapport d'évaluation de ces solutions, nous sommes en train d'instruire les données de cette évaluation et allons prochainement réunir une nouvelle fois le comité de suivi d'ici une dizaine de jours pour travailler sur les mesures à conserver, nous pouvons cependant déjà tiré un bilan positif de ces mesures. Elles ont mobilisé les professionnels dans une logique de responsabilité collective, partagée entre la ville et l'hôpital, elles ont enfin sensibiliser nos concitoyens à la fragilité du système de santé en général et des soirs nos pratiques non programmés en particulier générant des premiers changements notables de comportement chez les Français, notamment dans le recours aux urgences et l'appel préalable au 15 une idée forte de cette mission, sur lequel je tiens à insister et de retrouver le sens de ce que signifie urgence une urgence médicale se définit d'une façon précise qui la distingue par nature d'un soins non programmés, c'est une situation requérant une intervention médicale immédiate afin de secourir une personne dont le pronostic vital au fonctionnel et susceptible d'être engagée l'urgence relève ainsi nécessairement d'une décision médicale et répond à des critères stricts et limitatif, or, au cours des 20 dernières années, le nombre de passages aux urgences, a plus que doublé, nous le savons, c'est public qui se présentent aux urgences sont en partie et même souvent ceux qui n'ont pas accès autrement à notre système de santé parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant parce qu'ils ne parviennent pas à obtenir un rendez-vous dans un délai rassurant, c'est en cela que les jours Jeanson, comme je le disais un symptôme du malaise que nous connaissons. Nos urgences sont en quelque sorte victimes de leur succès et cela pèse sur la sécurité des patients l'inflation du recours crée des situations d'engorgement, et le temps de passage aux urgences, a, de ce fait beaucoup augmenté il n'est pas question de limiter ou de restreindre de quelque manière que ce soit l'accès aux soins, encore moins de filtrer ou de trier les malades comme certains ont pu le laisser entendre parfois certes sous l'effet d'une inquiétude légitime mais parfois guidé par des motifs politiques, il s'agit donc de replacer chacun dans son rôle, le long de la chaîne de prise en charge afin de se donner les moyens de proposer à chacun, à chaque patient le parcours de soin le plus adapté à sa condition concentré les urgences sur leur coeur de missions et leurs plus-values nécessite ainsi un travail de régulation pluri-dimensionnelle que nous avons mis en place la meilleure orientation dans le système de santé a fait l'objet d'une campagne de sensibilisation sur le bon usage des services d'urgence, il est en effet important de faire évoluer les mentalités, d'où cette campagne menée depuis plusieurs mois pour inviter nos concitoyens, a contacté avant toute chose le 15 pour être orienté vers la meilleure solution à leur problématiques de santé pour reprendre un slogan de l'assurance maladie que nous avons tous encore à l'esprit les urgences, c'est comme les antibiotiques c'est pas automatique, cet effort de pédagogie. Il est couplé. Ah, une mise à niveau des des effectifs d'assistants de régulation médicale ARM dans les SAMU centre 15 et un renforcement du déploiement du service d'accès aux soins, notamment par leur ouverture à l'ensemble des professionnels de santé pour favoriser le développement des filières directe de prise en charge dans d'autres spécialités médicales, en effet, la régulation des urgences est un sujet transversal qui dépassent les murs des hôpitaux et doit mobiliser l'ensemble du système de soins par optimisation du temps médical et l'augmentation des capacités de réponse non programmés en ville. Le comité de suivi de la mission flash nous a permis d'avoir en continu, un tour d'horizon du déploiement de l'application et de l'effet de nos mesures en ce sens, ainsi nous savons que les mesures dérogatoires de l'été ont permis de faciliter le recrutement d'assistants de régulation médicale ces professionnels ont, à leur plus orienter les patients dont l'état le justifiait vers des cabinets médicaux en ville, où des maisons médicales de garde dont le nombre de maisons ouvertes le samedi matin, a quasiment doublé sur la période considérée, sur prescription de la régulation, les ambulanciers ont d'ailleurs pu être mobilisés en assurant un transport sanitaire des patients vers ces structures. Preuve de la nécessité de renforcement des effectifs et du succès de la démarche, le nombre de recours au quinze a augmenté de 20 % au cours de l'été, l'appel au quinze est en train de devenir un réflexe et c'est ce que nous souhaitons. Et nous avons assumé la responsabilité d'absorber cette hausse, notamment en donnant toute leur place aux médecins rêves libéraux régulateurs, le renforcement des équipes de régulation est ainsi une mesure que nous avons souhaité inscrire dans le temps long, dès le projet de loi de finance de la Sécurité sociale pour 2023 dans le budget de la Sécurité sociale qui arrivera très prochainement devant votre assemblée nous renforçons en effet les équipes médicales, en charge de la régulation grâce à 2 leviers nous encourageons la reprise d'activité des médecins retraités sur des activités de régulation médicale téléphonique en les faisant bénéficier du régime simplifié des professions médicales, ce qu'il fallait facilite les démarches administratives, nous permettons à tout médecin participant à la régulation en dehors de la permanence des soins ambulatoires de bénéficier de la couverture assurantielle de l'établissement, support du centre de régulation pour éviter que les médecins n'aient à souscrire individuellement un contrat d'assurance, ce qui était une de leurs revendications, ancienne le PLFSS comporte par ailleurs une autre mesure forte liée aux urgences, qui est l'exonération du ticket d'orateurs sur les transports sanitaires urgents pré-hospitalier, cette mesure s'inscrit dans notre politique volontariste en faveur de l'accès aux soins dans un contexte d'urgence en supprimant le reste à charge des bénéficiaires qui n'auront plus rien à débourser, tout cela est efficace, puisque le nombre de passages aux urgences, toutes causes confondues Abéché de fête de mesure de l'ordre de 5 % à l'été 2022 par rapport à l'année dernière, c'est un progrès concrets une tendance encourageante que nous devons confirmer et approfondir un autre chantier majeur que nous devons nous être celui de la pénibilité du travail de nuit que la mission flash sur les urgences et soit nos programmé a reconnu pour la première fois, celle-ci a été mieux valorisés grâce à la majoration des indemnités de nuit pour les personnels non médicaux et la majoration des indemnités de garde pour les personnels médicaux je tiens également à souligner que la hausse du point d'indice à hauteur de 3 Himad qui a. Et Madame la Ministre, je je garde des, je vais vous demander de conclure : oui Notre ambition, avec le ministre de la Santé et de la prévention et de fonder un nouveau modèle pour répondre toujours mieux aux besoins de santé de nos concitoyens partout sur le territoire, aujourd'hui et demain, je vous invite donc à participer au CNR en santé, qui aura lieu dans vos régions, respectivement, je vous remercie. dans la suite du du débat s'il vous plaît, chaque orateur dispose de deux minutes maximum, y compris l'éventuelle réplique et le gouvernement Madame la Ministre. Dispose pour répondre d'une durée équivalente de deux minutes maximum. Le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire de répondre à une réplique pendant une minute et l'auteur de la caisse. Si on disposera à heure à son tour du droit de répondre en pendant une minute et je passe tout de suite la parole à Madame Patricia Schillinger pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Merci madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues, affaibli par 2 ans de crise sanitaire notre système de santé a connu cet été une situation de tension majeure: les services d'urgence menacés de ne pouvoir assurer la continuité des soins durant la période estivale, si les difficultés rencontrées par ses services, ce sont que des que le symptôme d'une crise plus large touchant notre système de soins à l'hôpital, il a fallu rapidement trouver des solutions, la mission flash commandées par le président de la République a ainsi formulé de nombreuses recommandations, l'une d'elle consistait en la possibilité de réguler les entrées au service d'urgence de manière à orienter les patients dont l'état de santé ne révèle pas de la médecine d'urgence vers une offre de soins adaptés, l'engorgement des urgences se voit ainsi aggravée par la désertification médicale de nombreux patients se tournent en effet vers les urgences pour des soins auxquels pourrait répondre : la médecine de ville ou d'autres professionnels de santé, la mission flash a notamment fait le choix d'accroître le recours à la télémédecine dont la crise sanitaire, a mis en en évidence la pertinence et les bien fait plus largement le numérique constitue un vivier potentiel d'outils qui demeure en France largement sous-exploité le Danemark peut nous inspirer, en effet, en s'appuyant largement sur ces nouveaux outils, l'hôpital et la médecine de ville sont utilisés en complémentarité, tout en préservant caractéristique d'université s'aliter d'accessibilité, madame la ministre, quelle place, entendez-vous accorder à l'innovation numérique dans la transformation nécessaire de notre système de santé et pensez-vous poursuivent le développement du recours à la télémédecine dans le but de répondre de manière pérenne à la crise des urgences

les gaz dans le rapport sur l'évaluation des mesures de l'été, a d'ailleurs mené un travail de comparaison avec le système danois qui fait de la régulation préalable, une condition d'accès aux urgences, constitue un outil intéressant pour favoriser l'accès aux soins dans les territoires les moins bien dotés et une facilité supplémentaire pour tous, le gouvernement a d'ailleurs soutenu le développement de ces téléconsultations puisqu'elles ont été prises à 100 % % à partir du début de la crise sanitaire jusqu'au 30 septembre 2022 les téléconsultations ont représenté en 2021 environ 5 % du nombre total des consultations des médecins généralistes, par ailleurs, dans le cadre des mesures de l'été 2022 faisant suite aux recommandations de la mission flash sur les urgences et les soins mon coup non programmés, le recours aux unités mobiles de téléconsultation a été encouragés dans des situations qui ne relèvent pas de l'urgence vitale, il s'agit d'envoyer une infirmière au domicile du patient pour organiser une téléconsultation et assurer un 1er niveau de prise en charge du patient, si nécessaire, le rapport de l'IGAS sur l'évaluation de ces mesures soulignent l'intérêt de ces téléconsultations dans ces situations ne ne donne pas lieu à un passage aux urgences nn ou à une hospitalisation dans 75 % des cas, c'est donc bien un outil qui permet d'éviter des passages aux urgences, néanmoins, nous souhaitons maîtriser le développement de la télémédecine, d'abord parce que nous devons rester vigilants à ce qu'une possibilité de prise en charge physique puissent toujours être garanti pour les situations des soins urgents ou de soins non programmés, ensuite parce qu'il ne faut pas que le développement d'tel médecine viennent retirer des médecins implantées dans les territoires pour les spécialiser sur un exercice exclusivement digitale, enfin, nous devons lutter contre les dérives que nous voyons apparaître avec le recours à la télé, consultation c'est pour soi, nous limitons la prescription d'arrêt de travail en téléconsultation au seul médecin traitant ou un médecin déjà connues du patient face aux abus qui ont pu être détectés dans certaines situations. Madame Schillinger vous avez non merci. Alors la parole est à madame Annie Le Houerou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues, personnels, épuisés, surmenés, accroissement des départs en cours de carrière, difficultés de recrutement, l'hôpital public est en crise sans précédent malgré les revalorisations Sana salariale, la dégradation des conditions de travail, cumulé à la difficulté d'accès aux soins, aux soins en ville provoque l'engorgement voir la saturation des urgences et la fermeture de service, l'accès aux soins s'annonçait très problématique, ce début d'été vous amenant à un plan pour les urgences et pour les soins non programmés, selon vous, des réponses rapides et fortes pour l'été une régulation de l'accès aux urgences, via le quinze, une plus grande disponibilité des professionnels déjà très éprouvée, la mobilisation des hospitaliers va via des majorations de rémunérations, la recherche d'une meilleure coordination des acteurs déjà très mobilisés ne sont que des réponses conjoncturelles pour que notre système de santé passe l'été, l'été est passé si le pire a souvent été évitée, parfois pas, c'est grâce au dévouement à la mobilisation sans faille des personnels soignants à qui je témoigne ici de notre grande grande reconnaissance les recommandations de la mission flash ont été insuffisantes et ne permettent pas d'assurer un fonctionnement sécurisé optimal pour une prise en charge de qualité, la difficulté rentre rencontrer sont caractéristiques d'une crise profonde du système de soins et de l'hôpital, Madame la Ministre, quelles sont vos propositions pérenne, durable, garantissant un accès aux soins à tous, quelle que soit la l'endroit où ils se trouvent, sur notre territoire national concertée au travers du Conseil national de la refondation par des réunions moment hier comme au Mans hier pour imaginer des solutions innovantes ne me paraît pas être une méthode efficace le diagnostic partagé, nous l'avons vu dans vos propos, il est urgent de décider de la refondation de notre système de santé au service des patients d'abord et permettant aux soignants d'excès dans la sérénité, quel est votre calendrier et pour quelles priorités. D'action Nous devons répondre à cette question de manière globale, en ne regardant pas seulement le fonctionnement des urgences de services d'urgence fondée face à des tensions majeures qui reflète les difficultés de notre système de santé, en effet, les urgences se retrouvent à la jonction entre les difficultés en amont de la ville et les difficultés en aval des services hospitaliers mot aurait durablement la situation, nous devons mieux répondre à la demande croissante de soins non programmés et non urgents qui contribue à l'engorgement massif de nos urgences il y a tout d'abord les services d'accès aux soins, ce service se déploie progressivement sur le territoire national et a vocation à pouvoir aider les citoyens à s'orienter dans le système de santé pour le patient, confronté à un besoin de soins non programmés et lorsque l'accès à son médecin traitant n'est pas possible, ou s'il n'a pas de médecin traitant le sas permet d'accéder par téléphone à un professionnel de santé, ce dernier pourra lui fournir un conseil médical lui proposer une téléconsultation l'orienter selon la situation vers une consultation de noix de soins non programmés en ville vers un service d'urgence ou déclencher l'intervention d'un SMUR selon son état de santé, l'objectif d'un sas et d'apporter une réponse pour des besoins de soins urgents ou de soins non programmés sous 48 heures lorsque le médecin traitant ou un médecin de proximité n'est pas disponible en première intention, il repose sur la mise en place d'une chaîne de soins lisible et coordonnée entre les acteurs de santé, de l'hôpital et de la ville d'un même territoire, incluant une prise en charge des appels des passions communes entre les médecins urgentistes Les médecins généralistes une mobilisation des médecins généralistes effecteur pour prendre en charge en journée les les patients préalablement régulé par le sas, nous devons accélérer le déploiement du ça sur tout le territoire national en 2023, c'est une nécessité, nous savons aussi que nous devons travailler notamment sur l'attractivité des métiers pour favoriser le maintien des professionnels de l'urgence dans leur domaine d'activité, par ailleurs, il n'y aura pas de solution unique, mais un panel de mesures qui sera décliné sur chaque territoire, hier c'était le lancement du CNR devant 400 personnes s'étaient pas les ateliers de travail qui ont eu lieu le vendredi, la méthode du CNR, c'est ce qui c'est qui ce c'est au Mans, des ateliers de 15, 20 personnes qui travaillent pour apporter des solutions. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, avec plus de 20 millions de passages par an, les services des urgences dans les hôpitaux sont confrontés à de graves problèmes d'engorgement du fait d'un manque criant de généralistes et d'une pénurie de personnel hospitalier qui démissionne massivement pour ne plus subir la maltraitance institutionnelle de décennies d'austérité, de moyens humains et financiers 10000 médecins sont formés chaque année comme en 1975 Madame la Ministre, or depuis 47 ans, la population a augmenté de 30 % avec des besoins plus importants car elle est vieillissante et présente des poly- pathologies, le président de la République a confié au Docteur Braun, futur mais mais Ministre une énième mission flash, donc j'avais avec mon groupe critiquait l'utilité puisque les constats et les propositions alternatives sont connus depuis des années et les rapports, y compris du Sénat ont tous pointé le désengagement financier de l'État dans les hôpitaux, entendent le ministre-Brown la boîte à outils de 41 recommandations, a permis de sauver le système alors que ce sont les personnels qui l'ont sauvé au prix d'un épuisement et d'une dégradation subit des conditions de prise en charge des malades madame la Ministre, que pensez-vous de notre proposition d'un service public de soins primaires construit autour d'un réseau de centres de santé pluri-professionnelles allez-vous et rétablir l'obligation de la permanence des soins ville hôpital pour tous les médecins, y compris les spécialistes exerçant dans le privé. Madame la présidente, madame la sénatrice tout d'abord, la boîte à outils et ses quarante, mais d'urgence, on paye ont permis de tenir bon, c'est très clairement ce que nous disons avec beaucoup d'humilité, la boîte à outils, a permis de tenir bon, grâce à l'investissement des personnels et je crois l'avoir dit très clairement la place des centres de santé dans la permanence des soins doit être renforcée, nous avons commencé à en parler avec les représentants des centres de santé qui, s'il partage le principe d'une participation mettent en avant, de difficulté logistique que nous avons travaillé avec eux les charges logistiques, tout d'abord ouvrir un centre de santé aux horaires de la permanence des soins nécessite une logistique lourde car il faut également ouvrir l'accueil et le fonctionnement de la structure, même s'il y a un seul cabinet merdique médical de permanence, une des solutions identifiées pour être aide-d'effectuer cette permanence dans une maison médicale de garde, la rémunération de l'astreinte les personnels intervenant dans ces centres de santé sont salariés et les rémunérations sont aujourd'hui versées à l'employeur, ces sujets ne sont pas insurmontables et nous souhaitons les travailler dans la concertation avec les représentants des professionnels de santé pour trouver les voies et moyens de permettre au Centre de santé de mieux s'insérer dans la permanence des soins, le principe est clair : nous souhaitons que tous les médecins d'un territoire participent de manière équitable à la permanence des soins pour mieux partager l'effort et faire vivre cette logique de responsabilité collective. Madame Cohen, vous avez 35 secondes. Oui, je me réjouis que vous souteniez effectivement l'effort des Centres de santé, j'espère que vous allez aider à ce qu'il se développe dans tous les territoires, ça serait déjà une première chose j'entends également que vous allez discuter pour qu'il y ait des gardes qui soient prises par les médecins qui travaillent dans le privé et bien écoutez, c'est une bonne chose, il faut je crois que c'est le le décret Mattéi qu'il faut faire sauter, mais il faut agir en amont, madame la ministre, y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant, et il faut agir en aval parce que le dernier chiffre que vous avez publié 4300 lits supprimés en 2021 n'est pas de nature à nous rassurer donc, Madame la Ministre, au lieu de simplement vous abriter derrière les 41 mesure de cette mission flash, il faut vraiment vraiment aller plus loin, plus vite, il y a urgence. Parole est à Madame Jocelyne Guinness pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, force est de constater comme tout comme nous tous de réalité d'abord l'engorgement des services d'urgence avec des conséquences en chaîne sur l'hôpital et sur la qualité de vie au travail des soignants, ensuite le problème d'accès aux soins dans les territoires face à ces difficultés, je voudrais mentionner le rapport législatives de ma collègue Élisabeth Doineau concernant la création de points d'accueil pour immédiat madame Nice je rappelle que c'est pas, il n'aurait pas vocation à ajouter un étage au mille-feuilles, puisqu'il s'appuieraient sur les structures existantes, les dispositions de cette proposition permettrait aux directeurs généraux de l'Agence Régionale de Santé de labelliser pour 5 ans sur l'initiative des soignants, des structures destinées à prendre en charge des soins non programmés ces points d'accueil seraient créés sous plusieurs conditions, en particulier leur inscription dans un projet territorial de santé ou le projet de santé d'une ou plusieurs communautés professionnelles Thierry territorial de santé c'est pas assurer une prise en charge, intermédiaire entre le cabinet médical et le service d'urgences pour des soins qui ne relèvent pas de l'urgence médicale comme la petite traumatologie et contribuerait ainsi à la permanence des soins, le cas échéant le SAMU pour orienter soit vers un Pasi, soit vers les services d'urgence avec mes collègues du groupe Union centriste je souhaiterais savoir Madame la Ministre, si le gouvernement conserve comme son prédécesseur, un avis favorable quant à ce dispositif, voir s'il envisage de se l'approprier, je vous remercie. Madame la présidente, madame la sénatrice la réponse ce soins non programmés, doit être amélioré, c'est une nécessité, elle manque de visibilité pour nos concitoyens, même si le service d'accès aux soins en cours de déploiement facilite l'accès à une consultation non programmés, la proposition de loi Pasi contient des éléments intéressants pour permettre de rendre plus visible, les solutions alternatives aux urgences, il convient cependant d'être vigilant face aux solutions qui spécialiste des professionnels de santé dans la réponse aux soins immédiats en effet les premiers retours disponible, il apparaît que certains centres de soins immédiats n'assure pas le rôle du médecin traitant, or face au développement des pathologies chroniques, nous devons consolider la place du médecin traitant et le tenir informé les points d'accueil pour son immédiats doivent découler d'un projet d'organisation partagé entre tous les acteurs d'un même territoire, il paraît important que ces points d'accueil émerge plus particulièrement au sein des C Pts et en étroite articulation avec les organisations ambulatoire et les établissements du territoire, et non pas en concurrence, il convient aussi d'éviter que ce type de structure constitue un appel d'air pour les médecins urgentistes, alors même que les services d'urgence ont du mal à les recruter, enfin, pour améliorer la réponse en soit non programmés, je souhaite que nous puissions trouver des solutions locales qui permettent une large partie participation participation du plomb grand nombre des professionnels de santé aux dispositifs de permanence des soins plus aucune de plutôt que d'une spécialisation d'un petit nombre ainsi notre proposition et de travailler un meilleur encadrement des structures qui se spécialise dans le soin immédiat. Merci madame guider, hein, vous avez 30 secondes non merci, donc, la parole est donc à Madame Véronique Guillotin, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci madame la présidente, madame la Ministre de la question va être un peu près similaire et je souhaite effectivement vous vous interrogez sur les centres de soins non programmés ou centres de soins immédiats qui ont commencé effectivement à s'installer sur de nombreux territoires ils prennent en charge sans rendez vous des patients dans un état peu grave, ils ont à leur disposition, du petit matériel technique et permettent la plupart du temps d'éviter un passage aux urgences, nous en avions débattu, il y a, il y a 2 ans, à l'initiative du groupe Union centriste et sur la base d'une proposition de loi venus de l'Assemblée, je n'ai j'y étais à l'époque, pas spécialement favorable, un an après la vote le vote de la loi, ma santé 2022, et alors que le Ségur se mettait en place, nous avions effectivement à l'époque, toutes les raisons d'espérer, depuis malheureusement la situation ne s'est pas vraiment améliorée, ce week-end encore aux urgences d'un des hôpitaux de mon territoire, une jeune fille de 18 ans a passé plus de 36 heures seul un problème de vertèbre sur un brancard aux urgences et je parle pas d'un lit dans un box, mais on voit bien que la situation est compliquée et selon les soignants, ils ont qualifié ce week-end de week-comme jamais dans ce contexte, toutes les initiatives, me semble-t-il, qui vise à mieux prendre en charge le bon patient au bon endroit, doivent être soutenus et le modèle de centres de santé non programmés divise le ministre de tutelle, monsieur François bonne n'a d'ailleurs pas caché ses réticences sur le sujet, alors certes c'est pris en charge se font hors parcours de soins mais comme la prise en charge aux urgences d'ailleurs avec un modèle économique, je vous l'accord peu satisfaisant pour le moment et des professionnels ayant parfois renoncer à leurs pratiques hospitalières pour des conditions de travail plus acceptable, ils ont la conviction mais je la partage, que l'insertion de ces centres de soins non programmés, si on y veille et qu'on mette des des conditions nécessaires dans un paysage sanitaire et dans l'offre de soin de chaque territoire peut se faire à condition que l'on trouve en concertation, un modèle, pérenne pour ces structures aussi j'aimerais connaître, Madame la Ministre, les intentions du gouvernement pour que ces centres de soins non programmés s'intègre dans notre système de santé sur la base d'un modèle qui soit acceptée et acceptable pour l'ensemble de la chaîne de soins. Merci madame la ministre. Madame la présidente, madame la sénatrice les centres médicaux de soins immédiats sont un objet relativement similaire au point d'accueil pour soins immédiats évoquée par votre collègue précédemment leur développement peut être bénéfique, je l'ai déjà dit, c'est notamment le cas des centres trompe horaire qui ont pu se monter cet été, souvent à l'initiative de personnels de santé libéraux désireux d'offrir une offre de soins non programmés afin de soulager les tensions dans les services d'urgence ces initiatives peuvent également avoir des effets regrettables en spécialisant des ressources médicales sur des prises en charge aiguë et en délaissant les patients ayant besoin d'un suivi chronique, c'est un véritable écueil, en effet, certains de ces centres, indique clairement refusé d'être le médecin traitant des patients, or nous souhaitons remettre le rôle du médecin traitant au centre des parcours de prise en charge ces centres médicaux de soins immédiats doivent découler d'un projet d'organisation partagé entre tous les acteurs d'un même territoire, donc il est important, je le redis que ces projets s'articuler autour des chez PTS, et sans doute, peut-être que la prise en charge de soins immédiats seraient plus effectives, il convient aussi d'éviter, je l'ai redit, mais je pense que c'est important de le redire que ce type de structure constitue un appel d'air pour les médecins urgentistes, alors même que les services d'urgence ont du mal à à les recruter et vous avez souligné ce fait vous-même notre position et donc de travailler un meilleur encadrement de ces structures qui se spécialise dans le soin immédiat. Merci, Madame le Ministre. La parole est à Madame Dominique Estrosi Sassone pour le groupe Les Républicains. merci, madame la. Présidente, Madame la Ministre, le 11 juillet dernier un pic de 310 admission a été enregistré en une seule soirée au CHU de Nice, ce flux a pu être régulé in-extremis grâce au filtrage médical efficace du SAMU 06 qui à réorienter les patients vers cinq autres hôpitaux du département ou vers des cliniques privées, les plus grandes inquiétudes ont plané tout l'été, avec bien sûr la forte affluence estivale, aggravant la saturation quotidienne déjà constaté malgré l'engagement sans faille de l'ensemble des professionnels de santé qui oeuvrent avec dévouement pour soigner au mieux toutes les personnes qui se présentent la risque la situation reste très préoccupante, l'organisation en sous-effectifs fait craindre à tout moment un défaut de vigilance médicale et les professionnels de santé sont en souffrance d'une charge de travail toujours plus grande, banalisant l'inacceptable puisque certains patients reste plusieurs heures sur des brancards, à cela s'ajoutent les violences dont sont victimes les professionnels de santé, en raison surtout des temps d'attente plusieurs agressions ont été constatés au CHU Pasteur de Nice à l'hôpital Lenval, mais également à Cannes alors Madame la Ministre, non comme notre système de santé n'a pas globalement tenu comme vous l'avez dit dans vos propos, non, oui, notre système de santé est en train de s'effondrer, nous n'avons pas besoin d'un nouveau diagnostic mais que proposez-vous concrètement comment entendez-vous mobiliser durablement les médecins de ville pour épauler les structures hospitalières allez-vous entendre enfin les demandes de SOS Médecins dans le réseau ne cesse de se déliter dans les territoires, alors que les structures locales sont de nature à éviter l'embolisation des services d'urgence. merci, même la ministre. Madame la présidente, madame la sénatrice, je tiens tout d'abord à redire oui que cet été, les urgences ont tenu la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu, elles ont tenu grâce à la forte mobilisation de nos soignants, elles ont fortement tenu grâce à la mobilisation de nos soignants que je souhaite vivement remercié de fait, les établissements sont parvenus à organiser leur fonctionnement en se saisissant des opportunités qui leur a été offerte d'aménager les parcours des patients et des mesures prises pour valoriser la pénibilité du travail, s'agissant de la situation du CHU de Nice, le secteur des urgences a fait face à une activité soutenue en juillet et en août, 230 passages en moyenne par jour, ce pic d'activité combinées aux difficultés de ressources ont conduit début juillet à une seule occasion à la mise en place une procédure de fermeture partielle du service des urgences de Nice pendant 5 heures la solidarité territoriale, vous l'avez souligné cette exercer a permis un rétablissement rapide des conditions normales de prise en charge en rayon en réorientant moins de 20 patients pendant ce court intervalle sur près de 14000 passages sur la période estivale, au plan national, à la faveur d'une grande communication nationale, le nombre de passages aux urgences a décru de manière sensible, ce qui constitue un actif réel est certainement le plus marquant du plan été avec moins de 5 % de passages aux urgences en miroir le nombre d'appels au quinze à augmenter significativement le sujet n'est pas celui des moyens qu'on ne donnerait pas au service d'urgence, le sujet est d'abord celui des postes vacants non pourvus faute de candidats, les médecins urgentistes choisissent ainsi parfois d'autres modes d'exercice et il nous faut travailler sur les conditions de travail pour favoriser le maintien des personnels en poste, attirer les jeunes médecins et faire revenir ceux qui sont partis, enfin, il faut le souligner les initiatives remarquables mises en place dans plusieurs territoires, en particulier celles autour d'une mobilisation renforcée des professionnels paramédicaux télémédecine embarqué astreintes d'infirmières libérales ainsi que la collaboration entre professionnels. Compte parmi les enjeux de la reconquête du temps soignant dans nos territoires, ces initiatives doivent être fortement soutenu et leur passage à l'échelle encourager car elles permettent de décharger les services d'urgence de passage évitable en mobilisant utilement l'ensemble des composantes de notre système de santé. Madame Estrosi Sassone vous avez 15 secondes. Alors, je le répète. Santé va mal, il s'effondre, il faut guérir le malade avant qu'il ne soit trop tard. Mais si la parole est à Monsieur Daniel Chassain pour le groupe, les indépendants. Madame la présidente, madame Namyst mes chers collègues, les services d'urgence hospitaliers sont un maillon clé de notre système de soins chaque année près d'un Français sur 6 se rend aux urgences, les urgences hospitalières se trouve actuellement dans une situation critique en effet tout en continue à assurer une prise en charge de pointe, elles sont confrontées à un personnel souvent soignants souvent en sous-effectif et la carence de lits d'aval, faute de lits, les patients vont en Bolliger les services d'urgence qui se trouve déjà sous tension, la problématique, bien sûr, c'est d'assurer les besoins de santé des Français l'égalité d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire et la prise en charge d'une partie croissante de soins non programmés, due à un manque de médecins libéraux, Madame la Ministre, en 1er lieu quelles réponses concrètes entendez-vous apporter afin de remanié à la pénurie d'infirmières qui conduit à fermer des lits d'aval par manque de personnel et qui entraîne une embolisation des urgences : que comptez-vous faire également pour qu'il y ait davantage de médecins urgentistes cette infirmière au sein des urgences hospitalières en second lieu, envisagez-vous de mettre l'accent sur un service de soins non programmés pour les cas peu grave en amont, tout proche du service des urgences afin de désengorger celle-ci enfin quelle solution entendez-vous mettre en oeuvre afin d'avoir plus de médecins généralistes dans les maisons de santé pluridisciplinaires, ne faudrait-il pas obliger des médecins en dernière année de 3ème cycle a

en incluant les six derniers mois mais avec un classement en médecin, insistant pour avoir la même rémunération que le médecin installé merci. Merci madame la ministre. Madame la présidente, monsieur le sénateur, nos services d'urgences font face à des tensions majeures, ça a été déjà dit plusieurs fois, qui reflète les difficultés de notre système de santé, en effet, les urgences se retrouvent à la jonction entre les difficultés en amont de la ville et les difficultés en aval des services hospitaliers. Nous avons de trop nombreux postes vacants mais je tiens à le souligner, pour éviter toute ambiguïté, non par manque de financement, mais par manque de candidats cette mesure et de ressources humaines concerne cette pénurie de ressources humaines concerne tous les services hospitaliers puisqu'au plan national 30 % des postes de praticiens hospitaliers et 6 % des postes infirmiers, vous l'avez souligné sont vacants, nous travaillons à démarche forte pour favoriser l'attractivité des métiers du système de santé, c'est d'ailleurs l'un des axes majeurs du Conseil national de la refondation enchanté que j'ai lancé au Mans avec le ministre de la Santé et de la prévention hier mais nous apportons aussi des solutions de court terme, c'était tout l'objet des mesures de la mission flash de cet été, avec la possibilité, dans chaque territoire de mobiliser les solutions réunis dans une boîte à outils ont ainsi la possibilité de le faire en rappelant d'abord cette recommandation simple à nos concitoyens n'allait pas directement aux urgences, mais appeler d'abord le quinze si votre médecin traitant n'est pas disponible en ayant plus de professionnels de santé disponible avec des incitations dans les cabinets de ville ou les médecins qui ont pris des qui ont pris des patients adressés par le quinze pouvaient bénéficier d'une majoration de consultation de 15 euros à l'hôpital, en reconnaissant les contraintes de travail de nuit par le doublement des majorations pour les personnels soignants et une revalorisation de 50 % des gardes pour les médecins, nous évaluons actuellement les résultats de chacune de ses recommandations et souhaitons maintenir de façon durable, toutes les solutions qui auront fait leurs preuves. Parce que. Merci madame la ministre, la parole est à Madame Raymonde Poncet mon jeu pour le groupe écologiste territoire Merci madame la présidente, madame la Ministre, depuis la présentation de votre mission flash le moral des soignants, continue de baisser, selon l'enquête, oh Odoxa un quart des soignants travaillent plus de 45 heures par semaine, un quart pense en mauvaise santé à cause du travail et les soignants sont 2 fois plus nombreux à se voir prescrire un arrêt de travail pour stress que le reste de la population active, conditions de travail dégradées, manque de personnel et de lits, le 30 août à Strasbourg 50 patients se trouvait aux urgences pour seulement 30 places 50 % des lits d'hospitalisation d'urgence était fermé par manque de personnel, 26 personnes sont restées plus de 12 heures sur un brancard à attendre, et un homme âgé de 81 ans a attendu plus de 22 heures jusqu'à y mourir sur son brancard, ce drame a eu lieu malgré la politique de régulation que vous avez mis en place et qui a abouti à des grèves comme au CHU de Bordeaux où le personnel, soulignait que le problème n'est pas tant le flux de patients mais et les soignants qui manque dans son rapport d'évaluation de la mission flash le syndicat SAMU Urgences indiquait clairement que la non-dispose de débilité de lits d'aval des services d'urgence reste le problème principal de dysfonctionnement, conséquence, il faut ouvrir des le problème des urgences n'est pas principalement un problème de régulation mais de moyens d'attractivité des métiers à cet égard le PLFSS 2023 se montre malgré l'annonce de la fin des économies demandées toujours insuffisant, la Fédération hospitalière de France estime que l'augmentation de l'Ondam hospitalier et dès à présent, insuffisante pour absorber l'inflation le Ségur la revalorisation du point d'indice et le paiement des heures supplémentaires, elle ne permettra aucune embauche supplémentaire alors qu'il est crucial d'augmenter le ratio de 2 soignant par patient, ma question est donc : compte tenu de la PAC mécanique de ses coups que je viens d'évoquer, de l'avis de la F. H. F, envisagez-vous de réajuster à la hausse l'Ondam pour répondre enfin aux causes aux causes structurelles des difficultés de l'hôpital. je vais rappeler à tout le monde, de bien vouloir. Respecter son temps, même à 5 secondes parce que multiplier par tout le monde, ça fait quand même beaucoup à la fin, merci beaucoup, Madame la Ministre, vous avez là-bas. Madame la présidente, madame la sénatrice l'objectif national des dépenses d'assurance maladie Ondam vient apporter des finances en plus en apportant une progression par rapport au financement de l'année précédente pour l'Ondam 2023, aucune mesure d'économie ne repose sur l'hôpital, au contraire, les dépenses relatives aux établissements sont en hausse de plus 4 virgule un % dans l'Ondam 2023 soit 4 milliards d'euros supplémentaires par rapport au budget de l'année 2022, nous maintiendrons une attention particulière dans les prochaines années sur l'Ondam établissement pour porter des réformes d'organisation et une ambition d'excellence mais également pour garantir l'attractivité des métiers ce niveau dont armes lui permettra aussi de faire face à l'augmentation de l'inflation sur cette période avec un soutien financier aux professionnels de santé et un soutien aux établissements pour faire face à l'augmentation des charges hors rémunération des personnels, par ailleurs, pour soutenir les hôpitaux et ces personnels nous lançons dans le cadre d'une nation du Conseil national de la refondation enchanté un chantier pour me vivre à l'hôpital, qui aura vocation à aborder les sujets des conditions de travail, l'enjeu est de permettre aux soignants actuellement en exercice, de retrouver le sens de leur engagement pour qu'il reste en poste et que les jeunes et envie de rejoindre les établissements de santé, enfin le niveau de l'Ondam, en 2023 hé bien supérieur à celui que nous pouvions connaître précédemment l'Ondam, en 2016 étaient ainsi à 1 virgule 8 % et l'Ondam, en 2017 à 2 avec un Ondam 2023 à 3 sets hors dépenses de crise, nous investissons donc massivement dans notre système de santé. Si beaucoup la parole est à Madame Étienne Pumerole pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame le président, si ça vous dérange pas, parce que je m'appelle Émilienne. Franchement, je crois que je suis un tout petit peu fatigué parce que vraiment je n'oublie pas votre prénom Émilienne Pumerole. Merci madame la présidente, la Ministre, mes chers collègues. Beaucoup d'annonces beaucoup de consultations encore celle du CNR et en fait pas beaucoup de mesures structurelles pour répondre à la crise de l'accès aux soins en France et en particulier sur le problème des déserts en santé et pourtant l'organisation territoriale des soins représente un enjeu majeur pour répondre aux besoins aux besoins de santé de notre population, avec une nécessaire meilleure articulation des acteurs de ville et des acteurs hospitaliers la question cruciale de l'engagement de l'engorgement pardon des services hospitaliers est connue depuis longtemps, puisqu'on considère et tout le monde s'accorde à le dire qu'au moins 30 % % des patients qui arrivent à l'hôpital aurait pu être évité, il avait eu une régulation préalables effectivement qu'au fait, or depuis 2002 et la décision du ministre de Jean-François Mattéi, de supprimer l'obligation de garde des médecins libéraux, on observe une érosion permanente de cette permanence des soins, le volontariat n'est plus suffisant pour répondre à la demande de permanence des soins sur le territoire et cela est particulièrement avéré dans les déserts médicaux et ma collègue Laurence Cohen l'a évoqué tout à l'heure, à quand une PDSA obligatoire pour tous les médecins et pas simplement les médecins généralistes au regard de cette situation, vote au gouvernement, a mis en place cet été différente dispositif suite à une mission flash une énième mission demander au professeur Brown, comme si l'on Découvrez j'allais dire le problème de notre hôpital, face à des problèmes structurels vous répondiez encore et toujours par des mesures prises dans l'urgence, pour ne pas dire dans la précipitation et pour des objectifs à court terme, ma question va se centraliser sur un seul point petit focus sur le problème des mesures qui ont proposé une majoration pour les soins non programmés pour les actes effectués par les médecins généralistes après régulation, vous l'avez évoqué tout à l'heure quinze euros supplémentaires pour eux dans ce type de consultation malheureusement le cadre cette régulation inclut celle effectuée par SOS Médecins, mais si elle effectuée par les Pts ne paraissent pas l'être, ce qui paraît incompréhensible et c'est une notion doit donner MG France. Merci, cher collègue, merci, même la ministre. Madame la présidente, madame la sénatrice, nous avons souhaité encourager les médecins libéraux à prendre leur part à la prise en charge des soins non programmés cet été, pour cela, nous avons suivi la recommandation de la mission flash sur les urgences et soins non programmés, de créer une majoration en attribuant à titre dérogatoire et temporaire, un supplément de 15 euros pour tout a effectué par un médecin libéral à la demande de la régulation du SAMU sas pour un patient qui ne fait pas partie de sa patiente elle habituel cette majoration n'a été utilisé que par 4 % des généralistes libéraux pour un total d'environ 50000 actes, beaucoup de médecins généralistes nous ont cependant signalé qu'il prenait en charge des soins non programmés sans que ceux-ci ne soient nécessairement orientés par le SAMU ou les sas, nous sommes en train d'analyser ces données pour voir quel serait le meilleur schéma de financement des soins non programmés, je tiens à souligner la mobilisation des médecins libéraux qui se sont engagés cet été, dans beaucoup de territoires des organisations ont été montés par des libéraux pour permettre la prise en charge des soins non programmés, de manière temporaire pour soutenir le système hospitalier très attention cet été et cela a très bien fonctionné. Merci, la parole est à monsieur Olivier Henno pour le groupe Union centriste. Merci madame la présidente, madame la Ministre, lorsque nous abordons le sujet des urgences hospitalières et des soins non programmés, une question vient à l'esprit, comment en sommes-nous arrivés là, au-delà du constat, il nous faut apporter des réponses au problème et le problème, évidemment on tourne autour, hein, c'est le temps médical disponible pourtant une évidence, c'est avec du temps médical disponible qu'on assurera la bien-traitance des patients et que les personnels soignants retrouveront ce qui font de leur dévouement, apporter des soins dans des conditions dignes les dernières politiques publiques cherche à redonner du temps médical, le bouquet de solutions et de plus en plus large, mais dans le même temps l'accès aux médecins généralistes et de plus en plus difficile sur nos territoires et a fortiori les soirs et les week-end, notamment en province où le sentiment d'abandon du droit fondamental de l'accès à la santé pour tous se fait sentir dans son bilan de l'année 2021, l'Ordre des médecins disaient que le taux de participation globale des médecins généralistes à la permanence des soins ambulatoires et malheureusement reparti à la baisse, 36 pour 100 des territoires de permanence de soins sont couverts par moins de 10 de 10 médecins volontaires et 20 % des territoires de ces permanences sont couverts par moins de 5 médecins volontaires, c'est grave, pas loin de chez moi, nos amis belges ont mis en place une permanence de médecine générale sur le même site que leur accueil d'urgence avec un accès unique et un triage commun ainsi les urgences traite des urgences et les médecins généralistes traitent de ce qui est de leurs compétences, le suivi médical face à l'urgence, chacun doit prendre sa charge la méthode Madame la Ministre, pourrait être bénéfique puisque la santé des Français en dépend, et donc notre question est la suivante : le gouvernement entend-il soutenir l'ouverture de ce type d'unité dont les équipes seraient constituée de médecins généralistes volontaires, voire de réinstaurer l'obligation de garde des médecins généralistes pour assurer l'efficience de ses structures, je vous remercie. Merci madame la Ministre. Madame la présidente, monsieur le sénateur, nous avons assurément nous inspirer de bonnes pratiques mises en oeuvre dans nos pays voisins et et là on prend en l'occurrence la Belgique, c'est certain, les services des urgences en Wallonie repose souvent sur un modèle d'accueil par une infirmière dont les fonctions sont assez proches de l'infirmier organisateur de l'accueil, également en France, par ailleurs, la régulation des appels d'urgence en Belgique ne comprend pas de régulation médicale comme en France, or je crois que sur ce point, nous devons garder la plus-Value du système français qui associe des opérateurs dédiés les assistants de régulation médicale et la présence de médecins dans les centres de régulation malheureusement nos voisins belges sont confrontés aux mêmes problèmes que nous, avec les mêmes difficultés à recruter dans les hôpitaux et des taux d'absentéisme élevé, le gouvernement fédéral a adopté des mesures au mois de juillet 2022 destiné à contrer le manque de personnel soignant dans les hôpitaux, en favorisant la reprise d'activité de soignants, retraités, de même le ministre fédéral des Affaires sociales et de la santé publique de Belgique a annoncé au mois de juin un New Deal visant à réformer l'organisation de la médecine générale en Belgique, partant du constat qu'il y avait un nombre insuffisant de médecins généralistes en Belgique et qu'il fallait mais améliorer l'accessibilité aux patients, vous le voyez, nos voisins européens connaissent les mêmes difficultés que nous, ce n'est pas propre à la France, mais c'est en recherchant les bonnes initiatives dans nos territoires ou chez nos voisins que nous pourrons construire ensemble ensemble des solutions durables et pour la problématique de la permanence des soins, nous savons et nous sommes au moment où nous allons, entretenir et ouvrir la convention collective avec les médecins, pouvoir d'engager les sujets sur la responsabilité collective, c'est bien ensemble, que nous trouverons les solutions à ces problèmes. Merci, la parole est à Madame Florence là Sarah donc pour le groupe Les Républicains. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre système de santé connaît de fortes tensions dans un contexte de démographie médicale tendu qui un Pacs, notamment les services d'urgence ma question porte sur la crise des urgences en Gironde sur le territoire sud- Gironde les urgences vitales dépendent d'une seule équipe d'urgence celle d'urgence et du SMUR du centre hospitalier de Langon pendant toute la période estivale, ce service à assurer ses missions, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans fermer ses portes, une fois de plus, le service d'urgence, a tenu grâce aux professionnels de santé, malgré des conditions d'exercice très difficile cet investissement est liée à une équipe d'urgentistes, fidèle à l'esprit hospitalier invincible le système depuis plusieurs années, les internes du service, ils sont encadrés dans leurs apprentissages, le stage aux urgences de Langon et plaidé plébiscité par les internes de Gironde. Pour motiver les jeunes Inter les jeunes urgentiste à intégrer cet hôpital de périphérie, un plan d'accompagnement hospitalier, en effet, été élaboré, l'objectif est de leur faire découvrir cette médecine polyvalente exigeante et difficile sur un vaste territoire mais riche et intéressante, on est emporté par une solidarité d'équipe, or ces jeunes, spécialiste de la médecine d'urgence qui ont pourtant apprécié de venir travailler à Langon se tourne ensuite vers les centres hospitaliers voisins qui propose des contrats très lucratifs sur le long terme, monsieur le Ministre, Madame la Ministre, la situation des services d'urgences de l'hôpital de Langon, on n'est pas un cas isolé, il ne faudrait pas en arriver à la situation des urgences d'Arese sur le bassin d'Arcachon, qui viennent de fermer leurs portes pour un mois, faute de médecins aussi, Madame la Ministre : envisagez-vous une valorisation des gares, des urgentistes à la hauteur de l'engagement fourni et de leur activité à très haute responsabilité afin de maintenir et de consolider les services d'urgence dans les territoires périphériques, quelles sont vos propositions pour lutter contre le retour massif à l'intérim, dont le coût est prohibitif. Madame la présidente, madame la sénatrice, comme vous l'indiquez, le service des urgences de Langon à continuer à assurer ses missions 24 heures sur 24 et certains jours sur sept cents, fermer ses portes, il faut d'abord saluer l'engagement des soignants de cet établissement, pour faire le faire fonctionner concernant le sujet que vous évoquez de concurrence des rémunérations, l'ARS Nouvelle Aquitaine à analyser la situation, notamment après avoir pris connaissance des départs vers l'hôpital de Marmande, il ressort que cet hôpital de pratiques pas des conditions statutaires ou de rémunération dérogatoires à la réglementation, j'en profite aussi pour souligner le rôle remarquable du centre hospitalier de sud-Gironde cet été pour venir en appui des évacuations des populations dans le cadre des incendies massifs du département, le sujet de la rémunération et de la valorisation des gardes et bien sûr un des facteurs de reconnaissance à ce titre, les recommandations de la mission flash sur les urgences et les soins programmés ont reconnu pour la première fois la pénibilité du travail de nuit et mis en place pour 3 mois un doublement des indemnités de suggestions pour la nuit pour les personnels paramédicaux et une majoration de 50 % applicable aux personnels médicaux de manière plus globale, le Ministre de la Santé et de la prévention, a annoncé hier lors du lancement du CNR de la santé, l'ouverture d'un chantier au niveau national pour mieux vivre à l'hôpital, qui aura vocation à aborder ces sujets, des conditions de travail, créons les conditions pour que les soignants actuellement en exercice, retrouvent le sens de leur engagement pour que les jeunes se sentent accueillis dès la première heure de leurs études en santé dès le 1er jour de leur stage, qu'ils aient envie de rejoindre les établissements de santé, et que les plus expérimentés et envie d'y rester, enfin, s'agissant de la lutte contre les dérives de l'intérim, c'est un sujet majeur face à de telles pratiques, le risque est grand de fissurer profondément l'esprit d'équipe dans nos hôpitaux, la députée Stéphanie Rist apportées par la loi, l'encadrement des rémunérations, il est temps de la mettre en application, le ministre de la Santé a annoncé un calendrier à compter de printemps 2023, il ne sera plus possible de payer démesuré ne ment en intérimaire d'ici cette échéance, les situations à risques devront être identifiés dans les territoires, avec le concours des ARS et parce que les hôpitaux aussi nous le demande, il ne sera plus possible à la sortie de sa formation de soignants, de démarrer sur l'exercice professionnel par de l'intérim, c'est une des mesures qui a été inscrite dans le PLFSS pour 2023.

les personnels n'pas d'espoir d'amélioration de leurs conditions de travail, il est à craindre que l'hémorragie de démission à l'hôpital continue, ce qui entraînerait encore des fermetures de lits et de services à Morlaix par exemple entre arrêts de travail et postes non pourvus, ce sont les gardes et les remplacements qui sont difficilement assurés et cela malgré la sur-majoration des heures supplémentaires en oncologie, on fait des chimios thérapies dans les couloirs, les services sont en Bolivie, et les patients demeurent dans le service des urgences, même le retour à domicile et compromis face au manque d'ambulanciers, malgré cela, l'ARS, Bretagne, déclare le 21 septembre dernier dans un grand quotidien que l'été s'est globalement bien passé, quel mépris, quel déni de la réalité, 6 millions de Français n'ont pas accès à un médecin traitant 15000 personnes dans le Finistère, non pas de médecin référent, l'hôpital absorbe donc de plus en plus des soins non programmés et on annonce une baisse des médecins généralistes jusqu'en 2030, le système de santé dans son ensemble est à revoir, depuis la loi hôpital, patients, santé, territoires nous alertons Chancet sur la disparition de l'offre de soins dans les territoires, nous proposons, en vain, des solutions qui nécessairement devront être coercitive pour une offre de soin hospitalier et de médecine de ville au plus près des besoins réels, il ne doit plus y avoir de place pour les mercenaires de la médecine comme les appeler Madame Buzyn qui mettent à mal les Budgets des petits hôpitaux, du fait de leur exigences financières exorbitantes, madame la ministre, il y a urgence, quelle décision, penchez-vous prendre immédiatement pour les Françaises et les Français qui n'ont plus accès aux soins médicaux. Si Madame la Ministre. Madame

comme tous ici, après ces 4 mois de campagne qu'il y avait urgence à agir, il y a urgence à agir, pourquoi, parce que les décisions prises lors du dernier quinquennat sont des mesures du temps long et qu'elles ne produisent pas encore l'effet escompté, il y a urgence à agir, pourquoi, parce qu'après 2 ans de crise sanitaire, nous avons des personnels soignants qui sont épuisés, il y a urgence à agir, pourquoi, parce que nous vivons, nous vivons un phénomène sociétal où les profs et les nouveaux entrants sur le marché du travail, les nouveaux médecins ne souhaite plus travailler comme les médecins d'avant, un médecin qui part en retraite aujourd'hui, doit être remplacée par 3 médecins. Non, je ne pense pas raconter de conneries, madame, je suis désolé mais. Donc nous sommes, nous sommes vraiment sur une situation où l'urgence à agir, elle est là, nous travaillons depuis le mois de juillet avec les collectivités territoriales, avec les professionnels de santé, le CNR n'est pas un énième diagnostic, nous, nous proposons déjà dans le PLFSS des mesures je le, je le dis, il y a urgence à travailler ensemble pour sur les territoires, permettre à nos personnels

pour former des nouveaux médecins, donc nous allons avec les professionnels, avec l'évolution des formations, nous avons ouvert tous les sujets, laissez-nous encore quelques mois pour pouvoir répondre à ces sujets mais nous c'est ensemble, c'est pas le ministère de la santé tout seul qui des donnera des mesures qui s'appliqueront sur le territoire, elles devront s'adapter à chaque territoire. Merci monsieur fiché, vous avez 19 secondes. Oui, Madame la Ministre, merci pour votre réponse, pensez aux élus locaux, qui sont tous les jours, sollicité face à des administrés qui n'ont pas de réponses à leurs questions depuis 10 ans que je m'occupe de ces sujets, je peux vous dire que les réponses sont toujours les mêmes, des augmentations des stages mais jamais de vraies réponses dans les territoires où des administrés, non plus, aujourd'hui, de médecins, et ça c'est extrêmement grave, il y a urgence apporter de vraies réponses immédiatement. La parole est à monsieur Jean Sol pour le groupe Les Républicains. madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai 90 ans j'ai mal, j'attends au fond d'un couloir depuis 24 heures sur un brancard inconfortable que l'on Vienne me prendre en charge, mal, mal de savoir que ma grand-mère mon père, ma femme ou mon enfant souffre et d'attendre interminablement des nouvelles les concernant, j'ai mal de ne pas pouvoir gérer l'afflux de patients pouvant générer une perte de chance mal de voir mon serment d'Hippocrate bafouée par le poids des normes de la charge administrative et du manque de moyens humains, comme vous le savez, madame la ministre, une au service d'accueil des urgences, véritable vitrine des établissements sont en souffrance et c'est toute une chaîne d'hommes et de femmes qui en pâtissent, alors que l'accueil, la qualité et la sécurité de la prise en charge devrait naturellement s'imposer à tous, cependant, nous ne voyons pas dans nos territoires d'amélioration significative, je le regrette et la prévision démographiques en matière de vieillissement ne rassure pas sur les flux à prendre en charge dans un contexte de désertification médicale de médecine de ville essoufflé et de dégradation des conditions de travail cet été, le président de SAMU Urgences France nous a rappelé que c'était aussi le SMUR et le centre 15 qui était en grande difficulté de fonctionnement, le nombre de prises en charge aux urgences a doublé en 20 ans, passant de 10 à 20 millions j'interrogé ici-même Madame Buzyn en 2018 sur l'ensemble de ses préoccupations, mais aujourd'hui encore, les mêmes problèmes remontent non seulement du terrain mais aussi des enquêtes le SAMU Urgences France pointait en effet récemment l'insuffisance de lits d'aval et de SSR, la fermeture de certains services d'urgence ou les inquiétants départs en masse de nos soignants alors Madame la Ministre, qu'allez-vous faire pour éviter la fuite de nos personnels personnel qui sont épuisés depuis la crise sanitaire pendant laquelle ils ont tout donné, qu'allez-vous faire pour lutter contre la désertification médicale qui Majour langage d'engorgement aux urgences, qu'allez-vous faire pour mettre en fait en adéquation les rémunérations, avec un niveau de formation et les diplômes tout le personnel soignant. Madame la présidente, monsieur le sénateur. Nous avons tous mal à notre système de santé, c'est bien pour ça que nous y travaillons tous et que nous allons devoir y travailler tous ensemble, tout d'abord, dans le cadre du CNR en santé, je l'ai déjà dit le groupe de travail mieux vivre à l'hôpital c'est bien : comment accompagner nos personnels soignants accompagner l'attractivité des métiers pour redonner du sens, 2 ans de crise sanitaire dire, j'allais dire de d'accélérer le process d'un système de santé qui ne va pas, qui ne va pas bien, maintenant, vous l'avez dit vous-même, un médecin, je le redis, un médecin, c'est ses 10 ans nous avons supprimer le numerus clausus, il y a maintenant 2 ans, il était effectif, il faut 10 ans pour former un médecin en attendant que faisons-nous pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens, il nous faut dégager du temps médical, c'est le sens des mesures qui sont prises, notamment avec le déploiement des assistants médicaux, il nous faut améliorer les processus de coopération entre tous les professionnels, c'est bien ce qui est fait, notamment dans le cadre des C Pts il nous faut enfin rayon chantier tous les métiers de la santé et les rendre attractif, c'est le sens du chantier que nous allons ouvrir avec mes collègues sur les formations, les formations initiales, mais aussi les formations continues de toutes les professions et non pas uniquement de celle des médecins généralistes, nous le savons tous notre Sosthène de santé ne va pas bien, il ne va pas bien uniquement depuis 2022, c'est la conséquence je peut être d'une faillite collective depuis des années maintenant, il nous faut nous mettre tous ensemble, les élus, et c'est bien pour ça que mon ministère par le nom d'organisation territoriale et c'est bien avec les élus, avec les professionnels, avec les usagers que nous allons pouvoir répondre aux solutions en organes en s'organisant de façon territoriale et apporter des réponses, territoire par territoire. Merci, la parole est à monsieur Bruno Belin pour le groupe Les Républicains. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, par votre expérience et votre engagement, vous savez. La réalité des souffrances. Des désespérances dans nos urgences des attentes aussi des peines vous savez aussi, la réalité des lits fermés, rien que dans l'hôpital Poitiers dans le département, je suis élu 271 lits fermés cet été, d'ailleurs, à mon avis, il faudra que vous nous disiez la réalité du nombre de lits fermés depuis quelques années, vous savez, la désespérance aussi des territoires qui se sentent abandonnés, tous ces hôpitaux de proximité sur les territoires où on a l'impression que les politiques de santé sont désertées dans le département où je suis élu, pardon, de prendre des exemples que je connais le moins mal à Loudun ou Montmorillon il y a plus de services d'urgence, alors vous savez, la différence entre urgence ou soins non programmés, elle est compliqué quand vous qui avez quelqu'un qui vient effectivement souffrance un dimanche, il attend une réponse, hé bien dans ces territoires, là il n'y en a pas, et on est face à cette aberration alors moi, ma question elle est simple et tient en 5 mots, quelle est votre stratégie territoriale, que comptez-vous faire sur ces territoires que vous avez oublié et quand et comment vous allez répondre sur ces territoires avec les suites de la mission flash et dans quel calendrier, quel est votre stratégie territoriale Madame la Ministre. Madame la présidente qu'avant. L'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine qui tient des réunions territoriale hebdomadaires pour assurer un suivi resserré détention hospitalière en lien avec la préfecture du CHU de Poitiers, face aux tensions hospitalières rencontrés par le CHU engendre une diminution des effectifs de l'équipe territoriale d'urgence qui fonctionne sur les 4 sites. Je tiens à souligner que le CHU de Poitiers, tout particulièrement mobilisés pour la recherche des professionnels de santé les urgences de Loudun et de Montmorillon, que vous avez cité font l'objet d'un suivi et d'une vigilance toute particulière pour limiter au maximum les garde non couvertes et organiser un accès régulé des patients dans les 2 sites, l'accueil des patients est organisée de la manière suivante : quand les gardes ne peuvent être couvertes, la régulation est assurée par le quinze et la population est informée de la nécessité de ne pas se rendre aux urgences, mais d'appeler le 15 sur site, si une personne se présente un accueil est organisé par une infirmière qui sollicitent le quinze pour déterminer la réorientation à effectuer, orientation vers Poitiers ou une autre structure hospitalière renvoie vers le médecin traitant ou programmation d'une consultation le lendemain. Pour vous répondre précisément à votre question. Cher ancien confrère. Vous dire que j'étais dimanche face aux maires ruraux face aux maires ruraux, donc les territoires ne sont pas oubliés, je le redis, si le ministère dont j'ai le nord d'avoir la charge, c'est bien parce que la conscience, elle est prise que les elle est prise que les solutions, elle ne se décrète pas uniquement de la rue de la rue Duquesne et applicable dans les territoires, c'est bien avec les élus, avec les territoires avec le collectivités et avec les professionnels de santé que nous allons répondre et trouver les solutions pour répondre aux besoins de santé, ça n'est pas la solution qui serait valable dans votre commune ne serait pas valable au Havre à Montpellier ou à Marseille, les problématiques, elles sont différentes, les situations, elles sont différentes, donc c'est bien du travail, territoire par territoire que nous avons commencé à faire, c'est bien le sens de nos déplacements au Ministre Brown et au miens dans vos territoires pour venir à votre rencontre pour voir quelles sont les solutions qui fonctionne aussi celles qui ne fonctionne pas et comprendre pourquoi elle ne fonctionne pas. Merci madame la Ministre. Monsieur Beulin, vous avez 40 secondes. Merci madame la présidente, madame la Ministre. Ma chère consoeur fait de ces hôpitaux de proximité. Une chance est une priorité, il dont le ressenti d'être victime d'un délestage, or c'est un non-sens, c'est un non-sens d'abord vous même, vous l'avez dit son rayon réorienter vers voilà tel CHU, c'est un non-sens parce que c'est un non-sens écologique, on est dans une stratégie bas-carbone on met les gens sur les routes, ça bloque des pompiers, c'est un non-sens aussi territoriale parce qu'on a des coquilles vides dans des hôpitaux de proximité. Et puis, c'est un non-sens, surtout en termes de santé parce que, de la perte de temps, c'est de la perte de chance merci madame la présidente.

monsieur le sénateur. L'enjeu des hôpitaux de proximité des hôpitaux périphériques, il est pour moi essentiel, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu des formations et de l'évolution des formations, elle est primordiale. On va y arriver si nous pouvons aussi faire en sorte que nos interne qui se forment, ne fassent pas tout leur stage dans les CHU qu'puisse aller faire leur stage dans les hôpitaux périphériques dans les hôpitaux de proximité, c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler, je n'ai pas le. Voilà, c'est pas facile de tout vous expliquer ce chantier, il est ouvert, mettons les interne devant laisser dans les hôpitaux de proximité et dans les hôpitaux de périphérie et que un bon nombre d'entre eux pourront après s'y installer et on évitera ce genre d'écueil ce genre de situation. Chiche, Madame la Ministre, alors je vous attends dans les territoires ruraux dont vous venez de parler parce que vous verrez si moi je veux bien qu'on lui fasse des stages, il faut qu'encore qu'il y ait des maîtres de stage, faut encore qu'il des médecins pour former, on va pas à prendre en Irlande, en Iran, donc je vous attends dans les meilleurs délais sur les territoires ruraux dans ces hôpitaux de proximité pour que vous veniez voir la réalité, merci madame la présidente. D'un prix merci, la parole est à Madame Sylvia de Noël pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, avec plus de 20 millions de passages par an, les urgences de nos hôpitaux sont engorgés au plus haut point, confronté à un double effet ciseaux : d'une part, la pénurie de soignants plus grave que jamais et une forte augmentation du recours aux urgences pour nos compatriotes en effet pour des millions de Français, le recours aux urgences, c'est une absolue nécessité, faute de pouvoir bénéficier des services d'un médecin traitant, la médecine de ville ne sont plus aujourd'hui en capacité de remplir de façon efficiente, son rôle de soins de 1er recours souffrant d'un maillage déséquilibré un complet de l'ensemble du territoire face à cette situation préoccupante, j'aurais souhaité vous entende sur 2 propositions : d'une part une participation plus large des médecins libéraux à la permanence des soins via les ces puisque cette permanence repose aujourd'hui essentiellement sur les hôpitaux s'agissant des week- end et des jours fériés, d'autre part, une réforme de la libre installation des médecins généralistes est elle partie des pistes envisagées par le gouvernement pour tenter de lutter contre les déserts médicaux et remédier à l'inégale répartition des médecins généralistes, je vous remercie. Merci madame la ministre. Madame la présidente, madame la sénatrice répondra à vos 2 points tout d'abord sur la permanence des soins, nous devons améliorer la situation de la permanence des soins ça déjà été dit plusieurs fois, la permanence des soins est une mission de service public et elle doit être assurée partout sur le territoire, nous souhaitons placer les médecins en situation de responsabilité collective sur la question de la permanence des soins pour ça, il y a 2 solutions : soit les professionnels de santé s'organisent par eux-mêmes et remplissent entre le tableau de garde selon les contraintes là où il y a une ces BTS, cela peut être le bon échelon pour organiser cette permanence, soit il y a défaut de couverture et l'État devra prévoir une organisation pour assurer aux Françaises et aux Français, un accès à des soins non programmés en soirée le week-end, le code de la santé publique prévoit déjà la possibilité de réquisitionner des médecins en cas de défaillance sur la libre installation la libre installation beaucoup demandent à ce qu'on revienne dessus, on nous répète par exemple qu'on contraint bien les enseignants à aller partout sur le territoire d'une part je trouve que cette comparaison ne fonctionne pas et, d'autre part, je ne crois pas à l'efficacité de l'obligation, notre objectif, c'est d'inciter plus fortement et même de convaincre nos territoires sous-dotés mérite des médecins qui s'y installe volontairement et qui s'y investissent oui nous devons travailler à d'autres modalités modalités d'installation des médecins sur le territoire, nous y travaillons d'ailleurs dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, en prévoyant un nouveau dispositif simplifié en matière d'aide à l'installation et concertée dans le cadre d'un comité local d'association, les représentants des élus locaux, les professionnels de santé et les administrations. Merci madame Noël vous avez. 53 secondes merci madame la Ministre pour vos réponses, j'aimerais aborder à présent le le la seconde partie de mon intervention, qui concerne la pénurie de soignants, les causes sont diverses, nombreuses et ancienne et les réponses à cette problématique sont tout aussi complexe et multiple, il met cependant impossible de ne pas profiter de ce temps de parole pour à nouveau vous sensibiliser sur la réintégration des milliers de soignants et pompiers suspendus ou interdits d'exercice depuis plus d'un an maintenant dans notre pays, cette situation n'est plus tenable la quasi-totalité des pays ont abandonné cette mesure vous laisser même aujourd'hui aux soignants la libre-choix de recourir au nouveau vaccin contre la Covid 19 dans ces circonstances, le maintien de cette mesure est incompréhensible et relève davantage de la punition et de l'obstination que de la justification sanitaire notre système de santé est à l'agonie, nous ne pouvons plus nous passer du moindre soignant, ma question est simple : quand envisagez-vous de lever cette mesure, qui engendre un peu plus de dysfonctionnements et d'engorgement Même les ministres, vous souhaitez répondre. Sinon normalement une réplique. ça concerne la la question au au départ, en fait, hein, c'est pas de séparer la question en 2 voilà, Madame la Ministre, vous avez une mine. Merci madame la présidente, madame la sénatrice. Je veux dire à celles et ceux qui pensent que c'est une réponse miracle là pour répondre aux problèmes d'effectifs de l'hôpital, qu'ils se trompent, il faut dire, cela concerne quelques centaines de personnes sur plus de 300000 soignants qui ont donc refusé de se protéger, pour protéger les autres, ce que je préfère retenir, c'est le sens citoyen et l'éthique des professionnels de santé qui sont au contact des Français les plus fragiles, il faut rendre hommage à tous les professionnels mobilisés qui ont accompli leur devoir avec courage les avis du conseil scientifique de la Haute autorité de santé ont été rendus et ils sont favorables au maintien de l'obligation de vaccination contre la Covid 19 des personnels exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux, nous avons toujours géré cette crise, en nous basant sur les recommandations des scientifiques, et ce n'est pas aujourd'hui que cela va changer. Madame Noël, vous avez une minute pour répondre. il faut quand même savoir qu'il y a aujourd'hui aussi des étudiants en médecine qui sont suspendus demain vous vous vous vous vous permettez pas d'aborder dignement les enjeux de l'hôpital en terme d'effectifs en maintenant cette mesure, je vous donne un exemple dans mon, dans mon département, de la Haute-Savoie, la plupart des soignants partent en Suisse, parce que cette obligation vaccinale, elle a été levé et ça fait encore un argument de plus pour ses soignants pour partir, donc moi, franchement, il faut qu'on m'explique quel est aujourd'hui le sens du maintien de cette mesure. Merci, la parole est à monsieur Laurent Somon pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la Ministre, la situation de notre système de santé avec les fermetures de lits et de celle des urgences en particulier n'ont jamais été aussi préoccupante en France, notamment 2 raisons majeures ressortent des différents constats rapport mission flash tout d'abord l'attractivité des cas des carrières médicales hospitalières en dépit du de la réforme du statut unique en effet l'équité de temps et de rémunération au sein d'un même service n'est toujours pas une réalité demi-journée de travail temps continue seuil du statut unique plages additionnelles activités mixtes et activité libérale intra-hospitalière recours à l'intérim, autant d'occasions pour un même service de faire cohabiter des rémunérations des rémunérations disparates et d'aggraver les tensions, c'est le sentiment d'appartenance à une équipe médicale solidaire qui peut faire accepter les difficultés inhérentes à la profession, en Hauts-de-France les effectifs par vers la Belgique ou le Luxembourg, que comptez-vous mettre en place pour redonner ce sens à ces professionnels, ensuite, la deuxième, c'est la gestion des des causes majeures des de la gestion des flux des urgences questions inhérentes à la pénibilité et au sens de l'activité, comment le gouvernement permet de le décloisonnement entre la médecine de ville et l'hôpital général avec l'objectif de fluidifier le parcours de soins des Français et de désengorger les urgences à côté des grands CHU, les hôpitaux de proximité, comme ça a été dit, la médecine de ville doivent être organisés pour assurer le même service à une patiente, elle le l'urgence en milieu rural ou pour des populations souvent sans ressources, ce qui est possible aux urgences comme le tiers payant doit être vrai et faciliter en première ligne, quel dispositif d'implantation des praticiens en ville mettait près prévoyez-vous en l'état actuel, les personnels qui ont quitté le secteur de la santé ne sont pas près d'y revenir, allons, ne pouvoir arrêter l'hémorragie en réactivant la médecine de ville, avec le retour et le soutien aux gardes et des soutiens aux installations obligatoire ou pas en ville, y compris pour les Ehpad parce que les services d'urgence en restreignant leur accès faute de personnel, seuls, en tout cas le cas dans la Somme. Madame la présidente, monsieur le sénateur, la réforme du statut unique poursuit hé bien l'objectif que vous décrivez, pour amener davantage de cohésion au sein d'un même service pour autant les conditions d'exercice et les suggestions demeure hétérogène est-il nécessaire de pouvoir reconnaître les situations individuelles, de même le recours à des professionnels de santé libéraux a pour objectif de renforcer des équipes qui sont confrontés à de fortes difficultés de recrutement, les professionnels de santé libéraux qui sont intervenus dans les établissements ont conservé les charges de leur cabinet en parallèle et de leur activité hospitalière pour favoriser leur engagement il était justifié de pouvoir les indemniser de manière appropriée. Concernant l'intérêt nous avons tracé un chemin nous allons appliquer la loi risque d'ici le printemps 2023, l'encadrement des rémunérations de même comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne sera plus possible à la sortie de sa formation de soignants, de démarrer son exercice professionnel par de l'intérim, c'est une mesure du PLFSS pour 2023 concernant votre 2ème question : vous avez raison : une partie du flux des urgences peut être prise en charge si on fluidifie la réponse aux soins non programmés en ville, c'est l'objet du service d'accès aux soins qui se déploie progressivement sur le territoire national, nous devons accélérer sa mise en place, il a vocation à pouvoir aider les citoyens à s'orienter dans notre système de santé le patient pourra ainsi bénéficier d'une orientation vers la réponse la plus adaptée à son besoin de santé. Pour compléter ce schéma, nous devions mieux partager la réponse aux soins non programmés entre l'ensemble des professionnels de santé, c'est la logique des transferts de compétences, les ordres professionnels sont en train de travailler à ces sujets et doivent nous faire très vite des propositions c'est collectivement avec les médecins, les infirmiers et les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les autres professionnels que nous pouvons contribuer à mieux répondre aux soins non programmés.

Voilà cher président. Alors pour conclure le le débat, la parole est à madame la présidente, Catherine Deroche pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre groupe, les républicains, a choisi d'inscrire ce débat sur les urgences hospitalières et les soins non programmés à l'ouverture de cette nouvelle session et je m'en félicite, après avoir décidé la crème à la création d'une commission d'enquête sur l'hôpital, que j'ai rapporté au début de cette année, cela montre bien la volonté du Sénat au-delà du travail de la commission des affaires sociales de ne jamais relâcher l'attention portée à notre système de santé René-Paul Savary, il a souligné en introduction la ville comme l'hôpital, traverse une crise profonde et les réponses doivent être rapide, comme plusieurs collègues l'ont rappelé ce débat vient aussi après un été, que nous redoutions pour les services d'urgence à l'hôpital ou un risque de rupture d'accès aux soins étaient bien avancés par de nombreux professionnels de santé, si la situation a bien été difficile et beaucoup en ont témoigné et a conduit de grands établissements hospitaliers à des mesures de régulation stricte à l'accès de leurs services, l'hôpital a néanmoins une nouvelle fois tenu une nouvelle fois, mais à quel prix, ce que nous voyons, c'est une succession ininterrompue de périodes de tension sur différents secteurs hospitaliers, ce que nous voyons c'est la survenue continue de crise dans les crises à l'été sur les urgences hospitalières et les maternités aujourd'hui sur la réanimation pédiatrique en Île-de-France et ce, alors que la crise Covid dont on ne parle presque plus, a toujours un impact sensible sur l'hôpital, quelles conséquences des risques immédiats pour la sécurité des patients dans leur prise en charge des soins parfois assuré sur un mode dégradé des retards d'accès aux soins et donc des pertes de chance mais surtout à moyen terme, comme un court terme des conséquences majeures sur l'état de l'hôpital et la situation des soignants, car ces crises successives ne font que renforcer l'épuisement des équipes appelées à se mobiliser toujours plus, elles ne font que renforcer les départs de médecins et d'infirmiers et fragilise donc encore notre système, l'hôpital a tenu, mais jusqu'à quand mon intervention en conclusion, on va se concentrer sur l'avenir, madame la Ministre votre ministre de tutelle aussi l'auteur d'un rapport, celui de la mission flash sur les urgences qui devait nous permettent, selon l'expression du moment, de sauver l'été 41 mesure dans la mise en oeuvre inégale s'est surtout faite par voie réglementaire, même quand elle relevait du domaine de la loi, mais force est de constater, à la fin de cet été, que nous peinons à trouver dans votre feuille de route des mesures pour prendre le relais de ces mesures d'urgence, vous l'avez un peu évoqué mais la régulation de l'accès aux urgences vers le quinze sera-t-elle par exemple généraliser pérenniser, quel sera le tarif durable des consultations de médecine générale le soir et le week-end, j'entends bien que la convention médicale qui sera négocié sera l'occasion de discuter des conditions de revalorisation de la permanence des soins ambulatoires, une négociation longue pilotée par l'assurance maladie mais qui échappe disons-le pour partie au gouvernement, mais surtout au Parlement qui ne peut en prescrire le cadrage, j'attends que désormais nous sommes aussi suspendu à de nouvelles concertations conférence des parties prenantes, Conseil national de la révélation de la refondation avec un volet CNR santé encore des discussions dans les soignants sont fatigués pour des conclusions dont on peine attendent une originalité quelconque on concerte, on concert et pendant ce temps, disons-le, on n'agit pas et puis soyons lucides pendant concerne on ne parle pas de financement, or il y a bien un enjeu financier qui n'a pas non plus être traité, Madame la Ministre, nous ne savons pas et nous le Parlement, le droit de savoir combien ont coûté les mesures urgence du plan Brown cet été, bien sûr nous ne regardons pas à la dépense quand il s'agit de la santé des Français, répond-on souvent et alors que nous allons examiner le mois prochain le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, il est de notre rôle aussi en tant que parlementaire, de vérifier que les moyens alloués à la politique de santé sont bien en adéquation avec les besoins, alors que la loi de programmation des finances publiques prévoit une main des rations de la progression de l'Ondam inférieure à la croissance du PIB à l'horizon 2027, il y a là matière à s'interroger, je constate par ailleurs qu'après cet été aussi aucune mesure relative aux urgences, aux soins non programmés ne figure au Plfss pour 2023 à penser donc aucune des mesures visant à renforcer la prise en charge en ville, la structuration des maisons médicales de garde les téléconsultations ou l'orientation des patients ne seraient

prenant acte de vos mesures dérogatoires, Madame la Ministre, nous avions un tulle télé le rapport de la commission d'enquête sur l'hôpital, sortir des urgences, nous revendiquons au Sénat, pas sur les seuls bancs des républicains mais très largement dans cette assemblée, la nécessité de laisser l'hôpital respirer en lui donnant des moyens clair et durable, sortir des urgences, cela voulait dire qu'on envie comme à l'hôpital, les conditions étaient donnés pour assurer correctement les soins programmés anticiper au mieux les soins non programmés en ville comme à l'hôpital cela voulait dire marquer la reine de l'enchaînement de crise qui ne permettent pas aux soignants de faire leur travail dans de bonnes conditions pour les patients comme pour eux, or je le regrette, je ne vois pas l'ouverture de cette session le chemin que le gouvernement entend proposer sur ce point, je vous remercie même la présidente. Alors je Alors je vais suspendre la séance pour quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour, la séance est suspendue.

La séance est reprise, l'ordre du jour appelle le débat sur la prise en compte des territoires, des savoir-faire et des cultures dans l'élaboration de réglementation européenne d'harmonisation. je vous rappelle que dans ce débat, le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de 2 minutes et l'orateur du disposera alors à son tour du droit de répartis pour une minute madame la Ministre, vous pourrez donc, si vous le souhaitez répondre après chaque orateur, une fois que celui-ci aura retrouvé sa place dans l'hémicycle, la parole et tout d'abord à l'orateur de la commission qui a demandé ce débat et je donne la parole donc à messieurs Jean-François Rapin, président de la commission des Affaires européennes pour huit minutes Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, Union européenne respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du Patrimoine culturel européen cet impératif fixé par l'article 3 du traité sur l'Union européenne trouve une résonance à l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union européenne contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leurs diversités nationales et régionales, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun, elle tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions des traités afin notamment de respecter et promouvoir la diversité de ces cultures cette exigence n'est pas ignorée par l'Union européenne mais elle est parfois négligé, notamment dans l'élaboration des règles d'harmonisation et plusieurs cas récents ont conduit la commission des Affaires européennes, que j'ai l'honneur de présider à solliciter l'organisation de ce débat afin de mieux apprécier l'ampleur de tels dysfonctionnements et de tenter d'en d'en identifier l'origine, l'Union européenne s'emploie assurément à prendre en compte la richesse que constitue son Patrimoine culturel, matériel et immatériel, l'objet de notre débat de ce jour n'est pas de faire le bilan de l'action qu'elle mène en ce domaine au printemps dernier la commission des Affaires européennes a d'ailleurs adopté à ce sujet, le rapport que lui ont présenté nos collègues Catherine Morin-Desailly et Louis-Jean de Nicolaï et qui appelle de ses voeux une stratégie européenne encore plus ambitieuse pour le Patrimoine, éléments d'identité, facteur d'enracinement, mais aussi puissant levier d'attractivité de développement durable et de cohésion pour nos territoires. qu'elle apprend en même temps qu'elle approfondisse et l'intégration de son marché intérieur, l'Union européenne se doter des moyens de protéger les dénominations des produits pour lesquels il existe un lien intrinsèque entre leurs qualités ou leurs caractéristiques et leur origine géographique divers produits agricoles denrées alimentaires et 20 européens sont aujourd'hui protégés par des appellations d'origine protégée, les AOP ou des indications géographiques protégées les IGP, l'Union européenne s'apprête même à étendre le Champ de cette protection puisqu'en avril dernier la Commission a proposé un tout 1er cadre réglementaire visant à protéger la propriété intellectuelle des produits artisanaux et industriels reposant sur l'originalité et l'authenticité des pratiques traditionnelles de leur région, ce cadre s'appliquera à des produits tels que la porcelaine de Limoges ou le verre de Murano ainsi la protection européenne pourra bientôt bénéficier à des savoir-faire, donc au Patrimoine immatériel de nos territoires, comme le fait valoir la Commission ce règlement aidera à promouvoir à attirer à préserver les compétences et les emplois dans les régions européennes, contribuant ainsi à leur développement économique, jusqu'à l'international. Si elle témoigne ainsi de son intention, culture et savoir faire locaux l'Union semble toutefois les ignorer, parfois brutalement la tension de la commission des Affaires européennes a été attiré ces derniers mois sur 2 exemples frappants, illustrant tous de les dangers d'une harmonisation aveugle des réglementations qui fonde le marché intérieur en mai dernier notre collègue Jean Michel Arnaud, lui, a ainsi soumis une proposition de résolution européenne que notre commission a adopté et qui est devenu résolution du Sénat le 5 juillet 2022 pour alerter sur le risque que faisait courir aux producteurs de lavande, la prochaine révision de de règlements européens d'une part le règlement Reach qui tend depuis 2006 à sécuriser l'utilisation des substances chimiques, il oblige à cet effet des fabricants à fournir des informations sur les propriétés toxicologiques, éco-toxicologiques des substances à commercialiser tout en justifiant de mesures de gestion des risques adaptées à leurs usages, d'autre part, le règlement dit CLP datant de 2008 qui porte quant à lui sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances permettant que les dangers correspondants soient correctement identifié par les consommateurs dans le cadre de la transition environnementale en cours, la Commission européenne engagé récemment un processus de révision de ces règlements pour en accroître le niveau d'exigence jusqu'à faire craindre aux producteurs de lavande, de devoir faire bientôt évaluer chacune des composantes des huiles essentielles et non le produit dans son ensemble, les coûts induits et les risques en terme d'image des civils essentiel de lavande menacerait alors toute la filière, c'est-à-dire des emplois mais aussi un savoir-faire et une culture prisé jusqu'en Amérique, Madame la Ministre, puisque même le Wall Street Journal a fait écho de nos préoccupations exprimées au Sénat dans cette résolution européenne en juin, c'était notre collègue Vanina Paoli-Gagin qui déposait une proposition de résolution européenne visant, pour sa part à préserver l'activité des vitrailliste très inquiets d'une prochaine interdiction du plomb susceptible de survenir, elle aussi, lors de la prochaine révision révision du règlement Reach, sous l'impulsion de l'argent, l'Agence chimique européenne, la commission des Affaires européennes a également adopté ce texte, elle en a même étendu la portée, puisque l'enjeu est partagé par de nombreux autres métiers du Patrimoine comme les facteurs d'orgues, pour qui l'usage du plan est une substance présentant les propriétés des propriétés sans équivalent est une condition de survie. Ces résolutions européennes ont tiré la sonnette d'alarme et sont en voie d'envoyer un une mécanique européenne d'harmonisation réglementaire dont nous ne contestons pas les objectifs, mais qui, faute de prendre en compte l'impact local entretient l'image d'une Europe en résumant une à une, se résumant dès la fin de ce mois, je me rendrai à Bruxelles avec les rapporteurs pour sensibiliser le cabinet du commissaire Thierry Breton et m'assurer que la commission proposera les adaptations utiles pour éviter le pire, mais la question reste entière comment empêcher de tels dérapages il est manifeste pas périlleux de laisser les cinquante-quatre agences que compte l'Union européenne ou même la Commission européenne par le biais d'acte d'exécution ou d'actes délégué régler les questions qui sont des de des, des éléments techniques sont hautement sensible sur le terrain, en effet, les procédures de révision des règlements européens concernés échappe au contrôle des Parlements nationaux, auquel seuls les propositions d'actes de nature législative sont transmises pour vérifier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité heureusement, mes chers collègues, notre enracinement local nous permet de jouer le rôle de lanceur d'alerte, ce faisant, nous sommes au service des territoires, mais également, indirectement, de l'Union européenne en lui évitant de commettre l'irréparable, par méconnaissance des savoir-faire et des cultures locales, j'y vois Madame la ministre, une démonstration évidente du rôle des Parlements nationaux et de l'intérêt que l'Union européenne trouverait à mieux les reconnaître, c'est une convention devait prendre le relais de la conférence sur l'avenir de l'Europe et entreprendre une révision des traités, elle ne devra pas l'ignorer, telle est selon moi le filigrane qui se lit derrière notre débat de ce jour, l'Union européenne ne saurait durer 100 renforcer le contrôle démocratique de son action, je vous remercie. Merci beaucoup monsieur le président, dans la suite. Que du débat, la parole est à monsieur Lucien stationnent pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour cinq minutes pardon Madame la ministre veut répondre. Oui, d'accord ici. merci, madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires européennes, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est évidemment un honneur pour moi de pouvoir participer à un débat au sein de cet hémicycle sur un thème de je mesure pleinement l'importance puisqu'il touche à la prise en compte des territoires dans l'élaboration des réglementations européennes et comme vous l'avez souligné cette prise en compte est essentiel car les territoires, ce sont avant tout des citoyens qui les habite et des cultures locales qui les anime. Et j'en ai conscience vous l'avez mentionné, beaucoup de nos concitoyens peuvent avoir l'impression que l'échelon européen est trop éloignée ou trop large pour saisir les spécificités de leur environnement quotidien et l'objectif même d'une harmonisation des normes peut paraître aller à l'encontre de la diversité des territoires, des cultures et des pratiques et c'est pour cela que les procédures d'élaboration de la réglementation européenne intègre des échelons nationaux, régionaux et locaux, c'est une exigence démocratique, mais c'est également une condition essentielle pour que les réglementations soient pertinentes et efficaces et, surtout, et je crois que c'est important de garder cet élément en tête, l'Union européenne protège nos territoires souvent elle constitue l'échelon le plus adapté pour en assurer la défense, notamment face à la concurrence internationale. L'harmonisation des normes qui ne doit pas conduire à une uniformisation des cultures et des produits est une condition en revanche indispensable pour que l'excellence de nos savoir-faire locaux puisse rayonner au sein de l'Union européenne, mais également à l'international, c'est ainsi que, grâce aux négociateurs européen depuis 2017 les appellations jambon de Bayonne Brie de Meaux reblochon piment d'Espelette et j'en passe, hein, et son protégé à l'international. Bien sûr, tout ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir, à juste titre des inquiétudes quant à certaines règles européennes, qu'elle soit ou comme vous l'avez dit en préparation. Et lorsqu'un effet collatéral d'une réglementation européenne est avérée ou anticiper sur nos productions locales, nous devons tous collectivement faire un maire pour le corriger, il faut conclure madame la Ministre, absolument, je voulais juste ajouter que le gouvernement est pleinement mobilisé sur les différents dossiers que vous avez identifié et que je salue votre rôle de vigile dans ce domaine, merci. Merci monsieur 100 Dieu, vous avez la parole et toutes mes excuses. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la filière lavande et la Vendée, constituent un sujet particulièrement propice pour alimenter la discussion et fournir des exemples variés de difficultés avec la réglementation européenne, en effet, l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence est le révélateur de l'inadaptation des réglementations européennes par l'absence de prise en compte des difficultés des territoires historiques de production des savoir-faire et des cultures traditionnelles, cette présentation se déroulera à 2 voies avec ma collègue Marie-Pierre Monier, ici présente, point n'est besoin de rappeler les enjeux nationaux agricole, économique, touristique patrimoniaux énergétique. et du maintien de l'emploi mais aussi climatique de l'aménagement du territoire autour de l'huile essentiel de lavande, la France est le pays leader mondial du point de vue de la production de l'essence de la Vanda et occupe la seconde place en matière de d'essence de lavande, ces productions sont concentrées sur 3 départements du Sud-Est de la France, le Vaucluse, la Drôme, les Alpes, d'autres Provence qui comptabilise 87 % des superficies ces productions emblématiques de la province sont créatrices de valeur ajoutée dans le département de Vaucluse, qui comprend notamment les contreforts du mont Ventoux, j'ai été alerté dès le mois d'août 2021 par les maires, les agriculteurs et distillateurs de la Vendée, la de la crise économique majeure que la la que traverse la filière en raison de la très forte baisse des cours, moins 60 % en 3 ans, engendrée par une surproduction importante par un doublement des surfaces plantées en dehors des zones historiques de cette culture, en particulier dans l'image, l'immense plaine de la Beauce, les coûts de l'énergie sont venus s'ajouter à cette situation, ainsi que les aléas climatiques telles que le gel, puis la sécheresse et le manque d'eau cet été et la prolifération d'un ravageur la Cissé Domi, pour lesquels il est urgent d'agir, nous pilotant avec la sénatrice Monnier et moi-même, une série d'actions, permettez-moi d'attirer votre attention sur la lutte sanitaire nécessaire pour la filière l'avoir Nicole alors que le gouvernement a toujours martelé le message qu'il n'y aurait pas d'interdiction de produits phytosanitaires, actif ne les solutions n'était pas trouvé, nous sommes face à la situation inverse, l'interdiction est bel et bien là et les produits phytosanitaires ne sont plus fabriqués alors qu'aucune solution n'a été trouvé aussi, il convient de soutenir, de renforcer la recherche de méthodes alternatives. La solution la plus ma pas pragmatique serait de re-homologué temporairement les anciens produits dans l'attente de trouver des solutions efficaces dans l'incertitude de cette possibilité, la filière via le crier Pam souhaiterait soutenu, je ne peux que déplorer cette situation en ayant interdit ce type de produits avant que des solutions intermédiaires et pu être trouvé, l'une des réponses élaborées pour répondre à cette grave crise a été d'envisager des mesures d'aide à l'arrachage dans les territoires, ça été évoqué les 2 pleine est possible pour le en plantant des céréales. à l'initiative commune de Marie-Pierre Monnier de mon collègue Jean Yves Héroux et moi-même, le Sénat a voté décidé une large majorité, lors de la loi des finances rectificative de 2022, de créer une enveloppe budgétaire de 10 millions d'euros en vue d'aider à la rachat de certaines dans certaines zones, or les services ministériels explique aux professionnels de la filière que la réglementation européenne relative à la concurrence pour interdire de mettre en oeuvre de telles mesures considérées comme une aide exclusive en faveur des lavandes ni culteurs français toutefois, il semble que des solutions pour être trouvées, si les mesures d'arrachage intervient dans le cas de une restructuration une diversification de la filière, nous espérons que vous pourrez donner ou être convaincante pour défendre auprès de la Commission européenne l'octroi de ces 10 millions d'euros qui sont indispensables à la survie de l'des producteurs et des transformateurs de la bande, il faut peut-être pour éviter toute autre blocage que cette tête par la Commission puisse être envisagé de très étendu aux pays producteurs européens de la bande et de la vente d'un, Italie, Espagne et Grèce, par exemple, qui pourrait utiliser en cas de nécessité la sauvegarde de leur culture également, je vous remercie. Merci.

à un moment donné, vous pouvez avoir aussi un peu les mêmes interventions et donc vous aurez déjà déjà répondu donc il y a pas d'obligation, mais vous, c'est vous qui le c'est vous qui le souhaitez c'est pareil pour ne les collègues de venir à la tribune ou pas à la tribune, c'est comme comme une souhaite voilà et donc après vous, madame la ministre, le notre, notre collègue peut aussi avoir une minute là, vous avez 2 minutes et le collègue à une minute, voilà, j'espère avoir expliqué, c'est nouveau, un peu pour tout le monde aussi et puis c'est la rentrée là aujourd'hui. Je vous remercie, madame la présidente, et merci de votre question, et messieurs les sénateurs, évidemment je suis consciente des difficultés que traverse la filière colle et notamment, comme vous le disiez, en raison de l'augmentation rapide de la production de la Vendée de lavande, hein, ces dernières années et évidemment également le gouvernement soutient cette filière d'excellence et nous allons être très vigilants à ce que des solutions puissent être trouvées dans le sens d'une préservation, à la fois de la qualité de la production et des mythes et des métiers que la filière représente. Nous avons aussi conscience que la réduction de recours aux produits phytosanitaires, doit être associée à un accompagnement des filières professionnelles concernées et notamment pour les producteurs de lavande sur l'amendement que vous avez mentionné un dessinateur, qui prévoit effectivement 10 millions d'euros. Le cadre Le cadre réglementaire, sur les arrachages comme vous savez n'est pas très simple. Nous sommes en train d'expertiser avec la Commission européenne quant à la lecture précise de ce que permettent de faire ou non les textes européens en termes de diversification derrière un arrachage et pour cela, nous avons des échanges en cours avec les professionnels et nos services, il y a eu 2 réunions de tenues une troisième est prévenu, le 6 octobre pour établir les actions possibles et effectivement un plan d'action et j'ai bien noté ce que vous suggériez et je vous en remercie à ce stade, pour nous, c'est de travailler sur l'aide en trésorerie qui est sollicité et aussi d'objectiver le besoin en terme d'entreprise et de ciblage je vous remercie. Merci Je vous remercie, madame la ministre, une réflexion sur les produits phytosanitaires, la question d'aujourd'hui c'est que s'il n'y a pas une alternative rapide, il n'y aura pas de débat sur tout le reste concernant la lavande, parce qu'il n'y aura plus de la bande, aujourd'hui, la destruction de la lavande va à une vitesse vertigineuse et si il est pas décider dans les semaines qui viennent de proposer un mode de traitement efficace dans deux ans on aura plus besoin d'en parler, ce sera fini. Il la parole est à monsieur Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour cinq minutes chers collègues Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre groupe tient à remercier le président de la commission des Affaires européennes pour l'opportunité de ce débat qui interroge le sens de la construction européenne dans ses rapports avec les politiques publiques des États et la préservation de nos principes républicains, nous avons choisi de le traiter à la lumière du processus dit de Bologne et de l'élaboration par la norme d'un espace européen de lancement supérieur et de la recherche, cette thématique peut sembler surprenante tant cette politique paraît consensuel, nous estimons au contraire qu'elle est révélatrice, prise des aveuglements auxquels conduisent des gestion technocratique de domaines de l'activité sociale aussi spécifique et distinctif nos cultures nationales que ceux de la connaissance de l'éducation et de la science, le processus de Bologne a été lancée en 1999, il a été développé par l'Union européenne dans le cadre des objectifs économiques fixés par le Conseil européen de Lisbonne, en mars 2000 par les 15 États membres qui l'a composé alors et au sein du Conseil de l'Europe afin de constituer un espace européen de l'enseignement supérieur qui rassemble aujourd'hui 49 États, son ambition était de rapprocher les modes d'organisation des cursus universitaires de façon très pratique, il a notamment abouti à l'adoption par de nombreux systèmes universitaires de la succession des 3 années de licence des 2 années de master et les 3 années de Tess, son projet politique était de promouvoir un espace dans lequel les formations pourraient être évaluées, échanger et vendus comme des marchandises, il devenait alors possible d'assimiler les universités à des entreprises pour les mettre en concurrence et distinguer les meilleurs ce nouveau marché de la connaissance, ouvert sur le monde devait accroître l'attractivité de la science européenne susciter l'arrivée des chercheurs étrangers et augmenter les ressources des établissements par l'inscription d'étudiants étrangers sur le continent européen, la collaboration des universités de 49 États dans le cadre du processus de Bologne devait favoriser la démocratie par la libre-circulation des individus et des idées lors de la rencontre des ministre de l'espace européen de l'enseignement supérieur à Paris le 25 mai 2018, les participants ont constaté que plusieurs États ne respectait pas les libertés académiques des enseignants et des chercheurs, les signataires se sont engagés à les promouvoir et à les défendre, je les cite, grâce à un dialogue politique et une coopération intensifiée depuis lors les droits fondamentaux des universitaires n'ont cessé d'être bafoué dans l'Union européenne et dans les États membres du Conseil de l'Europe, c'est le cas, plus particulièrement en Turquie et en Russie, mais l'on pourrait citer aussi l'Azerbaïdjan ou la Biélorussie et plus près de nous, malheureusement, la Pologne et la Hongrie il y a une grande naïveté à penser que l'instauration d'un marché de la connaissance fondée sur les règles du management entrepreneurial, selon le processus de Bologne suffirait à garantir les libertés académiques et la démocratie, il est urgent de reconnaître que cette méthode technocratique et irénique a failli et qu'il est urgent de refonder la politique universitaire européenne sur les principes historiques théorisé par une Bolt la liberté de la recherche et de l'enseignement, l'unité de la recherche et de l'enseignement, la communauté scientifique entre enseignants et étudiants pour ceux-là, la déclaration de bonnes sur la liberté de la recherche est un outil précieux le gouvernement doit agir pour lui donner le statut d'une d'une norme juridique en France dans l'Union européenne et au sein du Conseil de l'Europe reconnaissons ensemble que la mise en oeuvre du processus de Bologne a accru les disparités entre les régions et finalement les conditions d'accès à l'enseignement supérieur, ne dispose pas d'université de 1er plan, tandis qu'en France l'offre universitaire se concentre de plus en plus sur les seules métropole cette polarisation du système universitaire est vécu comme une forme d'exclusion sociale supplémentaire par des populations qui subissent déjà une relégation économique dans ce domaine, comme dans de nombreux autres l'harmonisation européenne a été réalisée sans débat de fond sur le rôle fondamental de la connaissance et de l'enseignement dans l'émancipation des consciences, l'aménagement du territoire et la formation d'une citoyenneté européenne humaniste, je vous remercie.

je vais juste répondre à quelques points, vous m'en excuserez mais en 2 minutes, je, je dois être assez rapide, nous sommes très attachés au processus de Bologne et je crois qu'il n'est pas très juste de dire que c'est un processus commercial mais au contraire, c'est quelque chose comme vous l'avez dit vous-même, qui permet la libre circulation des individus, des idées qui offre à tous les étudiants européens la possibilité de travailler ou d'étudier dans tout l'espace européen. Ceci dit, le renforcement de l'éco-système, de la recherche n'est effectivement possible qu'en défendant les valeurs de liberté académique de recherche et d'expression et ce sont bien les piliers du monde universitaire c'est d'ailleurs pour cela que la France à oeuvrer en faveur de l'adoption de la maïzena charte Universiteit ou concomitamment au lancement du processus de Bologne et ah sous présidence allemande du Conseil de l'Union rejoint la déclaration de bonnes en faveur de la liberté de la recherche scientifique, bien sûr, nous allons être extrêmement vigilant à ce que les libertés fondamentales soient préservé et nous continuerons à l'être dans notre action et avec votre soutien je vous rejoins sur la protection de la liberté académique, c'est bien évidemment fondamental, mais c'est aussi dans cet esprit que la commode que la commission a adopté une boîte à outils dédiés au début de l'année, comme vous savez, elle incite des établissements à développer des stratégies pour prévenir et répondre notamment aux menaces d'ingérence étrangère si vous m'autorisez un mot de conclusion avec la PFUE, nous avons pu rappeler la vivacité du notre écosystème de recherche et notamment l'adoption, en mars 2022 de la déclaration de Marseille qui réaffirme le principe du respect des libertés académiques de toutes les collaborations internationales, je vous remercie.

il est pas disponible en français, nous avions espéré et le ministère des Affaires étrangères nous avait donné quelques assurances dans ce domaine que ce texte pourrait bénéficier d'une transposition dans le droit européenne, j'aimerais savoir où en est ce chantier, il est fondamental pour créer une citoyenneté scientifique européenne, nous devons aujourd'hui penser aux libertés académiques des universitaires en Hongrie et en Pologne, qui souffrent de la mainmise de l'État sur leur système universitaire, on ne peut pas concevoir un espace de la recherche, dans laquelle la liberté fondamentale des chercheurs ne soient pas respectées merci Namyst. Merci, la parole est à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Madame la présidente, madame la Ministre, mes très chers collègues merci à notre président de commission d'avoir permis ce débat important dans notre rapport, Europe et Patrimoine rédigé au printemps avec Louis-Jean de Nicolaï, nous proposions une stratégie européenne ambitieuse pour le Patrimoine, il semble que nos espoirs puisse aboutir sous la présente président tchèque dans le cadre du nouveau programme d'action quadriennal 2023 2026 pour la culture, dont nous espérons hein Dax Patrimoine fort, or cette Europe du Patrimoine des cathédrales, des châteaux, des monuments historiques des savoir-faire est aujourd'hui menacée en son sein par une tentative vertueuse dans son principe de réglementation de l'usage des produits chimiques. Alertés par les professionnels du vitrail à quelques-uns, nous avons écrit à notre ministre de la Culture, tandis que notre collègue Vanina Paoli-Gagin déposer une pépère dont nous avons été aéroport rapporteur avec mon collègue Louis-Jean de Nicolaï, nous avons établi les graves dommages qu'entraînerait la révision envisagée par l'Agence chimique européenne et du règlement Reach, l'inclusion du à l'annexe 14 de ce règlement concernant les substances Dick particulièrement préoccupante implique une procédure d'autorisation, un coût prohibitif pour les utilisateurs, plusieurs mois de montage de dossiers d'expertise et le versement d'une redevance à cas plusieurs dizaines de milliers d'euros selon la taille de l'entreprise, il en irait à court terme de la survie même des TPE et PME françaises du secteur du Patrimoine par une telle procédure devant de toute façon, selon which céder la place à une interdiction pure et simple, mes chers collègues doivent jouer leur rôle de lanceur d'alerte auprès de leurs gouvernements représentés dans le comité d'experts de l'Agence telle hé bien le sens de la résolution européenne du Sénat, Madame la Ministre, nous avons également adressé un avis politique, à la Commission européenne du reviendra en effet, de suivre ou non la recommandation de les cas puis de proposer en principe sous de 12 mois un projet de règlement qui devrait donc intervenir d'ici la fin de l'année 2023 madame la Ministre, confirmez-vous ce calendrier, tout comme les maires, maître verrier, nous sommes inquiets, car la France concentre plus de 60 % du Patrimoine de vitraux européens la plus grande surface du monde, de nombreux joyaux de nos régions sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco bien d'autres secteurs et métiers du Patrimoine sont concernés, nous en avons dressé la liste dans notre rapport et la pépère, adopté en commission, je mentionne qu'ici les facteurs d'orgues, près de 10000 or recensés en France, 1600 sont classés les Manufactures d'orgues représentent environ 65 entreprises toute petite par le nombre de leur employé mais grande oh combien par leur savoir-faire, l'interdiction du recours au plomb, mes chers collègues, ou la lourde procédure d'autorisation entraînerait la perte de cet immense Patrimoine et à terme de la musique d'orgue elles-mêmes certes le plomb est un polluant bien identifié, nous sommes bien conscients des risques, ceux-ci sont connus et pris en charge de manière générale dans le secteur du Patrimoine des procédures et des guides de bonnes pratiques ont été depuis un certain temps, élaboré par le ministère de la culture et les organismes professionnels, nous pensons qu'il devrait être plus largement diffusé, y compris au niveau européen. Alors nous ton malgré tout qu'à ce jour il n'existe. Aucune donnée épidémiologique fiable mettant en question en France ou en Europe, la santé des travailleurs exposés au plomb dans ce domaine, nous appelons donc Madame la Ministre à la réalisation d'études spécifiques dans le cadre des programmes de recherche européens, nous avons d'ailleurs récemment attiré l'attention de la commissaire Maria Gabriel sur ce sujet, il existe donc bien, d'autres voies et moyens d'agir pour la santé que celle d'une révision quasi automatique de riches, faute de quoi, c'est toute une culture européenne toute une économie touristique, patrimonial mes vitrines de nos territoires qui disparaîtront, l'harmonisation européenne ne saurait faire passer toute cette richesse par pertes et profits, au nom d'objectif certes louable mais au moyen de procédures contestables et manquant de transparence, Madame la Ministre du coton là vraiment sur la mobilisation du gouvernement dernière remarque l'alerte lancée par nos Lussier Arche Thiais quant à l'usage du Pernambouc, bois précieux d'Amazonie réglementée par la convention internationale sur le trafic d'espèces menacées : la France est

les conséquences très graves pour le secteur et la profession, merci beaucoup, madame la ministre, de vos réponses.

donc, sincèrement, je vous demande de de faire attention et quand je dis Stop, stop, Madame la Ministre. Madame la présidente, merci monsieur le président, madame la sénatrice, hein, d'abord, permettez-moi de saluer le travail que vous avez effectué, effectivement avec avec avec vos collègues sur ce sujet et soyez assurés qu'avec mes collègues de la culture et de la transition écologique, nous sommes pleinement conscients des interrogations, des inquiétudes, des corps de métiers du Patrimoine qui concerne la classification du plomb au titre du règlement Reach. d'abord les m'rappelé que l'identification des propriétés toxiques du plomb, notamment pour la reproduction n'est pas nouvelle puisque cette substance figure depuis juin 2018 sur la liste des substances extrêmement préoccupantes du règlement Reach, ensuite je souhaite revenir sur la procédure qui a conduit à la classification des substances et notamment, comme vous le mentionnez une éventuelle inscription à l'annexe 14 qui liste les substances dont l'usage est soumis à autorisation et pourquoi, parce que cette procédure repose sur une large association de l'ensemble des parties prenantes concernées comme vous savez, l'Agence européenne des produits chimiques procède systématiquement à une consultation publique pour recueillir des informations sur les usages et les tonnages qui seraient susceptibles de modifier les scores de la substance et donc son ordre de priorité par rapport aux autres substances préoccupantes et ce, avant d'adopter une recommandation, cette consultation a été organisée du 2 février au 2 mai 2022. Et l'ensemble des parties prenantes concernées fédérations professionnelles et autorités des françaises ont pu contribuer pour fournir des informations notamment sur les impacts socio-économique et culturels de cette mesure, en parallèle, la commission a mené une consultation publique pour obtenir des informations sur les mêmes impacts socio- économique et culturel que pour avoir une éventuelle inscription à l'annexe 14 et ces ces informations qui serviront à déterminer la proposition qu'elle fera une fois la recommandation n'Agence européenne des produits chimiques adopté, vous m'avez demandé le calendrier, effectivement, elle devrait l'adopter d'ici à la fin de l'année 2022, ensuite la commission proposera un projet de règlement et elle ne sera pas tenu de proposer l'inscription du. Selon à l'annexe 400 Madame la Ministre, vous pourrez répondent je pense sur.

nous les connaissons déjà puisque vous me réexpliquer le le processus, nous connaissons bien les règles qui ont présidé à la à la consultation, les résultats de la consultation, nous, nous voulons simplement vous alerter sur la procédure qui manque singulièrement pour nous de rigueur, pouvez-vous plaider à ce qui est des recherches épidémiologiques scientifiques rigoureuses fiable des chiffre sur lequel on puisse objectivement s'appuyer pour décider ou non de cette inscription au règlement Reach, c'est ni plus ni moins la méthode que nous contestons et son absence de transparence je pense, des gouvernants et des gouvernements en Europe d'agir dans ce sens, plutôt que de risquer des conséquences extrêmement graves pour tout un secteur de notre économie et de notre culture, merci madame la Ministre de votre écoute. Merci, la parole est à monsieur Jean-Pierre Corbisez pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour cinq minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, merci de cette proposition de débat aujourd'hui, mes chers collègues, au fil des décennies le projet européen s'est affirmée autour de valeurs communes et nourri de politique toujours plus protectrice pour nos concitoyens de la simple mise en commun des ressources nécessaires à la reconstruction de l'Europe d'après-guerre, nous sommes aujourd'hui à une Union européenne très volontariste sur presque tous les domaines, mon groupe RDSE il se il est effectivement actuellement profondément attachés à l'Europe, et bien entendu favorable à la mise en place et l'approfondissement de politique européenne répondant aux défis du quotidien qu'ils soient économiques, socio-sécuritaires environnementaux ou sanitaires, chacun des États membres, a ses spécificités liées à son histoire et à son territoire, je devrais même dire à ces territoires, ce constat est une évidence, mais il convient de le rappeler au triptyque institutionnel que forment le Conseil, la Commission, le Parlement européen, compte tenu de l'élargissement croissant des compétences de l'Union européenne et du principe de supranationalité du droit européen, il nous semble important d'être vigilant quant au chant des directives et règlements. C'est d'ailleurs ce que fait avec rigueur, le groupe de subsidiarité au Sénat, j'en profite pour saluer la qualité de son travail, il ne s'agit pas de dire que l'Union européenne, ni la diversité d'autant moins que le traité sur l'Union européenne, souligne que l'Union respecte respecte l'identité nationale des États ou encore la richesse de sa diversité culturelle toutefois certaines dispositions peuvent heurter des traditions, des cultures, des richesses territoriale, parfois même les menacer, nous avons tous connaissance d'exemples récents concernant les réglementations européennes % portant sur pesant pardon sur certains savoir-faire ma collègue vient de le dire, je pense effectivement aussi au règlement européen Reach sur le contrôle des substances chimiques qui m'en danger la profession des vitrailliste en interdisant purement et simplement l'usage du plomb, la France, terre de vitraux pourrait voir ainsi disparaître un artisanat unique que serait la reconstruction de notre dame de Paris sans ses vitraux à la française, comme vous le savez madame la Ministre sur le Sénat s'est ému de cette situation, à travers la résolution du 26 août dernier qui l'a adopté, vous avez été également il a alerté, comme l'a dit un de mes prédécesseurs en particulier par mon collègue Jean-Yves Roux sur la vie dans la filière de la lavande et du lavande, hein, dans la production et ses dérivés sont directement menacés par un changement de réglementation européenne alors que la filière doit faire face à une attaque parasitaire, ainsi qu'à une concurrence très importante et multiples tests qu'entraînerait la changement de classification des huiles essentielles à base de la vendre risque de fragiliser, de nombreux acteurs du secteur, au-delà de la richesse que représentent ces plantes dans la culture provençale, c'est d'abord près de 9000 emplois Directs qui seraient impactés et que serait le tourisme des Alpes-de-Haute-Provence ou du plateau de Valence sol sans ses champs de lavandes sans méconnaître les nouvelles exigences des consommateurs est important que les États conservent une certaine latitude dans la façon de les protéger, à mon sens afin et afin d'éviter les mauvaises surprises liées à une harmonisation trop rigide d'énormes, il faut garder à l'esprit quelques axes il faut tout d'abord veiller à ce que l'exécutif national et vite la surtransposition comme cela peut parfois arriver à cet égard, je rappellerais que nous avions adopté ici en 2018, un projet de loi portant suppression de surtransposition des directives européennes en droit français, il est également fondamental que notre pays se mobilise, très en amont de l'élaboration des projets de directives afin de peser au plus tôt, dans les négociations qui préside à leur élaboration je dirais je dirais également un mot de l'inflation normative il n'un épargne pas les institutions européennes dès 2014, la Commission européenne avait lancé un programme intitulé Mieux légiférer s'était traduit par une réduction importante du nombre d'initiatives nouvelles de la commission, madame madame la ministre, qui est devenue depuis cette volonté exprimée à l'époque par Jean-Claude Juncker, la lutte contre l'inflation des normes au sein de l'Union, enfin la une amélioration des analyses d'impact des axes européens dans les États mérite d'être explorées, c'est en effet le meilleur moyen de sauvegarder dans nos territoires toutes les richesses culturelles et patrimoniales qui participent de l'exception attractivité de la France. Je vous remercie,

Madame la Ministre, non, c'est bon, il sera donc oui bisous non c'est bon d'accord merci. Alors la parole est à monsieur Louis-Jean de Nicolaï pour le groupe Les Républicains et pour cinq minutes. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, à mon tour, je me réjouis de ce débat et je tiens à remercier comme l'a fait Catherine Morin-Desailly, le président Jean-François Rapin d'en avoir demandé et obtenu l'inscription je souhaite aussi apporter mon soutien aux propos précédents de ma collègue Catherine Morin-Desailly présenté au donc présenté au printemps, notre rapport d'information proposant une stratégie européenne ambitieuse pour le Patrimoine, nous avons cet été présenté un rapport qui est 2 abouti un avis politique destiné à la Commission européenne, ainsi qu'une résolution du Sénat afin de prendre en compte toutes les conséquences pour les métiers et filières du Patrimoine de la révision en cours du règlement européen Reach sur les produits chimiques, eu égard à l'éventuelle inscription du plomb dans son annexe or l'usage du plomb, comme l'ont montré les nombreux professionnels que nous avons est indispensable à la conservation et à la restauration de ce précieux héritage en effet la taille de Pierre classique utilise du plomb la la malléabilité et la durabilité du plomb concours à la conservation de long terme des bâtiments anciens certaines toitures historiques sont également constitués de plomb, c'est le cas de celle de nombreuses cathédrale tout pas culturellement là déjà citée notre hein de Paris mais aussi de de nombreux monuments comme le château de Versailles, le musée du Louvre où les châteaux de la Loire, c'est pourquoi nous avons entendu notamment le Groupement des entreprises de restauration des monuments historiques, qui fédère 252 entreprises de 12 métiers employant 10000 salariés dont environ 1000 apprentis en France, les tailleurs de Pierre, des monuments historiques ont 78 entreprises employant quelque 5000 salariés pour un chiffre d'affaires estimé à 600 millions d'euros et couvreur les monuments historiques, compte 39 entreprises employant 1500 salariés pour un chiffre d'affaires

de plus, les musées, les institutions patrimoniales de l'Union européenne et du monde entier conserve de très nombreux objets d'art et biens culturels contenant du plomb dont vous trop retrouverez la liste dans notre rapport, les insignes et des médiévaux et aux voitures anciennes nous ne négligeons nullement l'enjeu sanitaire, bien évidemment, nous avons constaté de visu en nous rendant sur le chantier de restauration d'une église historique au coeur de Paris, l'importance des mesures prises en terme de prévention par la législation française la réalité l'intense, l'intensité des contraintes pour les entreprises et les intervenants et les contrôles imposés pour la bonne protection de la santé des travailleurs concernés en matière de santé au travail, le code du travail français a prévu 2 indicateurs permettant de vérifier l'efficacité des mesures de prévention mises en place vis-à-vis du risque plomb la valeur limite d'Exposition professionnelle plomb et la plombémie avec des valeurs limites biologiques à ne pas dépasser le code du travail prévoit également que le médecin du travail, assure un suivi individuel renforcé dès le dépassement de certains seuils ces valeurs limites sont susceptibles d'être abaissé et harmonisées au plan européen, dans le cas de la révision de la directive de 1998 sur les agents chimiques, ce qui renforce les exigences de prévention, nous sommes toutefois favorable à ce qu'un protocole national, voire européen de prévention du risque plomb sur les chantiers des monuments historiques soit instauré sur le fondement des protocoles instaurée récemment sur les chantiers français comme à Paris, Nantes, Rouen, Clermont-Ferrand cette voie nous semble bien préférable à une révision du règlement Reach pour les fans, familles, il faut le dire du Patrimoine qui constitue l'objet de la présente proposition de résolution le moyen le plus sûr de garantir une telle exemption serait donc le statu quo, si la Commission européenne jugeait toutefois nécessaire de de durcir les règles d'usage du plomb dans le secteur industriel, elle pourrait aussi bien reconnu recourir à d'autres législations européennes existant par ailleurs dans le Champ du travail ou de la santé législation qui, elle, relève de la procédure de codécision, mais elle devrait alors veiller à bien d'exempter les filières patrimonial de telles dispositions, il importe que louer en français, Madame la Ministre, s'engage en ce sens et mobilisent son représentant au comité pour éviter une désastreuse, inscription du plomb à l'annexe 14 du règlement Reach, la France appartient aujourd'hui au groupe des pays les plus ambitieux en Europe en matière de gestion des risques des substances chimiques des des nos mérite déterminée à promouvoir des avancées ambitieuses pour la sécurité environnementale, elle est d'autant plus légitime, a plaidé pour une telle exception culturelle qu'elle est dotée d'un Patrimoine culturel exceptionnel, l'Europe peut et doit concilier l'un et l'autre, notre responsabilité de parlementaires et de le rappeler avec force et d'inciter le gouvernement madame la milice à le faire savoir auprès de toutes les institutions européennes, je terminerai en rappelant simplement que 84 % de l'utilisation du plan concerne les batteries. Merci ça ainsi : Madame la Ministre. Merci madame la présidente, merci, je vais répondre à messieurs les sénateurs corbeille et de Nicolas et ainsi qu'un complément de réponse pour la sénatrice Morin-Desailly en ce qui concerne les études, l'Agence européenne de produits chimiques et base ses recommandations sur des études scientifiques qui devrait pouvoir être consultés et qui sont ceux que vous avez demandé, et je voudrais juste ajouter que même si le plan devait être inscrit à l'annexe 14, ça ne veut pas du tout dire que l'usage de la substance serait totalement interdit, comme vous savez,

règlement Reach et sa révision et c'est moi d'abord dire que le projet de révision ne prévoit rien qui mènerait à une interdiction de facto de l'huile essentiel de la vente, c'est, c'est la première chose, la 2ème, c'est que bien sûr nous sommes conscients de l'importance de l'industrie des huiles essentielles, et plus particulièrement pour la France et qui n'est pas question d'accepter une révision du cadre existant qui serait déraisonnable au regard des enjeux socio-économiques et nous plaidons pour une proportionnalité afin d'éviter l'établissement de contraintes et de contrôles excessifs et aussi une étude d'impact suffisamment complète pour analyser toutes les conséquences potentielles pour l'emploi de la filière et je rajouterai en conclusion. Que bien sûr nous savons que la filière des huiles essentielles et t'inquiète des évolutions à venir du règlement CLP et nous en avons parlé notamment au sein d'un comité interministériel qui s'est réuni 3 fois entre décembre 2021 et avril 22 et comme on me demande des études, il y a une étude financée par FranceAgriMer, qui a été lancée pour mieux comprendre les impacts des évolutions réglementaires sur la filière dix-huit l'essentiel, ce qui va nous aider à mieux accompagner la filière : nous avons les premiers résultats, le rapport final devrait être bientôt disponible et nous vous transmettrons les résultats de cette étude, merci. Merci madame mamie monsieur de Nicolas que vous voulez. Contre monsieur Corbizet non d'accord, merci, donc, la parole est à Madame Colette Mélot pour le groupe, les indépendants et pour cinq minutes chers collègues. Merci madame la présidente, monsieur le président de la commission des Affaires européennes, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'élaboration des réglementations européennes ne se fait pas sans certaines précautions, ce que nous savons bien au Sénat où nous prenons à coeur notre rôle de contrôle de subsidiarité l'idée d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, pour reprendre l'article 1er du traité sur l'Union européenne ne signifie pas une harmonisation qui irait à l'encontre de certains principes l'article 3 du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du Patrimoine culturel européen, chacun sait dans cet hémicycle, la chance que représente l'Union pour nos territoires nos savoir-faire et nos cultures, elle, elle préserve les promeut et les accompagne dans leurs évolutions, avoir un système harmonisé au niveau européen, dans bien des domaines, permet à nos nos citoyens de mieux vivre et d'être mieux protégés, le dernier exemple en date, et le marché intérieur de l'énergie qui, bien que perfectible et c'est en bonne voie, nous montre toute l'importance de l'Union européenne et de nos interconnexion cependant cette harmonisation ne doit pas se faire au détriment de nos particularités le processus législatif européen très complexe, nous laisse parfois perplexe, beaucoup se rappelle encore du règlement encadrant la forme et la courbure du concombre abrogé depuis 2009, je tiens à le préciser, mais ce processus est toutefois ouvert et transparent, la Commission européenne procède à de nombreuses consultations sur des nouvelles législations ou à dix évaluation de laisser Gilles de législation déjà en vigueur autre coté en tant que parlement nationaux, nous avons le devoir de nous assurer du respect du principe de subsidiarité dans les législations proposées malgré tous les encadrements existant certains sur sujet ne sont parfois pas suffisamment pris en compte dans l'élaboration des règles et leur harmonisation cela peut mener à des situations compliquées sur nos territoires et pour nos concitoyens, 2 exemples sont particulièrement éclairant le 1er concerne notre savoir-faire et notre Patrimoine et a été porté par l'une de mes collègues du groupe, les indépendants, le sénateur Vanina Paoli-Gagin actuellement, la Commission européenne réfléchit à une révision du règlement que l'on appelle communément riche et dans ce cadre, envisage d'interdire l'utilisation du plomb, cela a été déjà évoqué pépère, adopté le 26 août dernier explique tout l'enjeu de nuancer cette interdiction, notamment pour le secteur du vitrail, nous avons la chance en France de détenir la plus grande surface de vitraux du monde, les rapporteurs du texte, faisait remarquer qu'environ 60 % des vitraux européens se trouvent dans notre pays, notre savoir-faire et quasi unique, il est impossible à nos artisans de se passer du plomb, d'ailleurs, cette filière a mis en place toute une série de mesures pour protéger et prévenir les risques liés à la manipulation du plomb, notre Patrimoine et certain savoir-faire, mais représente aussi des milliers d'emplois sur nos territoires et va même au-delà en mars 2001 le président Jacques Chirac, s'exprimant lors de la remise du titre du meilleur Oviir ouvrier de France a justement rappelé que ce sont des savoir-faire reconnus qui assure une très large part la renommée de notre pays dans le monde entier et j'ajoute la renommée de l'Europe, il était important que les territoires, les savoir-faire et les cultures soient mieux prises en considération dans la construction des règles européennes, au risque aussi de perdre nos identités, le second exemple se trouve sur mon territoire, il concerne l'AOP Brie de Meaux et l'AOP Brie de Melun l'obtention de ces AOP a été compliqué, ce qui est normal lorsqu'un cahier des charges doit être défini pour un produit d'excès d'exception grâce à de nombreux acteurs sur le département, et notamment les confréries, nous avons pu mettre en valeur ses fromages, les confréries sont précieuses sur les territoires, elles ont un rôle de garant de nos savoir-faire, de notre culture et de notre Patrimoine, elles connaissent les besoins et souvent soulève des problèmes, il en existe plus d'un millier en France, je dois dire, ainsi que des ambassades, des produits du terroir, c'est pourquoi je pense qu'il y a un besoin, certes il y a un besoin certains d'ingénierie territoriale sur le modèle d'une d'une des propositions que j'avais formulé lors de mon rapport d'informations pour une mobilisation plus ambitieuse des fonds européens au service de nos territoires, cela permettrait de faire remonter des besoins et des problématiques des territoires comme celle que je viens d'évoquer, de les accompagner, il me semble que l'échelon départemental serait tout indiqué, qu'en pensez-vous Madame la Ministre, c'est le rôle des centres Europe directe qui ont commencé à voir le jour dans certains départements ou dans des villes ainsi que le réseau des maisons de l'Europe, cela renforcera ainsi le lien entre l'élaboration des réglementations et les besoins des citoyens et territoires européens et, in fine, et parce que nous en avons plus que jamais besoin entre l'Union européenne et les Européens. Merci, chers collègue, Madame la Ministre. Madame la présidente, merci madame la sénatrice alors je je crois que j'ai assez parlé du plomb et du vitrail, juste 2 mots peut-être sur le brie de Meaux et avec un petit focus est un peu plus sur la question que vous m'avez posé comme vous savez quand on, quand on essaye et fait quand effectivement le l'Europe protège avec des appellations d'origine, AOP, les produits du terroir l'organisme de gestion et de défense, le DG a pour fonction de rédiger le cahier des charges des produits qui sont sous signe d'identification de la qualité d'origine tels que l'AOP, ou bien j'ai pris le Label rouge, tout n'est pas parfait mais dans le cas du brie de Meaux, je pense que la façon dont ça a été fait, le sujet a lieu à l'aire géographique de la production de Brie de Meaux pour lesquelles effectivement des oppositions ont été et qui n'ont pas été jugée recevable parce qu'elle ne portait pas sur le cahier des charges sur des éléments de cahier des charges qui peut faire l'objet d'une modification puisque il s'agit d'aires géographique, hein, et une des raisons pour cela, c'est que le DG n'a n'évolue pas dans son positionnement, donc c'est peut-être une action plus national qui doit être menée afin de la convaincre puisque son son et que la production actuelle est suffisante, qu'elle est bien répartis dans l'ensemble de l'aire géographique et qu'elle permet même. Une réserve de lait, alors j'ai bien conscience de la sensibilité de ce sujet et au regard notamment de l'ancienneté des demandes qui ont été faites en ce sens, si on peut en discuter à côté bien sûr, je serais ravi de vous écouter merci. Ah si Madame Mellow, vous avez une minute. Je vous remercie, madame la ministre, j'avais aussi évoqué la Brie de Melun, qui a été accordé, parce qu'elle correspond à l'aire géographique

Merci, cher collègue, hein dérouleur va vous êtes distribuée puisque nous avons une panne numérique, donc là je vais donner la parole à monsieur Jacques Fernique, donc pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour cinq minutes et ensuite ce sera Madame Schillinger. Merci madame la présidente, madame amis chers collègues oui on, on le voit les les propositions d'harmonisation des normes de la Commission européenne peuvent être hors sol ainsi, ça a été dit et répété, la révision du règlement Reach entièrement élaboré à Bruxelles manque un peu de prise en compte des réalités spécifiques, notre président de Commission parlait il y a quelques instants des des dangers d'harmonisation aveugle, déréglementation du marché intérieur avec Reach, c'est manifestement le cas, il concerne les substances chimiques mais aussi, on l'a dit, les huiles essentielles : la vendent particulièrement importante pour notre patrie en naturel, la révision des règlements, alors il y a, riche et CLP étiquetage avec ceux là les les exigences vont encore augmenter, et la filière d'huile essentielle dans sa diversité, il y a pas que le la la vente il y a l'eucalyptus, il y en a d'autres ne va pas réussir à s'adapter face à des méthodes d'évaluation, il faut il faut insister là-dessus, conçu pour la chimie de synthèse ne laissons pas des règlements, mettre à mal ces filières, alors même qu'il n'apporte, dans ce cas précis, aucun gain de sécurité pour les consommateurs Nous plaidons et le bon sens, je pense avec nous en faveur d'une harmonisation européenne des normes quand elles ont pour objectif des plus-values, sociales, environnementales, sanitaires économique quand elles savent tenir compte de la clairvoyance des acteurs locaux, mais dans ce cas précis, l'UE a une vision un peu technocrate sur des produits traditionnels les élevant même rang que des produits chimiques classiques, cette démarche est hors sol on l'a dit l'interdiction européenne du plomb et la lourde procédure d'autorisation prévue serait catastrophique pour les métiers du Patrimoine français des vitraux, on a alerté, donc ça a été dit par la résolution de la commission des Affaires européennes, et notre collègue Morin-Desailly vient de le rappeler très clairement notamment ceci dit critiquait les défauts des propositions de loi européenne n'exclut pas, à l'inverse de dénoncer également les retards français pour transposer et appliquer des directives, je pense à la qualité de l'air à la directive-cadre sur l'eau à la gestion des décès des déchets est un exemple précis, très actuel de non respect par la France de normes européennes, c'est celui du chanvre et plus particulièrement du CBD pour lequel nous observons des des blocages gouvernementaux importants limitant la possibilité d'une filière d'un savoir-faire, de se développer, alors même que nous disposons de ses savoir-faire, des conditions et du cadre juridique européen nécessaire pour se faire la demande de CBD non psychotrope non toxique, il faut le dire et forte et l'opinion publique est favorable, le développement de cette filière en France a un potentiel économique important pourtant nos autorités n'autorise pas l'usage de la fleur, et donc l'extraction de CBD non psychotrope, la France a donc été condamné, le terme est clair, par la Cour de justice de l'UE sa réglementation étant contraire au droit européen, je vous renvoie sur ce sujet à la résolution transpartisane cosignée par plus d'une cinquantaine de sénatrices et sénateurs et en novembre, je crois, nous aurons l'occasion d'un débat dans notre hémicycle enfin. Je dirais que l'harmonisation des législations fiscales, sociales et environnementales au niveau européen, c'est pas une orientation idéologique de pro-européen de fédéralisme forcené, mais c'est aujourd'hui une nécessité si nous ne voulons pas que l'Union européenne s'effondre et nos écosystèmes avec, en effet, si on prend la dimension écologique, l'harmonisation des normes européennes tombe sous le sens, on ne lutte pas, c'est évident qu'on ne le réchauffement climatique en agissant seul dans son coin et certaines règles pour les pesticides, par exemple, vont devoir être harmonisées au niveau européen la subsidiarité ne doit pas servir de prétexte à l'immobilisme, par exemple, élever des poules ou des lapins dans des cages de la taille d'une feuille format A4, c'est pas une tradition, c'est une mauvaise pratique qui perdure, quel bénéfice par ailleurs et je ne parle pas uniquement de bénéfices économiques tirons-nous de traditions comme la corrida, par exemple, pour conclure, puisqu'il me reste une minute, il me paraît nécessaire de rappeler que nous ne pouvons pas nous contenter de normes écologiques, sociales et sanitaires à usage interne, il s'agit d'éteindre ses exigences à nos importations, pour le devoir de vigilance sociale et environnementale de nos entreprises, pour toute leur chaîne de valeur par delà les frontières mais également Madame la Ministre, pour nos accords commerciaux, on nous a promis que nous allions entrer dans une nouvelle ère du commerce européen, nous attendons toujours un peu à quand désaccord contenant des clauses miroirs réellement appliquée, de respect de nos normes européennes, l'accord de libre-échange signé récemment entre la Nouvelle-Zélande et l'Union Européenne en est loin, très loin, c'est pourtant peut être aussi par là certainement d'ailleurs que nous préserverons la vitalité et la riche diversité de nos territoires de leur savoir-faire et de leur culture. Merci. Collègue, Madame la Ministre. Merci madame la présidente, merci monsieur le sénateur, vous avez couvert, hein, un vaste Champ des sujets, donc j'espère que je bénéficierais de votre indulgente pour ne traiter que quelques points en ce qui concerne la révision du règlement Reach permet moi témoin assisté la révision n'est pas fait et la Commission européenne devait ne devrait proposer ses projets de révision pas avant la fin de l'année 2022 il y a donc encore des consultations et des discussions qui sont possibles et, bien sûr, nous portons les intérêts de nos territoires, à ce sujet, permettez-moi aussi de rappeler que ce règlement permet aux États membres de s'appuyer sur des. Analyse de risques, hein, des listes de substance commune afin de protéger les consommateurs et l'environnement. Si je peux, outre le fait de souligner qu'il y a des consultations au niveau national, régional, départemental et que vous-même, vous pouvez faire des projets de propositions, on ne peut pas prendre ce qui nous arrange dans l'Union européenne et et rejeté, ce qui nous arrange pas, ce sont des discussions que nous avons à 27 et sur lesquels nous essayons d'avoir des positions communes, parce qu'à 27, nous sommes plus forts, notamment comme vous le savez, dans les négociations commerciales, et je vous remercie d'avoir mentionné ce projet, l'accord de commercial avec la Nouvelle-Zélande et le premier qui a des clauses environnementales fortes et qui, quand je le lis et je me demande toujours pourquoi les la Nouvelle-Zélande a accepté de signer, tellement il nous est effectivement favorable et protège nos appellations contrôlées, il y a effectivement des clauses miroirs qui sont de grandes avancées de la présidence française de l'Union européenne et qui, comme vous le savez, vont demander aux personnes qui souhaitent exporter dans l'Union européenne d'appliquer les mêmes règles

pour les autorités nationales, les acteurs locaux, régionaux, de se faire entendre, j'espère que notre gouvernement il contribuera en ce qui concerne la nouvelle génération d'accords commerciaux, vous le savez, je suis moins convaincu que vous. Merci, la parole est à Madame Patricia Schillinger pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour six minutes chers collègues. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'Union européenne à travers sa réglementation, d'harmonisation veille à lever les obstacles à la libre circulation permettant des l'existence d'un marché unique sur lequel les consommateurs ont accès à des produits sûrs de qualité et dans des conditions de transparence, il n'est pas impossible de voir certaines professions ainsi que leur savoir-faire mis en difficulté dans le cadre de l'élaboration des normes européennes en juillet dernier, notre commission a choisi de porter son attention sur le régime européen d'autorisation de l'usage du plomb et son incidence sur les éléments constitutifs du Patrimoine européen par une proposition de résolution européenne, nous avons souhaité encourager la commission et le gouvernement à préserver l'activité des vies et autres professions d'art menacés par l'interdiction du plomb qui pourrait intervenir dans le cadre de la prochaine révision du règlement dit Éric relatif aux substances chimiques par cette proposition, notre commission a ainsi affirmé la nécessité pour l'Union européenne de reconnaître et protéger ses métiers leur savoir-faire qui composent notre Patrimoine européen qui en font la richesse et celle de nos territoires, elle a en fait de même concernant la préservation de la filière 18 essentiel à base de lavande menacée elle aussi par par la révision du même règlement riche notre commission a défendu cette filière en affirmant que nos huiles essentielles de lavande, ce sont des produits agricoles, artisanaux non chimiques et que la filière de l'herboristerie fait partie intégrante du Patrimoine immatériel immatériel français en outre le Sénat chambre des territoires s'attelle à ce que ces derniers, les savoir-faire et les cultures dont ils sont porteurs soient défendus et représentés dans l'élaboration de la norme à l'échelon national comme européenne, je remercie d'ailleurs notre commission d'avoir mis à l'ordre du du jour ce débat plus largement dans un espace européen marqué par la libre-circulation des produits qui sont l'emblème des 2 territoires porteur d'un savoir-faire et fruit d'une culture peuvent être mis en concurrence avec des importations susceptibles dans le juge d'en usurpé la qualité, la provenance a aussi valoriser ces savoir-faire par une Indication géographique permet tout d'abord de rassurer le consommateur quant à la provenance et la qualité réelle d'un produit, elle met en avant les producteurs locaux authentique et les protège de la contrefaçon, elle valorise les particularités des patrimoines locaux favorise l'emploi et pérennise les savoir-faire, c'est ce que le droit européen autorise les États, sous couvert de la protection de la propriété intellectuelle et commerciale sont autorisés à protéger ses produits spécifiques au moyen d'appellation géographique avec la loi dite consommation : la France a ainsi, sur le modèle de ce qui se fait en matière agroalimentaire mis en place l'idée des indications des indications géographiques en matière d'industriel et artisanal, le recours à tel indication permet d'interdire l'usage de l'appellation aux entreprises qui n'en reste respecte pas le cahier des charges en France, c'est l'Institut national de la propriété propriété industrielle, qui gère les indications géographiques et les homologations toutefois une simple protection nationale présente des limites et c'est bien là tout l'enjeu d'une reconnaissance européenne plus accentuée, en effet, en l'état, l'absence d'un système harmonisé au niveau européen de reconnaissance des indications géographiques revient à laisser à la seule charge des États le soin de garantir et de préserver ce qui fait la richesse et aussi la raison d'être de l'Union européenne, sa diversité, inégalement protégée d'un État à l'autre, cette absence de cadre harmonisé pénalise les métiers traditionnels et leur production, or dans le prolongement de la crise sanitaire, l'exigence de protection et forte la libre-circulation et l'accès aux marchandises ne suffisent plus et les citoyens européens attendent de l'Union qu'elle les protège la culture et le savoir faire qui figure au coeur de leur identité et à forte au coeur de l'héritage européen font partie des éléments qu'il soulève souhaite protéger poterie d'Alsace savon de Marseille faïence de et espadrilles basse tous doivent pouvoir bénéficier d'une reconnaissance et d'une protection européenne, c'est en ce sens que nous saluons la proposition formulée en avril dernier par la Commission européenne d'un règlement sur les indications géographiques non agricoles, elle propose d'un d'instaurer au niveau européen une indication géographique des produits artisanaux et industriels dont la gestion serait centralisée et l'obtention simplifiées, les négociations devraient se poursuivre sur sous la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne pour une entrée en vigueur en 2024, c'est ce que nous encourageons et souhaitons ce sera une étape décisive pour la prise en compte des territoires, des savoir-faire et des cultures dans le l'élaboration des réglementations européennes d'harmonisation, nous y serons attentifs pour la défense de notre Patrimoine français et européens pour nos producteurs avec un souci de protection des consommateurs, je vous remercie.

qui, comme vous le soulignez, sont vraiment importantes pour nous et la révision législative européenne sur ses indications, est un sujet que nous suivons de très près, et bien que nous nous ne partageons évidemment les objectifs poursuivis par la Commission mais nous avons des points points de vigilance que vous avez pu évoquer et est mentionné dans vos différentes interventions, puisque l'harmonisation des pratiques et c'est un sujet qui est revenu beaucoup sur la table aujourd'hui ne doit pas amoindrir la spécificité des produits qui sont sous indication géographique en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux comme vous le savez, la France a porter le sujet pendant la PFUE et nous sommes ravis que la commission poursuive ceux-là. Elle a présenté en avril, cette proposition de règlement que vous mentionnez, nous avons fait avancer les travaux techniques sur le texte, l'examen se poursuit, je crois que nous partageons les mêmes objectifs et nous serons très très vigilant à ce que les dispositions de ce texte ne soit pas pas affaibli et puis être renforcées, notamment en matière de contrôle et donc je vous serez reconnaissant de nous signaler si ça n'était pas le cas, ou si vous avez des inquiétudes merci. Merci Madame Schillinger c'est bon alors je donne la parole à Madame Marie-Pierre Monier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 4 minutes chers collègues. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, donc mon intervention vient en complément de celle de mon collègue Lucien tension je ne reprendrai donc pas les éléments de présentation de la filière la Cole, j'en viens directement aux difficultés auxquelles elle sort avec de réglementation Reach et CLP emblématique des paradoxes que peuvent porter les réglementations européennes, précisant que, comme nous, les professionnels de la lavande et plus généralement des plantes à parfum aromatiques et médicinales, ne conteste pas le bien-fondé des objectifs de ces réglementations pour aller vite, Ridge instaure un système d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation qui a mis en place une harmonisation des exigences et un meilleur contrôle des substances chimiques, de son côté CLP et de règlements relatifs à la classification à l'étiquetage et en l'emballage qui vise à améliorer l'information sur les substances chimiques mises en oeuvre, selon des calendriers progressif ces réglementations avait déjà donné lieu à des adaptations pour les producteurs d'huiles essentielles dans la Live filière la vendit représente la plus grande partie de la production en France, des révisions doivent d'intervenir dans les prochains mois portant sur l'augmentation du niveau d'exigence des contrôles afin de supprimer les produits chimiques les plus nocifs, et sur une meilleure identification des perturbateurs endocriniens, une nouvelle fois la filière, la vente et plus généralement celle des huiles, c'est essentiel, ce vote ainsi confronté à des dispositions qui ne sont pas du tout adapté d'une part à leurs caractéristiques, celle d'un produit naturel simplement extrait de la plante, grâce à la vapeur d'eau qui passe à travers les grains qui doit être considéré comme un tout, un taux tombe et non réduit à une composition de molécules d'autre part à leur mode de production en petites entités dans des territoires historiques de production constituée de zones de collines de plateaux et de montagne sèche et en à l'usage traditionnel millénaire des huiles essentielles et des plantes en général Patrimoine vivant qui a vocation à être reconnus au titre du Patrimoine culturel immatériel ces inadaptation font peser un risque important sur la survie de la filière, en tous les cas dans des territoires de production historique où les cultures des pépés AM n'ont peu ou pas de substitut possible au delà des emplois Directs de la filière c'est l'ensemble de l'économie des territoires provençaux qui est menacée, car les champs de lavandes font aussi vivre l'apiculture et surtout le tourisme en outre en ne prenant pas en compte les spécificités de la filière des ils essentiel ces réglementations entre en contradiction avec les objectifs affichés par le Pacte Vert européen d'amélioration du bien-être et de la santé des citoyens mais aussi avec la volonté croissante exprimée depuis de nombreuses années par les consommateurs européens d'accéder à des produits toujours plus naturel. Il est donc indispensable pour l'avenir de la filière la que les révision de réglementation Reach et CLP tiennent compte de la spécificité des huiles essentielles de la même manière, la filière doit être aider mon collègue Lucien stand sur ne l'a dit, pour passer la crise de marché qu'elle aura qu'on rencontre et des solutions doivent être trouvées très rapidement, sans cela, cette filière est voué à disparaître, alors même qu'elle est en pleine dynamique de valorisation, en témoignent ses démarches pour trois l'été l'AOP Huile essentielle de lavande de Haute-Provence pour créer un IGP, la vingtaine de Provence ou encore pour lancer une demande de reconnaissance des paysages olfactif et poétique de la au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup, cher collègue, oui, oui, Madame la Ministre non après alors monsieur Jean Michel Arnaud pour le groupe Union centriste, hein, vous avez la parole pour 4 minutes. madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, vous l'avez bien compris par la résonance des interventions dans cet hémicycle, la lavande et l'homme de la Provence si j'emprunte aujourd'hui les mots de Jean Giono, c'est pour défendre un Patrimoine vivant un atout reconnu à l'international, il y a plus qu'une plante la lavande est un symbole notre tissu agricole un savoir-faire ancestral, une entité paysanne, bref un emblème culturel aujourd'hui sa production, tout comme celle des plantes à parfum aromatiques et médicinales, se voit menacée par la révision de de règlement européen sur les produits chimiques, le règlement et le règlement 10 LP en ce sens, je remercie la commission des Affaires européennes, et son président Jean fera pas ici présent, d'avoir permis l'inscription de ce débat à l'ordre du jour et d'avoir également permis à ce que la commission et ensuite, le Sénat adopte une résolution à cet effet, car oui, il s'agit d'un exemple criant du manque de prise en compte des territoires, des savoir-faire des cultures dans l'élaboration de réglementation européenne d'harmonisation si le règlement visent respectivement à sécuriser l'utilisation des substances chimiques vis-à-vis de la santé humaine et l'environnement et à communiquer correctement au consommateur les propriétés et dangers d'une substance si les objectifs en soit recherché par la commission, à travers ces dispositions sont plus que respectable pour même nécessaire, les objectifs et les modalités d'application

le résultat de ces tests conditionne les autorisations de mise sur le marché, ainsi que les modes de commercialisation, toutefois, la nature des tests ne prend pas en compte les réactions chimiques aux Ulis essentiel cette révision prévoit ainsi pour certains dangers d'évaluer les Ulis essentiel en utilisant uniquement les composants sans étudier le produit dans son ensemble la lavande, lavande, hein, les huiles essentielles sont pourtant utilisé depuis l'Antiquité pour leurs vertus les différents du des essentiel de lavande tasser dans leur globalité n'induisent pas à notre connaissance. Des faits graves sur le corps humain, la révision prévoit également des tests scientifiques supplémentaire que les producteurs devront prendre en charge et que ces derniers ne sont pas sûrs de pouvoir supporter pour des raisons économiques, mais aussi de capacités, alors que la lavande et l'avant d'un représentant France 9000 emplois Directs et 17000 points emplois indirects de telles mesures seraient dramatiques pour une filière regroupant majoritairement de petites exploitations et distilleries, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative grâce au Sénat 10 millions d'euros supplémentaires ont été affiliés et à tu as affectées à la filière, le durcissement de ces règlements mènerait inévitablement l'augmentation des prix des Ulis essentiel en en conséquence les industriels pourraient être tentés de substituer aux produits naturels des substances synthétiques contenant du pétrole. Contenant du pétrole menant ironiquement Alain fait inverse que celui recherché par la commission, à noter également que la Commission européenne propose la création d'une nouvelle classe de danger concernant les perturbateurs endocriniens, dont les critères sont en cours de consultation publique jusqu'au 18 octobre prochain dans ce contexte d'incertitude, les professionnels s'inquiètent d'une éventuelle confusion entre les perturbateurs endocriniens et la notion de modulateurs hormonaux laquelle obéit à des phénomènes psychologiques, pour finir imposer de normes restrictives à une filière aussi dépendant du commerce international a pour conséquence de l'exposé une publicité négative qui pourrait ternir sa compétitivité hors prix la simple annonce de révision de réglementation engendrer un vent d'inquiétude juste dans les colonnes du Wall-Street journal. Si dix-huit essentiel était a considéré à tort comme dangereuses et des pictogrammes dissuasif venait d'être imposé sur packaging des produits, les ventes en serait évidemment impacter le Sénat sera toujours là pour veiller sur ses Terres rares et ces territoires, je crois pouvoir dire également que nous attendons du gouvernement qu'il soit, côté des professionnels afin que l'âme de la Provence ne soit pas mise en jachère à jamais, je vous remercie madame la Ministre de vous assurer. du soutien complet du gouvernement tous les faire confondues afin que notre unité puisse porter ses fruits auprès de la commission, mais encore dans quelques jours, je vous remercie. merci, madame la présidente, madame la sénatrice émue, monsieur le sénateur Monsieur le Président, excusez-moi d'abord les permettez-moi de vous rassurer : nous avons évidemment à coeur les intérêts de la filière l'Amandine et de la vente et la Provence et toutes les pertes. Qui sont employées et qui vivent de cette de ces huiles essentielles, permettez-moi aussi de rappeler qu'en ce qui concerne la révision du règlement Reach il derrière un souci de santé publique, parce que comme le disait ailleurs l'ASN Edris Marie-Pierre Mounier, donc il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre l'impact socio-économique et la santé publique et c'est pour ça qu'il y a des consultations et un nouveau ma porte, celle du ministre de l'agriculture de la transition écologique, hein, et de la santé sont bien évidemment ouverte, pour discuter de tout ça, vous avez raison et permettez-moi aussi de souligner que cette révision parce que j'ai j'ai je le sentiment qu'il a une confusion parfois ne demande pas d'exiger l'analyse de chaque molécule des celui-là, mais en revanche des composantes de telle sorte que le pétrole, il apparaîtrait bien évidemment, j'ai entendu votre inquiétude Les huiles essentielles sont naturelles, mais pour les obtenir, on a besoin de processus chimiques et c'est pour ça qu'elle tombe sous le coup de la réglementation Reach, ce que je voulais vous dire aussi qu'un jeu, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, effectivement, quand je dis pas avant fin 2022 je souhaiterais rassurer madame la sénatrice, le projet de révision des règlements Reach devrait être présenté en 2023 par la commission et avec ça, je m'arrête, merci. Madame la Ministre Monsieur Arnaud, vous avez une minute si vous le souhaitez. Oui, le ministre, je vous remercie de cette réponse, elle me convient, pour partie, la consultation, la concertation, nous avons déjà rencontré certains d'entre nous, Marc Fesneau, moi ce que j'attends surtout c'est une coordination ministérielle pour une position française solide dans les discussions que nous aurons le moment venu dans l'unité auprès de la commission, première observation 2ème observation, vous évoquez le fait que nous aurions des molécules qui sont chimique oui effectivement, personne ne le conteste, mais lui, dans sa globalité ne l'est pas, en tous les cas, il faut que vous en fassiez la démonstration et que ce soit fait la démonstration par Bruxelles que elle ne porte pas atteinte à la santé publique et je crois pouvoir dire que, depuis 2 1000 ans que les unités essentielles sont utilisés, il n'y a pas eu hors usage inadéquat de conséquences particulières sur la santé des usagers, enfin, et je me permets une observation de procédure, on est sur un pouvoir réglementaire et le la commission souhaite utiliser un pouvoir réglementaire, il me semble nécessaire que nous puissions conserver un processus purement législatif qui permette au Parlement d'exercer leur contrôle comme le Sénat, le fait ici en position française merci. Si cher collègue, la parole est à monsieur Jean-Claude anglais pour le groupe Les Républicains et pour trois minutes chers collègues.

madame la ministre, monsieur le président, mes chers collègues, l'harmonisation et le plus souvent perçu comme une solution face à la diversité des cadres normatifs des pays membres de l'Union européenne, c'est pourquoi l'uniformisation des droits nationaux, connaît une expansion continue touchant de plus en plus de secteurs, néanmoins je crois important de relever une limite essentiel de cette harmonisation enfin afin de l'illustrer par l'exemple de la généralisation annoncée du Nutri score au niveau européen, un système d'étiquetage nutritionnel à 5 niveaux sur le principe, il est utile de rappeler que l'harmonisation normative, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui ne correspond bien souvent ni à la lettre, ni à l'esprit des traités européens l'étendue temps et l'intensité de l'intégration s'apparente parfois à une voie d'extension du Champ des compétences de l'Union, contrairement à ce que prévoient les traités et au détriment de l'intérêt des productions nationales, il en est ainsi de la généralisation annoncée du score au niveau européen qui résulte de la stratégie de la ferme à l'assiette, publié en mai 2020 par la Commission européenne, qui a annoncé une proposition législative d'étiquetage nutritionnel obligatoire et généralisée pour le 4ème trimestre 2022. Ce qu'on ne peut qu'approuver la volonté louable d'orienter le consommateur vers une alimentation saine, la généralisation du nutriscore à tous les produits et problématique pour 2 raisons principales d'abord, car l'indicateur retenu produira une information tronquée et trompeuse sur certaines productions alimentaires de qualité comme le fromage ou la charcuterie reconnu par des appellations d'origine protégées AOP ou des Indication protégée, IGP, ces produits qui sont au coeur des terroirs et des identités locales pourraient donc bientôt être bruyant, moins bien noté que la l'par l'algorithme nutriscore que les produits transformés ensuite car la généralisation du nutriscore se fait au détriment des territoires et de la variété des productions locales dans les pays membres de l'Union européenne, je pourrai ainsi évoqué les craintes des producteurs de la zone d'appellation roquefort ou celle des producteurs italiens et espagnols de la filière oléicole car l'incompréhension devant cette règle aveugle au territoire se retrouvent dans tous les pays membres, la stratégie de la Commission européenne, disons pas d'harmoniser des droits nationaux qui reconnaissent et protègent chacun la qualité de leur production locale mais bien de promouvoir une nouvelle, nouveau modèle par une une uniformisation juridique européenne à marche forcée, il ne s'agit donc pas d'un d'une harmonisation juridique mais bien d'une uniformisation idéologique pouvant conduire une dérive dangereuse devant ce risque, il est temps que le gouvernement conclure chers collègues ou les consommateurs et les producteurs et qu'ils défendent le terroir et la diversité des productions locales qui font de la culture alimentaire française, que le gouvernement demande l'exemption de certains mots AOP et du nutriscore européen, je vous remercie. Merci madame la présidente chez chez le président, et monsieur le sénateur, la France est en fait favorable à l'harmonisation d'un système d'étiquetage nutritionnel qui soit frontale et harmonisée à l'échelle de l'Union européenne et c'est notamment une priorité comme Marc Fesneau, l'a répété lors du dernier conseil des ministres de l'agriculture le 26 septembre. Et comme vous savez, il y a eu un report, un rapport récent du Centre de recherche conjoints européens qui montrent que les consommateurs apprécient cet étiquetage nutritionnel parce qu'ils y trouvent un moyen rapide et facile d'obtenir des informations. Bien sûr ce système doit être fondée sur des données scientifiques, il doit être solide et ces données doivent être indépendante et la France soutient un système qui évalue la qualité n'a triché, Neil globale des denrées alimentaires avec un code couleur est basée sur des quantités standard qui vont permettre la comparaison entre. Et depuis 2019, la France est mis en place une stratégie d'influence pour promouvoir ce nutriscore au niveau européen et répondre aux d'attaque, vous l'avez souligné de l'Italie, elle, elle y est en effet fortement opposés parce qu'elle juge un impact défavorable sur sa gastronomie et ses produits traditionnels et donc en janvier 2021, nous avons mis en place une gouvernance transnationale du Nutri, à laquelle participent 6 États membres dont la France et qui est constitué d'un comité de pilotage et d'un comité scientifique. Je comprends que vous soyez, préoccupés par le décalage observé entre l'étiquetage nutritionnel mis en place en France, la composition des fromages et notamment lorsqu'il s'agit d'appellation d'origine protégée, c'est pourquoi la France soutient une adaptation de l'algorithme du Nutri score et notamment pour les fromages, et vous savez que cette révision est en cours et qu'il y a une réflexion sur le traitement des produits sous signe de qualité, vous n'avez pas mentionné, mais je suis sûr que vous aviez le roquefort en tête également, et donc nous allons continuer de porter sur ce dossier, une position d'équilibre entre les objectifs d'amélioration de la santé publique et de la préservation de la production des produits locaux, vous pouvez compter sur nous. Merci, merci, madame la Ministre, Monsieur Anglade, donc je donne la parole à Madame Chantal de scène pour le groupe Les Républicains pour trois minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, pas simple d'intervenir en fin de débat parce que je souhaite aussi, Madame la Ministre, appeler votre attention sur le sujet de la restriction, voire de l'interdiction de l'usage du plomb et ses conséquences pour les entreprises du secteur du vitrail depuis 2018 le plan figure sur la liste des substances dites candidates à l'inscription de l'annexe 14 du règlement européen Reach, entré en vigueur en 2007 pour une pour sécuriser l'affaiblirait la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne, à terme, l'usage du plomb pourrait ainsi être interdit d'ici 3 4 ans en Europe sauf à disposer d'une autorisation au coût prohibitif pour les utilisateurs, les métiers du Patrimoine risque de prendre de plein fouet cette interdiction d'interdiction, la restriction de l'utilisation du plomb pour les vitrailliste risque de condamner un nombre important d'entreprises ayant développé un savoir-faire unique, Madame la Ministre, les professionnels de ce secteur sont légitimement inquiets car vous le savez, la fabrication et la conservation du filtrage reste indissociable de l'usage du plomb, élu d'Eure-et-Loir avec le centre international du vitrail à Chartres, je suis particulièrement attentive à l'évolution de la réglementation européenne, bien évidemment, l'enjeu sanitaire et centrale, le plomb est un polluant identifié depuis longtemps les artisans du du vitrail, ont mis en place des protocoles rigoureux garantissant leur sécurité et leur protection vis-à-vis d'une surexposition au plan je ne parle pas des 2 indicateurs du code du travail, rappelé par notre collègue Louis-Jean de Nicolaï. L'ajout officiel du plomb à l'annexe 14 du règlement Reach il sera tout un secteur d'activité ayant développé un savoir-faire unique contribuant à l'entretien, la restauration et la mise en valeur du Patrimoine bâti français, à terme, il pourrait même conduire à sa disparition aussi, Madame la Ministre, je souhaitais savoir quelles mesures le gouvernement va mettre en oeuvre auprès de la Commission européenne pour préserver le secteur du vitrail. Je vous remercie, merci beaucoup, madame la ministre. Merci madame la présidente, merci madame la sénatrice pour votre question, Monsieur le Président, à nouveau, pardonnez, pardonnez-moi de répéter vraiment que nous sommes ouverts pour le dialogue et que nous allons continuer de parler avec tous les acteurs de la filière et nous tous, membres du gouvernement, le ministre de la culture, la Ministre de la transition écologique et moi-même, et nous sommes. Pleinement conscient vraiment des interrogations et des inquiétudes de tous les corps de métiers du Patrimoine et notamment ceux des vitraux que vous avez mentionné ou ceux des des des fabricants d'orgue donc nous suivons vraiment avec beaucoup d'attention l'évolution du du cadre législatif en ce domaine. Il y a eu de consultation une part et chars basée sur des études scientifiques, nous en avons parlé tout à l'heure et une autre par la Commission, assortie d'une consultation publique et qui pèse à la fois les impacts socio-économiques et culturels qu'aurait une éventuelle inscription à l'annexe 14 que vous avez mentionné et bien sûr les éléments sanitaires. L'Agence européenne des produits chimiques ne va pas adopter sa recommandation avant la fin de l'année 2022, et c'est à ce moment-là que la Commission va proposer son projet de règlement, je voudrais insister sur le fait qu'elle ne sera pas tenu de proposer l'inscription du plomb à l'annexe 14 et que si elle devait le faire pardon, l'agence le recommandé, et même si le plan était inscrit à l'annexe 14, ça ne veut pas dire que l'usage de la substance est interdit, comme vous avez des demandes de dérogation ou d'autorisation pourrait être introduite dans les 18 à 24 mois après la date d'inscription. Et ces délais varient en fonction de la décision de la commission et vous pouvez être assuré que si c'était le cas où et jusqu'à ce moment-là, à l'ensemble du gouvernement à nouveau en particulier mes collègues collègues de la culture et de la transition écologique, nous serons mobilisés dans ce dossier, nous le suivons, en lien avec les filières concernées et permettez-moi de répéter que, vraiment, n'hésitez pas à nous faire remonter les inquiétudes et à venir nous voir aussi. Je laisse Madame la Ministre, même de scène merci, la parole est donc à Martine Berthet pour le groupe Les Républicains et pour trois minutes également. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, pour ma part, Madame la Ministre, je vais vous parler du pastoralisme, qui est un savoir-faire ancestral emblématique de l'identité de nos territoires de montagne, aujourd'hui il est malheureusement mis en péril par une forte prédation, faute d'une réglementation européenne et internationale adapté, en effet, le loup est classé comme espèce de faune strictement protégé au niveau européen, selon la directive dite Habitat Faune flore de mai 92 et au niveau international, selon la Convention de Berne, de 1979 si ce cadre réglementaire a permis de protéger sensiblement la biodiversité au sein de l'Union Européenne et nous pouvons nous en réjouir, il a également favorisé la prolifération des grands carnivores, on estime à 17000 le nombre de loups présents sur le territoire européen en France, l'Office français de la biodiversité, là récemment réévalué à 1 millier ou plutôt 3000 ou selon les chasseurs et des agriculteurs, d'après la réalité observée au quotidien, en témoignent les attaques incessantes qui exerce une pression considérable sur des éleveurs passionnés mais épuisés et découragés, parmi eux, beaucoup ne veulent plus faire monter leurs troupeaux dans les alpages, par crainte pour la survie de leurs animaux, certains pâturages ne sont par conséquent plus entretenus et se referme progressivement à terme cette dégradation des paysages posera d'importants problèmes de sécurité, en augmentant les risques d'avalanche d'hiver et d'incendie, l'été, par ailleurs, la multiplication des attaques non seulement sur des ovins et des caprins mais de façon croissante sur des bovins, conduit à une diminution du temps passé par les troupeaux dans les pâturages, voire même de leur taille, certains éleveurs arrêtent leur activité comme tout dernièrement dans le Vercors, derrière ce triste constat, ce sont toutes nos appellations d'origine protégée et nos indications géographiques protégées pour la viande et le fromage qui sont mises en danger le pastoralisme répond pourtant à nos objectifs de consommation locale responsable et durable en contribuant à la fois à notre sécurité alimentaire et au respect du bien-être animal, c'est pourquoi réviser la réglementation européenne et internationale en déclassant Le Loup de la catégorie, espèce de faune strictement protégée pour l'ajouter à celles des espèces de faune protégée est absolument essentielle pour préserver un savoir-faire traditionnel, la qualité, la qualité du travail de nos éleveurs nos AOP et IGP à travers un avis politique de ne devenu pardon résolution européenne le 21 août 2020, le Sénat avait déjà alerté sur les écueils de cette réglementation, en vain, mais à présent, d'autres pays européens réagissent ainsi le 26 septembre dernier lors du conseil Agriculture et Pêche la délégation autrichienne a demandé la révision de la directive Habitat Faune flore avec le soutien de la Croatie, la Finlande, la Hongrie, la Léttonie, la Roumanie et la Slovaquie, Madame la Ministre, nous devons faire bloc à leurs côtés dans nos territoires, nous voulons protéger nos éleveurs nos traditions les nos produits du terroir, pas le loup dont la survie n'est plus en danger. Merci beaucoup, madame la ministre. Merci madame la présidente, monsieur le président, madame la sénatrice est le sujet le loup est évidemment un sujet qui est qui a fait. Bon nombre d'États membres et vous avez raison d'avoir mentionné le conseil des ministres de l'agriculture et tous les pays qui demande à la Commission de réexaminer l'interprétation de la directive Habitat, puisque c'est également le cas de la France, comme vous le savez, et l'objectif pour nous est d'obtenir une souplesse accrue pour organiser une coexistence entre élevage et présence du loup, notamment en en zone pastorale et dans le respect de l'état de converser de conservation de l'espèce. Les résultats du suivi de la population de j'ai j'ai peut être mal compris vos chiffres, en fin d'hiver 2021 2022 pour nous font état d'une poursuite de la croissance de la population, mais un effectif estimé seulement à 921 loup qui est un chiffre largement inférieur au seuil de viabilité génétique de 2500 individus qui n'est pas atteint à l'échelle nationale, en outre, si l'augmentation de la population des loups évidemment une bonne nouvelle pour la biodiversité, comme vous l'avez souligné, elle n'est pas synonyme de dommages accrue au troupeau, au contraire, ceux-ci se sont stabilisées en 2018 et ensuite le nombre d'animaux domestiques tué a connu une légère baisse sur les 2 dernières années, il s'élève à 11000 ovins et caprins, ce qui, je le comprends, reste très élevé, hein, pour La volonté du gouvernement est donc bien de réduire encore le nombre de prédation et ce qui passe en priorité par le déploiement de mesures de protection puisque tous les élevages ne sont pas aujourd'hui protégé ce que nous faisons, c'est de continuer de mobiliser tous les moyens identifiés dans le plan national pour le loup pour renforcer la protection des troupeaux, notamment avec la filière qualité des chiens de protection et l'accompagnement il y a également la mise en place d'un observatoire des mesures de protection pour améliorer notre connaissance de la localisation et des taux de mise en place des mesures de protection et ainsi mieux venir en appui. Oh merci madame la ministre, merci beaucoup, je vous remercie, je suis madame Berthe et vous avez une minute. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, j'entends ce que vous dites, mais je pense qu'il est temps de réactualiser vos chiffres, vous ne me parlez que des ovins et des caprins, or le, le risque est maintenant sur les bovins qui sont de plus en plus touchés et donc ce sont ces bovins qui interviennent le plus dans nos filières à au pays GP fromages et viande, donc c'est vraiment des bovins dont il s'agit et si cela était si simple et si effectivement il y avait des diminutions d'attaque nos éleveurs n'arrêterait pas leur activité, comme c'est le cas actuellement,

puisque les observations locales des chasseurs et des éleveurs font penser plutôt à une présence de 3000 loups en France et pas seulement 900 921 voilà et donc moi je vous parle, surtout, bien sûr, il y a des mesures mises en place, ça ne suffira pas ça. Suffira jamais, en tout cas nos éleveurs se la Strache que l'arrête merci, cher collègue. Je vais maintenant passer la parole à Madame Laurence Boone, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de l'Europe pour cinq minutes, Madame la Ministre. Merci madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires européennes, mesdames et messieurs les sénateurs, je crois qu'il faut que je vous remercie pour ces riche débat et pour l'ensemble de vos questions et je sais qu'elles traduisent des inquiétudes de concitoyens d'artisans, d'entreprises, d'élus locaux quant à la possibilité pour eux de continuer à faire vivre leur savoir-faire et ses savoir-faire, anime les cultures locales et contribuent à la vie économique des territoires, il participe au rayonnement de la France hors de ses frontières, que ce soit le Patrimoine, la gastronomie, d'ailleurs c'est un Patrimoine ou les produits d'artisanat. Et de manière plus personnelle, je souhaitais vraiment vous remercier d'avoir apporté dans cet hémicycle, l'huile de la vente, je crois que nous en avons eu et allemands ont demandé encore voilà le brie de Meaux, celui de Melun aussi et et les pâturages alpins, il témoigne chose de la diversité de la richesse de nos tiroirs sans masquer les situations parfois difficiles de femmes et d'hommes qui les font vivre. Dès le 1er jour de son mandat, comme vous savez de son 1er mandat, le président de la République a fait de l'Europe un réflexe dans la recherche de solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés et ce n'est pas une posture mais c'est bien l'application stricte du principe de subsidiarité consacrée dans notre constitution, comme dans les traités européens parce que. Comme lui, nous croyons que face aux défis en matière de sécurité collective de crise énergétique de prospérité économique de transition vers de protection de la santé comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'échelon européen est souvent le plus pertinent et celui qui nous protège et protège nos artisans, nos éleveurs, le producteur, le mieux, c'est également le cas pour la protection des productions les plus local, que nous vivons dans une économie très mondialisée avec de forces discussion de concurrence et là, l'Europe nous protège le système des indications géographiques et je vous remercie de l'avoir mentionné et Anou précieux outil tant pour garantir la qualité de nos produits que pour en favoriser le rayonnement en France et à l'étranger et c'est pourquoi la France a plaidé, comme je l'ai indiqué tout à l'heure pour la création d'un système d'indications géographiques pour les produits non-agricoles pour permettre aux artisans européens de mieux défendre leur savoir-faire. Et évidemment, je me réjouis que la commission et publié une proposition et que vous l'ayez mentionné, nous la soutiendrons pleinement et en discuteront avec vous pour nous assurer que ce règlement soit bien adapté aux spécificités de nos territoires et à leur production. La question de l'adaptation de notre réglementation européenne aux spécificités de nos territoires et je crois que c'est vraiment l'essence de nos débats aujourd'hui est vraiment essentiel. Et nous sommes dans notre vie courante évidemment de plus en plus en prise avec les réglementations européennes et j'ai bien entendu le message que souvent elles sont perçues, elles sont encore trop souvent, je devrais dire, perçu comme le fruit d'une élaboration lointaine technocratique opaque, mais je vous assure que je veux qu'au quotidien, ce soit le contraire, pour nous tous, acteurs de la vie publique et que les éléments concrets que vous avez apporté aujourd'hui l'association des territoires, des secteurs professionnels dans l'élaboration de réglementation, d'harmonisation qui les concernent soit encore plus vivant et fort que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Bien sûr, nous avons aussi besoin de la participation des citoyens à la vie démocratique de l'Union, le dialogue régulier avec les oscillations représentatives de la société civile, tous sont des principes, fondements de l'Union européenne. Et je crois que ce qui traduit le mieux en fait la vie démocratique européenne, c'est l'association des Parlements nationaux dans l'adoption des textes législatifs comme vous l'avez mentionné cet après-midi, les procédures de pétition ou d'initiative citoyenne européenne les avis du comité de régions du comité économique et social européen et bien sûr tous les rapports que vous avez mentionné, hein, Monsieur le Président en début de votre de cette session et messieurs, Mesdames les sénateurs au fur et à mesure de vos interventions, j'entends vos propositions Monsieur le Président Rapin pour que la vie des parlements nationaux soient toujours mieux pris en compte et la diplomatie parlementaire à laquelle vous êtes très attaché, me paraît à cet égard, et, et, bien sûr, nous vous appuierons en ce domaine également voilà je voulais également vous assurer une dernière fois, que les autorités françaises sont les premières à porter les intérêts des territoires et à défendre les savoir-faire locaux dans le processus décisionnel européen

qui est nécessaire pour un cadre de vie plus sain, mais pour qu'elle se fasse en intégrant vraiment les considérations sociales, économiques et culturelles des territoires, il n'y a pas d'arbitrage à faire concurrence, Madame la Ministre, entre l'objectif de santé publique et la défense de notre Patrimoine, mais au contraire une position équilibrée à trouver et un accompagnement des acteurs concernés à mener, je vous remercie. Madame la présidente, merci madame la ministre. Alors pour conclure le débat, la parole est à monsieur Jean-François Rapin, président de la commission des Affaires européennes pour cinq minutes chers collègues. Merci, merci de me donner cinq minutes je ne sais pas si je les utiliserai, Madame la Ministre, vous auriez pu les prendre, c'est ça, madame la ministre, vous l'avez compris si cette enceinte respire l'histoire elle respire aussi les territoires tous les sénateurs qui se sont exprimés l'ont fait et je pense sincèrement au nom d'un territoire et avec une spécificité qui les honore, mais Madame la Ministre, juste quelques quelques 2,2 points importants à mon avis, à signaler, le 1er c'est finalement toutes les paroles que vous avez porté et qui sont finalement très ambitieuse, volontaire et et qui soutiennent nos propos pourraient se concrétiser avec un exemple tout simple que les institutions européennes pourraient mettre en place la question de la culture peut être et est porté finalement à la fois par les drapeaux des nations mais aussi par leur langue le multilinguisme, me semble quelque chose de très important à respecter dans les institutions, prenons l'exemple de riches qui nous a animés ce soir le rapport riche, c'est à peu près 1000 pages tout en anglais.

Et donc je pense que on pourrait là ne fresques là apporter une impulsion pas seulement française mais multi-linguiste le 2ème point sur l'aspect dérogatoire, vous nous avez fait des précisions, mais je pense qu'on doit aller plus loin et expliquer à nos collègues que finalement l'aspect dérogatoire nécessite quand même un combat, un combat des états parce que, au regard du comité riche qui est constitué d'un d'un membre de chaque État se confronte la Commission et la Commission fait une proposition et ensuite le comité Reach, charge au comité riche de l'adopter ou non à la majorité qualifiée, bien sûr, mais je pense que ça n'est pas si simple et on nécessite d'avoir une volonté forte de l'État, voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire en remerciant tous les collègues de de leur participation, puis vous redire, Madame la Ministre que pour porter ce de façon fier, il est important d'écouter aussi les parlements nationaux, mais je sais que je reçois une bonne oreille de votre part sur le sujet, je veux aujourd'hui et dans mon département du Pas-de-Calais si je n'ai pas évoqué les fromages ou la bière, on doit être aussi fier de toutes ces de toutes ces richesses et dire à ces richesses est assez porteur de richesses que si elles existent, c'est grâce à l'Europe et non pas si elle disparaissait grâce à l'Europe aussi, voilà Merci monsieur le président, alors je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 21 heures 30 pour le débat sur les conclusions du rapport dix, la dernière frontière, la séance est suspendue.